La séance est ouverte. Le compte-rendu intégral de la séance du jeudi 2 février, a été publié sur le site internet du Sénat.

lors du scrutin 122 portant sur l'article 1 de la proposition de loi visant à réhabiliter les militaires fusillés pour l'exemple, durant la première guerre mondiale. Bernard Fiolet aurait souhaité voter pour. Par ailleurs, lors du scrutin 123 portant sur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger. Contre l'occupation illicite Guilaine Pentel Jean-Pierre Corbisez Éric Gold souhaitaient s'abstenir. Merci. Acte est donné de ces mises au point. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l'analyse politique des scrutins concernés. Mes chers collègues, la conférence des présidents inscrit le prochain débat d'actualité à l'ordre du jour du mercredi 8 février à 16h 30. Après concertation avec les groupes politiques ce débat porterait sur proposition du président du Sénat sur le thème suivant quelle réponse européenne aux récentes mesures protectionnistes américaines sous forme de discussion générale d'une heure, y a-t-il des observations. Il en est ainsi décidé. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution exprimant le soutien du Sénat à l'Ukraine, condamnant la guerre d'agression menée par la Fédération de Russie et appelant au renforcement de l'aide fournie à l'Ukraine. Présenté en application de l'article 34 tirer 1 de la Constitution par Monsieur Claude Malhuret. Dans la discussion générale. La parole est à monsieur Claude Malhuret, auteur de la proposition de résolution et pour 10 minutes, Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je voudrais tout d'abord remercier les présidents de groupe et les très nombreux sénateurs qui ont décidé de cosigné cette proposition de résolution. Remercier également le président du Sénat qui lui confère une solennité particulière en demandant lui-même son inscription à l'ordre du jour du Sénat. Un an après l'invasion de l'Ukraine. Nous avons appris plusieurs leçons fondamentales. La première et l'ampleur des mensonges que le Kremlin a orchestré sans relâche depuis des années pour justifier ces agressions successives. L'Occident est responsable de tout le temps menace la Russie soutient des nazis et des criminels de guerre multiplie les provocations. L'Europe et le valet de l'impérialisme américain. Ces discours délirants relayés avec constance par le parti pro-russe en Europe ont trompé. Beaucoup de monde. Ils ont volé en éclats. Le jour ou de juin dernier à Saint-Petersbourg où Poutine lui-même a fini par avouer ce qu'il pense depuis toujours. L'Ukraine et russe et comme autant de Pierre le Grand. La Russie va reprendre par la guerre ces territoires perdus. Balayé la propagande balayer tous les mensonges balayer la fable de l'Occident menaçant. Empire colonial sous les tsars. La Russie veut le dernier empire colonial sous le communisme. Après la fin des empires anglais et français. Elle veut le redevenir. Et l'on comprend aujourd'hui le sens de la phrase prononcée par Poutine en 2005 la chute de l'URSS fut la plus grande catastrophe politique du XXe siècle. Parce que la chute de l'URSS c'était la fin de l'empire russe. La 2ème leçon de cette guerre et que l'ampleur de ce mensonge n'a eu d'égal que l'ampleur de nos illusions et de nos lâchetés. Ce n'est pas l'agressivité de l'Occident qui a conduit Poutine à envahir l'Ukraine, c'est sa passivité. En 2008, les leaders européens ont refusé à l'Ukraine et à la Géorgie, l'adhésion à l'OTAN pour ne pas irriter Poutine. Quelques mois plus tard il envahissait la Géorgie. Quand il a envahi la Crimée. Nous avons un nouveau répondu avec des sanctions bien modeste. Il est clair que les craintes infondées de provoquer Poutine en le convainquant de notre faiblesse ont ouvert la voie à l'invasion totale de 2022. Cette erreur majeure d'analyse fut d'abord celle de l'Allemagne et de la France. Depuis 30 ans la politique allemande est fondée sur la dépendance énergétique à la Russie. La dépendance commerciale à la Chine et le désarmement face aux de celle de la France fut de courtiser la Russie pour trianguler sa relation avec les États-Unis. En espérant acquérir une position indépendante sans en avoir les moyens politiques et militaires. Que signifie puissance d'équilibre quand il y a d'un côté une démocratie qui est notre allié depuis plus de 2 siècles qui nous a sauvés lors de deux guerres mondiales et nous a évité de devenir la province occidentale du Reich allemand ou de l'Union soviétique et de l'autre une crêpe ploutocratie mafieuses qui succède à un régime totalitaire ayant asservi l'Europe pendant des décennies. Les avertissements répétés des Européens de l'Est qui savent eux ce que c'est que l'impérialisme russe ont été rejeté avec mépris comme des agitations de va-t-en-guerre hystérique. L'invasion de l'Ukraine nous montre l'échec de ses de politique et surtout l'urgence à ne pas les poursuivre. L'apaisement et le compromis avec un dictateur n'ont jamais marché le dictateur avance devant la faiblesse et recule devant la force c'est aussi simple que ça depuis toujours. Si l'Europe veut une paix durable sur le continent. Elle doit apprendre le langage de la puissance, le seul que les dictateurs comprennent. La 3ème leçon et le degré de nuisance de bassesse et de complicité du parti pro-russes en Europe et particulièrement en France. Cette 5ème colonne des extrémistes qui cherchent sans relâche à nous désarmés face à un loup qu'il présente comme un mouton qui depuis des années nous avoir je ne répète que Poutine est le plus grand dirigeant du monde. Qui reprennent Motta sur les réseaux antisociaux avec les milliers de faux comptes de trolls et de bottes pilotées depuis Moscou sur les télés RT et d'autres la propagande de Poutine, l'Ukraine n'existe pas, elle est Russe ses dirigeants sont des nazis. Pouchkine. Le grand poète russe disait qu'on nous donne une je nous trouverons les cochons. Ils sont la boussole qui indique sans jamais se tromper. La direction du déshonneur par le chemin le plus sordide. Depuis l'invasion de l'Ukraine. Le Pen la barre honnête des guichets de Moscou et Mélenchon le génuflexions des plus infâme dictature condamne du bout des lèvres, car ne pas le faire serait un suicide. Mais il ne change pas d'avis tout est de la faute de l'Occident, surtout pas d'armes, surtout pas de sanctions, leurs députés européens ont refusé de voter, même l'aide humanitaire à l'Ukraine leurs parlementaires français ont refusé de voter l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN lors du discours du président de la Rada ukrainienne à l'Assemblée mardi dernier, ils ont déserté l'hémicycle pendant que tous leurs collègues étaient debout pour l'applaudir. N'écoutez pas ce que disent les dirigeants des partis de la France russes regarder leur vote regarder leurs gestes et vous comprendrez qu'ils n'ont rien lâché, qui sont toujours en embuscade comme des crapauds blottis sous une grosse Pierre en attendant que passe l'orage. Que faire aujourd'hui. D'abord tirer les leçons de nos erreurs passées, car nous ne les avons pas toutes tirées. Nous nous félicitons à juste titre que l'Europe ne soit pas diviser comme l'espérait Poutine mais unis. Que notre alliance avec les États-Unis et les autres démocraties se soit renforcée que le soutien à l'Ukraine reste constant. Que les opinions publiques horrifiée par les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité chaque jour sur leurs écrans tiennent bon. Mais attention les différences d'appréciation entre Européens de l'Ouest et européens de l'Est et du Nord n'ont pas disparu et chaque étape du conflit, voir réapparaître l'écart entre ce qui se qualifie de réaliste entre guillemets et ce qu'il veuille ta et, plus loin et plus vite les réalistes craignent l'escalade. Il pense qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir chaque épisode de cette guerre prouve qu'ils ont tort, en refusant l'escalade ils en laissent le monopole à Poutine et font perdre à chaque fois les semaines nécessaires à la contre-offensive ces semaines c'est moi. Parfois ce sont des milliers d'Ukrainiens qui meurent les lignes rouges, nous savons désormais qu'elles ne sont que le fruit de nos peurs. Chaque fois que Poutine les traces et qu'elles sont franchies, il ne se passe rien. Comment pourrait-il frapper plus fort alors que son armée minée par la corruption qui ronge son matériel l'incompétence de ses chefs et la défiance de ses soldats et déjà au delà de son maximum est paralysé sur tous les fronts. Quant à la rengaine du danger nucléaire. Poutine laisse désormais Medvedev le Pochard et Lavrov le croque-mort les brandir sur les plateaux des trash télé de Moscou, il a compris depuis la mortifiante réunion de Samarcande. Ouchy et maudit l'ont mis publiquement en piqué qu'elle lui est interdite, même parmi même par ses plus Cessons de nous faire peur avec ce disque rayé depuis 50 ans. Le but n'est pas de permettre à l'Ukraine de résister mais de chasser l'occupant. Si nous avions livrés dès le début, ce que nous nous apprêtons à livrer aujourd'hui. L'Ukraine n'aurait pas seulement reconquis Kharkiv Eckerson mais largement profité dans le Donbass, profitant de la déroute russe, ce sera bien plus difficile maintenant qu'on leur a laissé le temps de se retrancher mais c'est néanmoins un bon signe que de plus en plus de dirigeants européens hier dans le camp des réalistes, soit en train de comprendre que la livraison massive d'armes n'aurait pas eu pour conséquence de prolonger la guerre mais au contraire de l'écourté par la débâcle des envahisseurs. Mieux vaut tard que jamais. C'est maintenant qu'il faut livrer les chars, les missiles, les défenses sol-air et les avions. Si nous voulons comme le promettait le président de la République lors de ses voeux accompagner l'Ukraine jusqu'à la victoire finale. Il est en fait une dernière raison encore plus essentiel de ne pas répéter les erreurs du passé. Les démocraties, au terme d'une lutte implacable ont vaincu au XXe siècle. Les 2 totalitarismes aux dizaines de millions de morts. Certains les croyait disparu à jamais sous nos yeux. L'international des tyrans se reforme. Le boucher de Moscou le génocidaire des Ouïgours en Chine le Docteur Folamour de Corée du Nord le massacreur de femmes de Téhéran et quelques autres se sont regroupés. Leur seul but se venger abattre l'Occident mettre à bas la liberté. La deuxième Guerre froide a commencé et depuis plusieurs années. Beaucoup de dirigeants occidentaux proclame que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. J'espère bien que ce discours n'est que tactique et qu'il n'en croient pas un mot parce que les dictateurs eux l'annonce clairement ils sont en guerre contre nous. Ils veulent achever les démocraties qu'qui croient agonisante. Il n'y aurait rien de pire que de croire que nous ne sommes pas en guerre contre des gens qui sont en guerre contre nous et qui le disent. Quant au reste du monde, il attend l'issue du conflit pour voler au secours de la victoire. Ce qu'il en espérait une certaine sympathie se trompent lourdement. Les dirigeants bien peu démocratique de la plupart de ces pays se moque de savoir si Poutine a violé les lois internationales. Ils ont même pour mantra la justification de leurs méfaits actuels par la condamnation de notre domination passée. L'Europe doit comprendre l'urgence de redevenir une puissance militaire, d'avoir une stratégie commune et de consolider notre alliance avec les autres démocraties du monde, à commencer par les États-Unis. S'ils n'y arriveront pas. Si nous laissons les cinquièmes colonne des fachos des trotskistes, des populistes et des idiots utiles, nous conduire à l'aveuglement et au renoncement. Alors ce n'est pas seulement l'Ukraine demain qui sera vaincu. Mais la liberté. Il est temps de réarmer les démocraties face aux tyrannie du XXIe siècle. Le peuple héroïque d'Ukraine nous en montre le chemin. Je vous remercie. Je vous remercie. Dans la suite de la discussion générale. La parole est à monsieur Jean-Pierre Grand. Pour le groupe. Les indépendants pour cinq minutes. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Sidéré par la brutalité des événements d'Ukraine depuis le 24 février dernier. Nous nous devons de garder la mémoire du temps long. Pour en saisir le sens et la portée. Sachant, ne pas oublier la longue période de dictature et d'oppression du régime communiste dans l'URSS d'alors et l'enfermement de ce régime dans une confrontation toujours plus acharnée. Sachant, ne pas oublier ce qu'ont signifié la chute la chute du mur de Berlin et la partition de son empire, source de nostalgie de ressentiment parmi les dirigeants et ses forces armées. Vladimir Poutine a jamais fait mystère de ses sentiments sur cette page d'histoire qui l'a rappelé en 2005. La plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Remodeler les frontières de la Russie s'inscrire dans l'histoire comme le dirigeant qui lavera les enfants de l'histoire contemporaine à son pays, c'est son obsession. En 2008, Vladimir Poutine a jeté. Son dévolu sur le site, il Afzali. Hein. Géorgie et six ans plus tard sur le Donbass et la Crimée. Le 24 février dernier. L'emballement de l'histoire nous rappela que la Russie n'avait pas renoncé à conquérir l'Ukraine. Dans l'esprit des nationalistes russes. Une victoire militaire en quelques semaines contre l'Ukraine se serait traduite par un triomphe de Vladimir Poutine. Dans cet esprit. Poutine tentent aujourd'hui de réhabiliter Staline pour remotiver le un nationalisme russe confronté aux doutes que lui inspirent les revers de l'armée russe. La réalité est bien là. La Russie est loin d'avoir pu conquérir l'Ukraine et remplacer le gouvernement de Kiev. Vladimir Poutine a sous-estimé la réaction occidentale et en particulier la capacité de l'Union européenne d'organiser son unité pour porter secours à une nation voisine envahi. Les États-Unis par leur envoi massif d'équipements militaires leur aide financière affichent leur soutien moral et politique à l'Ukraine. Vladimir Poutine et ses généraux ont sous-estimé la force et le du patriotisme du peuple ukrainien ses capacités militaires tactiques mécanique et bien sûr le courage, la force politique du président Zelensky, qui a su mobiliser son peuple et obtenir le soutien d'une grande un grand nombre de démocratie. Mes chers collègues. L'indicible de cette guerre ces crimes sa barbarie ces milliers et milliers de morts, la déportation de citoyens et même d'enfants tout cela. L'histoire ne l'oubliera pas. Tôt ou tard les dirigeants russes devront rendre compte. Mais aujourd'hui, chaque Français. Voudraient voir cesser cette guerre aux conséquences désormais ressenti dans leur vie quotidienne. Monsieur le ministre. Beaucoup s'interrogent sur le rôle de la France.

Ne la dispense pas au contraire l'oblige à maintenir une action diplomatique ambitieuse et dans un même temps à livrer de l'armement aux Ukrainiens et en plus sécurisé sa présence sur tous les continents. dans dans dans l'engagement pour la paix n'est plus à démontrer. Seul état de l'Union européenne à disposer d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU se doit de développer une diplomatie de temps de guerre, c'est sa ligne politique de toujours. La France voit de la paix c'est anticiper les cataclysmes, souvenons-nous, il y a 20 ans presque jour pour jour de la position de Jacques Chirac et du discours. Dominique de Villepin à l'ONU contre la guerre en Irak. Le message de la supériorité du droit sur la force reste plus que jamais d'actualité. Aujourd'hui qui peut imaginer que le président de la République sa ministre des Affaires étrangères et notre diplomatie ne sont pas dans la même stratégie de lucidité pour aider à jeter les bases d'une paix durable en Ukraine sans renier ou affaiblir le soutien occidental à cette nation martyre et encore moins l'amener à renoncer à ses frontières reconnues par l'ONU par les Nations-Unies cette sale guerre menée par la Russie s'étend aussi dans le même temps auprès des pays émergents dont les peuples vivant dans la pauvreté sont une proie facile pour Vladimir Poutine et sa milice Wagner. Les récents coups d'État militaires en Afrique facilite le retournement contre la France des populations abusées une déstabilisation de l'Afrique conduira mécaniquement à l'exode de ses populations vers le continent européen. Voilà une arme redoutable, imaginé par le Kremlin pour déstabiliser l'Europe. Déstabiliser la France pour l'heure l'Afrique pour déstabiliser l'Europe c'est aussi cela la guerre que nous mène vers Vladimir Poutine. Enfin une autre conséquence de la guerre en Ukraine et la stratégie russe que la France doit gérer avec ses partenaires dans sa diversité, sa complexité, c'est le risque du retour d'un sentiment politique quand on l'Occident qui ne manquera pas là aussi de créer de multiples problèmes de tous ordres aux 4 coins du monde.

Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il y a près d'un an jour pour jour. Vladimir Poutine plonger l'Europe et le monde dans le chaos en agressant son voisin ukrainien. Un an plus tard, le bilan de cette invasion, devenue une guerre de tranchées d'un autre âge et terrifiant. Alors que les soldats se battent dans la neige et le froid glacial de l'hiver continental. Le conflit aurait déjà fait plusieurs centaines de milliers de victimes dans plusieurs dizaines de milliers de civils ukrainiennes et ukrainiens. La Russie qualifiée par le Parlement européen d'État promouvant le terrorisme de devra répondre de ses crimes. Qu'il me soit permis à cette tribune de renouveler au peuple ukrainien. Notre hommage le plus vibrant et d'autres admiration devant l'immense courage qui est le sien. Nous admirons tant le courage des militaires qui défendent la ligne de front, pied à pied face aux vagues des mâles des malheureux conscrits russes envoyés à la mort, que le courage des civils vivant à l'arrière, sous la menace des bombes et des drone qui prennent des vies et détruisent des infrastructures civiles pour plonger le pays dans le noir, le froid, la soif et la solitude de l'hiver. Un an plus tard, le bilan de cette guerre et déjà planétaire. Crise énergétique, inflation, pénurie alimentaire. L'économie mondiale qui était à peine sortie de la pandémie de Covid-19 est de nouveau plongé la tête sous l'eau. Les perspectives à court terme sont alarmantes. Le Programme alimentaire mondial des Nations unies considèrent que nous sommes face à la pire crise alimentaire depuis la fin de la 3ème de la 2ème Guerre mondiale, plus que jamais nos efforts de coopération doivent être décuplés pour éviter de mettre sur les routes des millions d'affamés. Un an plus tard, nous remercions le groupe les indépendants Libertés et territoires et son président, Claude, Claude Malhuret, même avec certaines de ses outrances déplacé de proposer un autre examen cette proposition de résolution pour exprimer le soutien du Sénat à l'Ukraine, cette guerre a trop duré. Nous devons tout faire pour atteindre son terme cela passe pas un renforcement du soutien à l'Ukraine pour lui permettre de repousser l'envahisseur russe et de recouvrer ses frontières de 1991. On peut légitimement s'en inquiéter et le déplorer, mais aucune autre alternative n'est sur la table. La France recevez la semaine dernière Monsieur Rouslan Stefantchouk, président le Dorada Rada qui nous a présenté la situation suivante, soit nous livrons à l'Ukraine davantage d'armement de pointe pour lui permettre de percer à nouveau le front et d'avancer vers l'Est soit la guerre va inévitablement s'enliser dans un meurtrier conflit de trancher où périront tant de soldats. Que la Russie a en nombre supérieur. Si cette guerre s'étire sur plusieurs années, les conséquences seront désastreuses pour l'Ukraine et pour le monde entier. Aussi nous sommes favorables à ce que la France et ses alliés renforcent leurs efforts en matière de soutien militaire, financier et de ravitaillement. À ce titre, nous demandons solennellement au président de la République de livrer quelques chars Leclerc à l'Ukraine. Au-delà de son efficacité militaire que nous savons limité. Cette décision est indispensable. Politiquement elle doit garantir à nos alliés que la France est à leurs côtés dans toutes les décisions importantes que cette guerre exige de nous. Dès à présent se posera la question de la fourniture d'avions de chasse demandée par le président Zelensky. La plus épineuse. À ce jour. Ayant constaté le grand sang-froid dont font preuve le pouvoir politique et l'État-Major ukrainien. Nous croyons possible de fournir collectivement des chasseurs à l'Ukraine, sans risquer de les voir utilisées à d'autres fins que la défense de son territoire. Aussi, nous invitons les partenaires Atlantique a entamé a entamé par où des discussions en ce sens. Nous saluons le nouveau paquet de sanctions annoncées par la présidente de la Commission européenne et nous appelons comme le demande le président ukrainien a et inclure les dirigeants de Rosatom à défaut de pouvoir nous passer de l'uranium enrichi en Russie pour notre fourniture électrique. Nous saluons la décision historique de la Norvège d'allouer une aide pluriannuelle de près de 7 milliards d'euros à l'Ukraine, tant pour le soutien immédiat aux pays que pour sa reconstruction future et nous invitons la France et l'Union européenne à agir dans le même sens. Cela doit aussi inclure. Une aide matérielle aux besoins logistiques immédiat, notamment l'envoi de groupes électrogènes. Enfin pour finir sur une perspective optimiste. Nous saluons les progrès réalisés par l'Ukraine dans son chemin vers l'adhésion à l'Union chemin que nous souhaitons le plus court possible. L'une des causes de ce conflit, c'est justement la volonté de l'Ukraine de rejoindre l'Europe, comme nous l'avons été depuis un an, nous devons nous nous devons d'être indéfectiblement à la hauteur de cet idéal de liberté et de démocratie que des flans le peuple ukrainien. Voilà, mes chers collègues, nous adopterons naturellement cette résolution et souhaitons que le vote de notre assemblée soit unanime. Merci. Merci Monsieur le Président. La parole est à monsieur André Gattolin pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes faisait indépendant pour six minutes. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en préambule à mon propos je veux tout d'abord remercier très chaleureusement notre collègue Claude Malhuret, qui a apporté cette initiative. Nous connaissons tous ici sa vigilance de longue date à l'endroit du régime de Vladimir Poutine. Les propos fermes et constant qu'il tient à ce sujet, ici au Sénat depuis 2014, l'honneur et indirectement honore notre assemblée. Au dollar. Je tiens également à saluer l'ampleur du soutien qui s'est déjà exprimé en faveur de cette proposition de résolution et en particulier son caractère éminemment transpartisan puisque pas moins de 5 présidents de groupe s'en sont cosignataires ce quasi-consensus est d'autant plus remarquable que les termes employés par cette proposition sont ferme précis et sans équivoque. C'est il est vrai, le moins que nous puissions faire face tes cette agression horribles perpétrés à l'encontre de l'Ukraine, cette guerre hybride et de haute intensité, avec son cortège inouïe d'exactions et de crimes de guerre dont la liste s'allonge malheureusement chaque jour davantage. Ce texte arrive aussi à un moment clé du conflit. Pas seulement parce que nous approchons du 24 février, date anniversaire du début de cette guerre. Non, nous sommes à un moment clé parce que contrairement à ce qui avait et prédisent certains commentateurs le fameux général hiver n'a pas gelé ce conflit, bien au contraire les combats redoublent d'intensité dans des zones qui s'étendent au du sud de Zaporijjia au nord de Bakhmout. Certes nous ne disposons pas de chiffres officiels, mais on évalue à au moins 120 150.000 morts le nombre de soldats russes qui ont été tués et à plus de 100.000 le nombre d'Ukrainiens, civils et militaires ayant connu le même sort. Le moment est clé car après une phase de reconquête entamée par l'Ukraine à l'Automne passé, nous sommes désormais dans une guerre de positions où les forces ukrainiennes sont sur la défensive tant les moyens humains déployés par la Russie sont importants. Les moyens militaires de l'Ukraine, en dépit de l'aide prodiguée sont insuffisants pour tenir sérieusement une ligne de front qui à l'Est s'étend sur plus de 1500 kilomètres et à laquelle il faut bien sûr ajouter les 900 kilomètres de frontière avec la Biélorussie, où le régime de monsieur Loukachenko définitivement vassalisée par le Kremlin fait figure de complice de celui-ci. Condamné fermement l'attitude de la Russie qui dans tous les domaines, rompt avec le droit international le droit humanitaire et le droit de la guerre est indispensable. Oleksandra Matviïtchouk présidente du Centre des libertés civiques, déclarait il y a 10 jours devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, que son organisation, je le rappelle, lauréate du prix Nobel de la paix en 2022, avait recensé documenté plus de 31.000 crimes de guerre perpétrés par les troupes russes et encore ne s'agit-il là que des crimes possiblement ressent sable car il en est certain dans les territoires de l'Est de l'Ukraine annexées ou occupées par la Russie qui ne peuvent être ni documenté ni précisément quantifiée. C'est la raison sans doute pour laquelle, en dépit de leur extrême gravité plusieurs de ces crimes sont si elliptique évoqué dans cette résolution. Je pense en particulier à la situation de centaines de milliers d'enfants qui ont été déplacés de force vers le territoire russe, osons le mot, c'est bien une déportation de masse sans précédent en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale qui est à l'oeuvre les médias propagandistes russes regorge le reportage louanges en c'était l'an deux soi-disant solidarité humanitaire de famille risque qui adopte spontanément ces pauvres orphelin de guerre orphelin qui en réalité disposent souvent encore de parents en Ukraine. Fait et le Kremlin ne s'en cache hier il procède à ce qu'il appelle la dénazification des territoires occupés en des Ukrainiens les déportés en procédant à leur russification. C'est à travers leur changement de nom, voire même d'origine à l'état civil, bien plus qu'une épuration ethnique constitutive en soi déjà d'crimes contre l'humanité. Ce procédé honteux visant à éradiquer l'identité d'enfants et à les prendre en otage s'apparente à un acte constitutif d'un véritable génocide aussi au delà de cette résolution en faveur de laquelle mon groupe le groupe RDPI se prononcera unanimement. Je voudrais conclure mon propos en interpellant notre haute assemblée sur une question qui jusqu'à présent n'a guère fait l'objet de son attention. On le sait. Rome ne s'est pas construit en un jour le pouvoir autoritaire de Vladimir Poutine non plus son attitude n'a pas soudainement basculé dans la nuit du 23 au 24 février 2022 qui a entraîné son pays dans cette guerre ignoble. Depuis 15 ans au moins. Des signes avant-coureurs jalonnés de 100 préfigurait déjà les charniers que nous commençons à déterrer aujourd'hui. Pourquoi n'avons pas vu venir cette guerre et la dérive démocratique et bellicistes de son principal artisan, avons-nous été aveuglé où nous sommes nous laisser aveugler. L'argument de l'imprécis Vidy imprévisibilité et de l'irrationnel IT supposée de Vladimir Poutine, Poutine a bon dos pour expliquer les erreurs d'analyse stratégique que nous avons commises. À l'heure où de multiples travaux de retour d'expérience sur cette guerre sont engagés. Je crois qu'un peu d'introspection sur nos faiblesses passé ici ne serait sans doute pas inutile. Je vous remercie de votre attention. Merci cher collègue. La parole est à monsieur le président Patrick Kanner pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 9 minutes. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Voilà 349 jours. La Fédération de Russie a décidé sur ordre de son président Poutine l'invasion d'un autre pays souverain, l'Ukraine en violation du droit international, cela fait 349 jours qu'un peuple souffre. Cela fait 349 jours qu'un peuple est bombardé. Cela fait 349 jours qu'un peuple se bat pour sa liberté. Et au travers libertés la nôtre. Au Sénat depuis presque un an, nous avons suivi l'évolution de la situation et nous sommes réunis, nous nous sommes réunis à de multiples reprises, encore la semaine dernière. Nous avons entendu les mots. Forts du président de la Rada Rouslan Stefantchouk qui disait. On nous tue par le froid et l'obscurité. Et un autre moment de la journée, il nous avait dit. La Russie a volé un an de la vie de l'Ukraine. Ces mots ne peuvent pas rester sans écho et je salue donc l'initiative du président du groupe les indépendants Libertés et territoires, qui a initié cette proposition de résolution, en 1er lieu de regarder derrière nous et de tirer un 1er bilan de cette année de guerre en Europe afin de tracer les perspectives qui devront conduire vers une paix victorieuse pour l'Ukraine et les Ukrainiens. Le 26 octobre dernier, nous avons eu un débat très riche, très fort. Nous avons condamné. Dénoncé cette invasion et ses conséquences, notamment à l'égard des populations civiles. Nous avons condamné une invasion et des exactions contraires au droit international. Nous n'oublierons pas. Boutcha, Irpin, Marioupol et toutes les autres villes martyres. Nous nous sommes inquiétés des conséquences collatérales pour l'Europe et pour le monde, particulièrement en matière d'énergie et de sécurité alimentaire. Nous nous sommes interrogé sur les risques d'usure que fait peser cette guerre une usure qui pourrait atteindre la solidarité et le soutien des pays et de leurs concitoyens à la cause de l'Ukraine. Ces quelques mois qui nous séparent de ce dernier débat permette de faire un certain nombre de constats et de tirer quelques leçons. Le 1er de ces constats et que le soutien à l'Ukraine reste non seulement indéfectible mais il se renforce dans l'opinion malgré l'inflation malgré les coûts de l'énergie, nos concitoyens n'ont pas fléchi et l'adhésion à l'Union européenne s'est même renforcé. Les pays européens, les alliés ont non seulement continuer à faire preuve de solidarité. Mais il ne cesse de renforcer leur aide. Qu'elle soit financière, militaire ou diplomatique et l'Union européenne a su démontrer ses capacités de ressources pour affronter les turbulences. Nous ne devons pas relâcher l'effort et continuer à relever collectivement certains filles. Qui n'ont pas encore été traitée. J'y reviendrai. Le second constat et que le soutien en termes de matériel notamment a produit des effets. L'armée ukrainienne a pu mettre à son actif une reconquête d'une partie de ces territoires. L'armée russe détenez 24 4 % du territoire ukrainien en mars 2022. Aujourd'hui, il n'en contrôle plus que 18% chez modeste mais c'est une avancée. Les premiers responsables en sont bien sûr les Ukrainiens dont le courage et la combat, dit-il, la combativité continue aujourd'hui d'être à l'oeuvre sur les différents fronts, on pense notamment à Bakhmout, où les combats sont particulièrement violents et à d'autres zones où la situation reste très fragile. Enfin, l'escalade de temps crainte n'a pas eu lieu. En tout cas pas sous la forme que certains prédisaient la seule escalade, que l'on observe et celle de la violence utilisée par l'armée russe à l'encontre du peuple ukrainien. changé. Nous avons observé un changement de nature de la stratégie russe qui s'est mise à cibler délibérément systématiquement les infrastructures critiques ukrainiennes et les populations civiles. Dans une fuite en avant à caractère mortifère. Contraire à toutes les lois. Cette stratégie ne peut que renforcer notre détermination à nous tenir aux côtés des Ukrainiens. Alors oui, les infrastructures nous aideront à les reconstruire. Alors oui, les populations, nous continuerons à les soutenir et j'réussis une pensée, mes chers collègues. Pour les Français qui sont encore en Ukraine. Certains, dans l'est du pays sous les bombes, notamment à Kharkiv. Ils ne sont pas partis qu'à leur vie là-bas leur attaches familiales sont là-bas. Certains n'ont pas les capacités financières pour partir et les contacts nécessaires en France pour le faire, il ne faut pas les oublier. Monsieur le ministre est à leurs côtés pour répondre à leurs éventuelles demandes. Cette résolution nous amène à nous interroger sur les prochaines étapes nécessaires pour aboutir à sortir de ce conflit. Personne sur ces bancs, comme partout ailleurs, personne ne veut la guerre. Nous recherchons le retour à une situation pacifiée. Mais de nouveau être clair sur un point. Quitte à nous répéter et à nous rend répéter il nous pouvons viser autre chose que la victoire de l'Ukraine sur son agresseur russe. Je l'ai déjà dit ici, je le répète, aucun traité ne saurait être arrachés par la force. C'est d'égal à égal, sous la protection de l'ensemble de la communauté internationale, rassemblés au sein de l'ONU que l'Ukraine et la Fédération de Russie doivent définir les modalités de leur coexistence. Même si nous savons qu'elle sera difficile notamment dans les premiers temps une fois, nous l'espérons la paix retrouvée. Car tout démontre que c'est dans un rapport de force, y compris militaire avec Poutine que la voie de la diplomatie pourraient être pour être pardon. Lui seul nous oblige à réagir, hein. Chine, ne l'oublions pas. Pour atteindre ce but. Il convient de saluer le saut qualitatif de l'aide militaire des chars seront fournis. Avec le temps nécessaire pour cette livraison, ils seront un renfort de poids pour la. Mais l'armée ukrainienne des avions pour l'être également la stratégie ukrainienne reste et doit rester une stratégie défensive que nous devons soutenir par ces moyens. Elle a toujours été parce que c'est l'Ukraine qui à la nation agressée et c'est l'Ukraine qui doit pouvoir se défendre. Un renfort d'autant plus nécessaire que la Russie a des ressources. Que ce soit en termes de matériel comme de soldats. On ne connaît pas encore les effets de la massification de son armée sur une éventuelle future offensive à la fin de l'hiver. Ou au début du printemps. Comment depuis le début de la guerre. L'aide européenne doit être combiné. Avec des sanctions pour l'économie russe. Il convient de saluer le nouveau paquet de sanctions annoncée par Ursula von der Leyen. Pour le 24 février prochain, date. Anniversaire entre guillemets. Si l'on peut dire de l'invasion. Dans ce cadre la résolution cite notamment la Biélorussie. Qui fait partie de l'équation. N'oublions pas non plus, c'était un vassal du régime de Moscou et ayons une pensée pour les opposants biélorusse emprisonné ou exilé. Comme le texte l'évoque. Nous devons combiner notre action avec une réflexion plus poussée qui pourrait aboutir à des enquêtes sur des faits susceptibles de constituer des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. L'Europe travaille sur différentes pistes en ce sens la France. Monsieur le Ministre devra prendre toute sa part dans ce cadre. La guerre vous oblige à l'humidité. Comme la résolution nous y invite, plusieurs questions restent à trancher, au niveau français à l'échelle européenne et au sein de l'OTAN et je voudrais les partager avec vous, mes chers collègues. Comment établir le basculement stratégique. Comment reprendre l'Avantage dans le cadre d'une stratégie défensive. Comment reconstruire l'Ukraine. Sur ce dernier point, la France devrait y participer aux côtés de ses partenaires à ce stade le classement en zone rouge de l'ensemble de l'Ukraine par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères empêche les entreprises françaises d'y participer, il faudra y travailler. Cette humilité, nous devons également l'appliquer à la France cette guerre interroge nos certitudes et nous devons, dès aujourd'hui, dès aujourd'hui, réfléchir ensemble sur les capacités militaires qui nous permettent de protéger notre pays sur la réaffirmation de notre place dans le sur la place de la France sur le continent européen et au niveau international ou encore sur nos capacités économiques et industriels cette réflexion doit s'inscrire à l'échelon national mais aussi dans le cadre européen ce sont des chantiers importants. Mes chers collègues. Pour conclure. Nous ne devons pas craindre Vladimir Poutine. Quand celui-ci souligne qu'à travers l'Ukraine. Il fait la guerre à l'Occident. Monsieur Poutine est un prédateur. Il profitera de chacune de nos faiblesses et ses provocations verbales lors de la célébration de la victoire de Stalingrad jeudi dernier ont pour terreau l'exaltation d'un patriotisme agressif soyons forts sachant résister. Oui c'est un prédateur. À l'extérieur de ses frontières. Comme à l'intérieur de ses frontières. Le peuple russe comporte aussi son lot d'opposants à la guerre, ceux qui ne veulent pas que leurs enfants se fasse dévorer par le nationalisme. Ceux qui ne veulent pas que la dictature s'étendent sur le monde

La résolution que nous discutons arrive à un moment crucial pour l'avenir du conflit et pour celui de la paix mondiale. Hier le secrétaire général de l'ONU s'est alarmé je le cite, que le monde se dirige les yeux grands ouverts vers une guerre plus large encore, mettant en garde contre les risques d'escalade. Allons-nous entendre. Chers collègues, cette mise en garde. Il y a un an l'agression militaire déclenchée par Vladimir Poutine a plongé dans l'horreur. Le peuple ukrainien et signé le retour d'une guerre inhumaine au coeur de l'Europe. Le bilan est d'ores et déjà effroyable probablement plus de 300.000 victimes tuées ou blessées un pays durablement meurtrie. Des millions de réfugiés et de déplacés internes. Vladimir Poutine croyait gagner la guerre. En un éclair, la résistance de l'Ukraine et des par la France et l'OTAN a changé la donne. Face à cette résistance qu'il n'attendait pas. Vladimir Poutine a choisi le pire toujours plus de guerre, crimes de destruction de violation des droits humains d'enrôlement forcé de jeunes Russes sans compter le chantage plusieurs fois brandi de la menace nucléaire. Ce choix du pire a provoqué en riposte un armement massif de l'Ukraine. Un peu plus tard. Malgré cet effrayant bilan des moyens colossaux engagés de part et d'autre et une ligne de front globalement figé depuis des mois, la guerre ne s'apaise pas mais semble au contraire à l'aube d'une nouvelle escalade. Et cela en dépit du constat dressé par le général Mac Mark Milley, chef d'État-Major des armées des États-Unis le 9 novembre 2022. Estimant, je cite, il doit y avoir une reconnaissance mutuelle que la victoire n'est probablement pas réalisable par des moyens militaires et qu'il faut donc se tourner vers d'autres moyens. J'entends aussitôt la critique admettre admettre ce constat ce serait hein d'y être indifférent au drame ukrainien ou pire se montrer complice de Vladimir Poutine, le président de la République lui-même Emmanuel Macron a été confronté à cette accusation larvée quand il a tenté de maintenir ouverte la porte d'une négociation sommet alors de rentrer dans le rang des partisans de l'escalade guerrière. Non, cher collègue affirmés notre soutien à l'Ukraine contre l'agression militaire de la Fédération de Russie. Dénoncer les crimes de Vladimir Poutine exigé le retrait des troupes russes et le respect de la souveraineté, élu de l'Ukraine des militairement et humanitairement l'Ukraine à se défendre et à protéger sa population. C'est indispensable, comme nous le disons depuis le 1er jour de la guerre mais cela de loi aller de Pair avec l'impératif de prévenir une guerre généralisée. Est allée de Pair avec une mobilisation internationale de tous les instants pour stopper le conflit pour explorer toutes les voies capables de remettre les belligérants à la table de négociations en vue du retour à la paix et à la sécurité mutuelle abandonner l'objectif de la paix au seul profit de l'escalade militaire, c'est abdiquer devant la perspective d'une guerre longue et durable toujours plus destructrices une guerre aux limites inconnues chaque jour plus proche d'un basculement aux conséquences incalculables. Ce travail est urgentissime chers collègues ne voyons-nous pas s'accumuler les vents mauvais d'une guerre toujours plus large. La Russie ne recule devant rien pour envoyer la jeunesse russe à la boucherie. Face à lui le surarmement des pays de l'OTAN s'accélère dans des proportions inédites. Les ventes d'armes à l'international des États-Unis ont dépassé les 200 milliards de dollars inondant l'Europe d'armes toujours plus sophistiqués. Les dirigeants polonais pas à proprement parler des figures de la démocratie ont augmenté le budget militaire de 9 milliards de d'euros en 2015 à 97 milliards en 2023 à grands coups d'équipements américains. Les surenchères nationalistes et les réécriture de l'histoire se propage partout et en tous sens excitant Les and des peuples. Au même moment. Ne voyons-nous pas excusez-moi, des périls encourus européens ayant traversé 2 guerres mondiales. Avons-nous perdu la mémoire. Voilà pourquoi, chers collègues, nous ne voterons pas la résolution qui nous est proposé. Elle énonce des rappels de principes que nous défendons nous-mêmes face à l'agression criminelle de la Russie, mais elle ne propose face à ce drame qu'un seul chemin de fait l'escalade militaire clairement revendiqué par l'auteur de cette proposition de résolution Claude Malhuret. C'est le sens de l'alinéa 31. Autrement dit après les chars lourds porteur d'obus à uranium appauvri. Des avions de chasse demain des missiles et à chaque renouveau des soldats formateurs de l'OTAN directement engagée. La résolution donne en fait, le feu Vert au franchissement futur de toutes les lignes rouges et surtout, elle fait l'impasse sur tout appel à une initiative de négociations et de paix. Ce n'est pas un oubli, c'est un choix, celui de la guerre comme seul chemin possible, oubliant la leçon de tous les conflits récents. Cette résolution est une occasion manquée je conclut d'une phrase, celle de faire rimer solidarité avec l'Ukraine et mobilisation pour une solution de paix. C'est cette double exigence qu'exprimera notre vote contre. Merci la parole est à madame Nadia Sollogoub pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur l'ambassadeur. Mes chers collègues. Depuis un an les auditions menées par le groupe d'amitié France-Ukraine que je préside ne parle ni d'échanges culturels ni de partenariat économique. Les auditions que nous menons sont des récits d'horreur de souffrance et de terreur des récits de courage et de résilience à chaque entretien. Nous promettons de porter des messages je remercie donc Claude Malhuret, qui me donne aujourd'hui l'occasion de le faire une tribune qui ne fera pas la mienne mais celle de ceux qui souffrent et nous appelle au secours. Ce sera aussi la tribune d'un groupe d'amitié qui n'a jamais relâcher ses efforts. Le 23 mars 2022. Nous étions une vingtaine devant l'ambassade de Russie à Paris nous porte sur un message simple exigeant le respect des termes de la Convention de Genève, signé par la Fédération de Russie. Nous demandions d'urgence des corridors humanitaires pour les populations civiles. Nous portons les signatures de 170 d'entre vous, sénateur de France. Nous n'avons pas été reçus traiter avec le plus grand des mépris. Le 7 février 2023. Nous exigeons de nouveau le respect des règles essentielles du droit humanitaire international. Le respect des populations civiles. Le traitement loyal des prisonniers de guerre le libre accès aux organisations humanitaires internationales et tout particulièrement à la Croix-Rouge. Le 2 novembre 2022. Nous avons auditionné celle que nous on appelle les femmes d'Azov dont les époux les père les fils ont défendu Marioupol jusqu'à la limite de leurs forces retenu désormais dans des endroits tenus secrets. Privés de nourriture, de soins. Ils sont sans contact avec leur famille que cette résolution leur prouve que nous ne les oublions pas et que nous partageons les preuves de cette inhumaine angoisse le 29 octobre 2022. Nous recevions Madame Hadewijch, Prix Nobel de la paix avocate qui dirige le Centre pour les libertés civiles, elle recueille des témoignages pour documenter les crimes de guerre on ne documente, pas seulement les violations des Conventions de Genève, explique-t-elle. On documente la souffrance humaine chaque jour hélas elle entend le pire, nous devons lui promettre que ces dizaines de milliers de récits ne seront ni vin ni perdue et qu'un tribunal international dédié rendra sa justice. Le 19 avril 2022. Les responsables de l'UNICEF témoigner des souffrances des enfants en temps de guerre en Ukraine tout particulièrement les enlèvements massifs d'enfants vers la Russie déjà ne faisait plus de doute, même si leur décompte manque encore de précision. Nous devons par cette résolution, les dénoncer vigoureusement à cette occasion des chiffres nous ont été rappelés en 1914 90 % des victimes de la guerre était militaire 10% été civils de nos jours la proportion s'est inversée et désormais dans un conflit où l'un des deux belligérants ciblent intentionnellement les populations civiles. Le nombre de femmes, d'enfants et de vieillards. Parmi les victimes est intolérable. Par cette résolution, chers collègues dénonçons une dérive inhumaine. Je voudrais aussi avoir une pensée pour nos collègues députés de la Rada d'Ukraine qui travaillent chaque jour et sans relâche parfois sous les attaques des bombes par exemple ou de Mila Buimister, qui au lendemain de l'agression du 24 février témoigné par visio-en gilet pare-balles demander des casques et supplier l'Europe de fermer le ciel voici quelques-unes des voix que je porte au nom du groupe d'amitié chaque jour de guerre est un jour de trop à la gare de Kiev, un grand nombre de jeunes gens chaque jour partent pour le front et une file d'ambulances récupère les blessés. C'est d'une tristesse infinie. Nous souhaitons tous que cette guerre cesse au plus vite, mais c'est aussi notre rôle et notre devoir d'exiger tout de suite le respect des valeurs essentielles de la France, pays des droits de l'homme. Enfin je dois vous dire chers collègues au fil des auditions mon Andrej russophones se familiarisent avec l'ukrainien. Un mot revient dans chaque phrase et j'ai fini par le comprendre Peter IMCA Peter le soutien. L'Ukraine a besoin de notre soutien de notre soutien sans faille à chaque instant. Le président Stefantchouk nous a dit la semaine dernière la question pour s'affoler. Une année de notre vie. Hé bien, mais vous avez aussi changé, oui nous avons changé. Et nous avons appris le sens du mot soutient je vous remercie. remercie. Alors la parole est à monsieur Jean Louis Masson pour 3 minutes, chers collègues. Monsieur Masson, je passe la parole à Monsieur le Président, Ruquier. Non, Monsieur Masson, je vous remercie de d'aller un peu plus vite, merci. La.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues. Je voterai contre ce projet de résolution pour 3 raisons. Premièrement en organisant un blocus économique contre la Russie et en fournissant des armes ainsi qu'une aide financière à l'Ukraine, les pays de l'Union européenne et de l'OTAN sont devenus des cobelligérants. Notre boycott du gaz, du pétrole et des matières premières russes est ainsi la cause de l'inflation et de la crise économique que nous subissons. Nous nous sommes donc pénaliser nous-mêmes. Deuxièmement, on ne peut pas faire de reproche à la Russie. Si dans le même temps, on laisse faire et même on cautionne une agression encore plus scandaleuse contre un autre pays. Or, l'OTAN et l'Union européenne n'ont rien fait lorsque l'Arménie a été attaqué par les 2 dictateurs d'Azerbaïdjan et de Turquie. Pire, on est même allé jusqu'à doubler nos achats de produits pétroliers à l'Azerbaïdjan. Ce qui ne peut qu'encourager sa politique d'agression. Quant à la Turquie. Nous soutenons un pays dont le dictateur se réjouit du 1er jet génocide contre les Arméniens et qu'il a actuellement une politique doublement génocidaires. D'une part contre les turcs contre les Kurdes et d'autres par contre les Arméniens. Si c'était la Russie qui avait attaqué l'Arménie, l'OTAN et l'Union européenne aurait réagi très vigoureusement. C'est bien la preuve que l'OTAN a des arrière-pensées. Enfin troisièmement. Nous sommes actuellement dans la même situation qu'à la veille de la première guerre mondiale. À l'époque l'Allemagne n'était pas la seule responsable de cette guerre car les pays de l'entente soutenez la Serbie et les terroristes serbo- bosniaques qui ont assassiné l'archiduc d'Autriche. Aujourd'hui la guerre en Ukraine est en apparence liée à l'agression de la Russie. Mais elle résulte aussi de l'extension vers l'Est de l'OTAN et de l'Union européenne, ce qui conduit à encercler littéralement la Russie. Les États-Unis n'ont jamais accepté que l'Union soviétique puisse installer des fusées à Cuba. Pourquoi voudrait-on que les Russes acceptent aujourd'hui d'être encerclée par l'OTAN. En voulant mettre la Russie à genoux le temps prend le risque irresponsable d'un conflit nucléaire, tout comme la première guerre mondiale, cela pourrait nous faire des dizaines de millions de morts, aussi bien d'un côté que de l'autre. Ceci étant, je suis je compatis avec la situation aussi bien de tous les Russes qui sont morts dans cette guerre que de tous les Ukrainiens, mais je crois qu'il y a une lourde responsabilité des pays occidentaux dans cette affaire. démocratique et social européen pour cinq minutes chers collègues la président. Mais madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes à quelques jours de la date tragique. De l'anniversaire de la gestion portée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine.

Face à cela, depuis des mois, ça se résigner s'affaiblir les Ukrainiens reste debout. Malgré a dû retirer les combats dans l'est de l'le de l'Ukraine, malgré le déluge des bombes qui fera la population civile. Au coeur de Kiev. Les Ukrainiens et le président Zelensky, force le respect Le courage du peuple ukrainien n'est plus à démontrer. Il a désormais valeur d'exemple. Il s'écrira certainement ou l'histoire Boutcha, Marioupol Bakhmout ou encore Solidar sont quelques-unes des vies de symboles d'une résistance acharnée. Ce sont aussi des villes martyres.

Comme l'a très justement souligné. Le président de la République de la Rala ukrainienne. L'Ukraine est devenue le bouclier qui protège l'Europe et l'ensemble du monde civilisé c'est une c'est évidence et qu'il y en a de plus en plus fortement la France et la communauté internationale. Il ne s'agit plus seulement de la. Souveraineté d'un territoire envahi mais bien d'un combat et collectif pour rétablir les règles élémentaires de l'ordre mondial. Mais Israël jusqu'à la rentrée. Depuis quelques jours sa position. Tant le macabre dessein stratégiques russes. A bouleversé tous les équilibres stratégiques dans ces conditions. Comme le souligne la proposition de résolution. L'aide fournie à l'Ukraine doit être accentué sur tous les fronts. Le front des sanctions, bien entendu. À cet égard. Mon groupe s'est réjoui doit arriver hein Didier, un paquet de mesures annoncées par Bruxelles. Pourvu qu'elles appliquent elles affaiblissent l'industrie de défense russe. L'Union européenne doit toutefois se pencher. Sur la question des contournements qui affectent la réalité d'une partie des sanctions. Quant au front militaire. La nécessité d'un effort constant des livraisons d'armes aux forces ukrainiennes apparaît désormais incontournable. On peut le rejeter certaines par l'escalade l'amorce n'a ouvert son les rôles comme le sait si bien la propagande russe jusque sur le continent africain qui a gravi les marches de l'horreur sous couvert d'une prétendue opération spéciale. À ce stade, nous savons qu'une clef d'une des clés de la victoire ukrainienne réside la défense anti-aérienne. Mon groupe entame de la France et qu'elle contribue à consolider les sur l'de l'Ukraine un complément du soutien militaire américain est significatif. c'est ce qu'ils vont à la réserve qui consiste à préserver le territoire russe des attaques et les missiles. Quant au front diplomatique. Doit-on y croit encore, nous avons espéré jusqu'à la veille du 24 février 2022, Alain Aujourd'hui hélas des des négociations de paix semble. Ne semble pas envisageable à. Déçu pour ne pas dire humilié par son insuccès militaires. Enfermé dans une spirale paranoïaque Vladimir le redoutable continue d'organiser son armée dans une logique de guerre. Un changement de général.

Comme organisation terroriste leur brutalité et sans équivoque et on ne doit par ailleurs s'inquiétait. De leur développement sur le continent africain. signataires de la proposition de loi de Claude Malhuret. Les membres du du RDR sur la moto en toute logique, nous espérons apporter notre modeste contribution au combat du monde libre.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes sur un sujet Affaires étrangères et avant de vous parler de l'Ukraine. Je voudrais que nous ayons une pensée forte et aussi exprimer notre solidarité, notre soutien aux populations syriennes et. Victimes du séisme de ce week-end. depuis un an. L'actualité internationale et dominée par cette guerre en Ukraine, à l'initiative de la Russie. Russie, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations-Unies. Membre de l'OSCE et du Conseil de l'Europe notamment. Autant dire que la Russie n'ignore rien des principes du droit international. Et pourtant les autorités. Les autorités russes n'ont pas hésité à déclencher une violente opération militaire contre un État souverain, l'Ukraine baptisé pudiquement opération spéciale, elle est en fait une vraie guerre d'invasion visant à la conquête de territoires au remplacement d'autorité légale démocratiquement élu à la mise au pas du peuple ukrainien. Et à la mainmise sur l'économie et l'agriculture. Ce coup de force illégale. Nous ne pouvons pas l'accepter. Ce serait la fin de l'ordre international et le retour à la loi du plus fort. Dans ce contexte, l'initiative de notre collègue Claude Malhuret est à saluer. Et enfin, adresse un message fort et clair du Sénat. Nous avons d'ailleurs reçu ici même il y a quelques jours une importante délégation ukrainienne conduite par le président de la Rada précédés d'ailleurs par un entretien avec le Ministre de la Défense ukrainien. Quelles que soient les causes invoquées par les autorités russes à la pluie de leur politique belliqueuse. Il reste que dans ce conflit. Il y a tout de même un agresseur et un agressé. L'Ukraine est un État souverain dont l'intégrité territoriale doit être respecté. Et les règles du droit international ont été volontairement ignoré par la Russie. Ce conflit brutal déciment les civils ukrainiens détruit des installations vitales race des villes et aboutit à l'occupation illégale de territoires. Pire encore, une partie des opérations et sous-traitée à des mercenaires recrutés dans des prisons russes, ainsi qu'à des forces tchétchènes dont les méthodes sont destinées à terroriser. En déplacement en Ukraine avec le président Larché, et quelques collègues nous avons vu in situ cette sale guerre dans laquelle les exactions sont commises quotidiennement contre des civils sans compter les missiles qui ciblent les habitations. Des comptes devront être rendues par les responsables de ces actions criminelles, contraire à toutes les lois, y compris contraires aux lois de la guerre. C'est le sens de cette proposition de résolution le conflit art arrive ravivé la peur sur le continent européen qui après 2 guerres mondiales se croyait à l'abri dans sa bulle de prospérité économique. L'économie européenne est désormais victime des effets collatéraux de cette guerre effets collatéraux qui s'étendent jusqu'à la rive sud de la Méditerranée et même au-delà, l'Europe a aussi dû faire face à un flot historique de réfugiés. Ainsi, je le crois. Les Européens ont eu tort de considérer les questions stratégiques comme secondaire quand d'autres États renforcer leurs outils de puissance et diversifier leurs modes d'action. Les inquiétudes les plus fortes s'expriment chez les voisins immédiats de la Russie ou la confiance, vous le savez n'a jamais véritablement régné ce fut la neutralité contrainte de la Finlande. Également le rideau de fer qui ajoute à l'Europe qui ampute et un certain nombre de pays traumatisé par cette expérience ont souhaité rejoindre l'Union européenne et l'OTAN. Les vagues successives d'élargissement ont porté l'Union européenne et l'OTAN aux frontières russes avec des conséquences géopolitiques peut être mal anticipé même nié parfois par certains, il s'agissait en effet de l'adhésion à un projet politique et économique européen. D'un côté et à une alliance militaire menée par les États-Unis de l'autre cette occidentalisation rapide de territoires longtemps liés à la Russie leur passage sous protection américaine n'est pas un changement anodin mais à l'époque, on croyait fermement. Peut-être à tort à la fin de l'histoire entre guillemets et à l'affaiblissement durable de la Russie. La politique européenne de partenariat oriental conçu au départ comme la création d'un cercle d'amis je cite est devenue plus ambigu pour les Russes, l'Union européenne travaille dans leur arrière-cour pour l'Union européenne, au contraire, les pays du Partenariat oriental, sont des pays souverains. C'est exact et qui compare librement les offres et leur liberté de choix doit être respecté. Au final, le projet d'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine. Les velléités ukrainienne d'adhérer à l'OTAN, ont donné lieu à la réactivation de tensions avec la Russie et à l'enchaînement de faits tragiques. Au cours de cette période, je crois que les Occidentaux ont peut être mal appréhender les ressorts du fonctionnement russe. D'abord le puissant complexe obsidionale historique qui aujourd'hui tourne à l'obsession, voire à la paranoïa, surtout pour des dirigeants formés dans l'appareil sécuritaire soviétique. Tout le narratif russe s'appuie sur ce sentiment d'encerclement de marginalisation qui justifie les investissements massifs dans le domaine de la défense, les actions militaires à l'extérieur. De plus, les Russes ont le sentiment avec les larges Isman successives d'un abus de faiblesse commis au moment où leur pays était au plus bas. Alors aujourd'hui où allons-nous quels sont nos objectifs, aider l'Ukraine à se défendre, récupérer la Crimée changer le régime à Moscou. Ces objectifs sont-ils partagés par tous les soutiens à l'Ukraine est en mesure-t-on bien toutes les conséquences. Toutes ces questions mériteraient une réponse claire des autorités françaises et européennes. Car l'émotion si légitime soit-elle, ne peut pas et ne peut en aucun cas être notre boussole. Beaucoup de choses ont été faites en matière de dénonciation de la Russie de sanctions et d'aide à l'Ukraine un nouveau paquet de sanctions contre Moscou est en préparation. C'est une bonne chose. Nous avons aussi livré des équipements individuels des munitions du renseignement du matériel de guerre tels que des systèmes d'artillerie. Le débat récent porte sur l'envoi de chars légers ou lourds en quelle quantité. Cette évolution doctrinale comporte nombre de difficultés d'ordre stratégique opérationnel et politique. Et déjà, les autorités ukrainiennes réclament des avions, on peut le comprendre. Le président Macron annonce que rien n'est interdit par principe on peut l'entendre aussi. Mais si une telle montée en puissance se confirmer, ils seraient de plus en plus délicat de se déclarer extérieurs au conflit et à être. Comme telle, il faut bien le mesurer. Malgré ces mesures et les dernières annonces. Nous ne voyons pas d'inflexion des autorités russes. Au contraire. Nous assistons à une radicalisation des discours à l'émergence sur la scène politique de personnages inquiétants, comme il l'a fait durant la Seconde Guerre mondiale ou plus récemment en Tchétchénie. Le pouvoir russe mise sur le stock. Sur le temps long, pardon dans une guerre de saturation. Une guerre d'attrition grâce aux immenses stocks accumulés et au peu de cas fait des vies de ses soldats, surtout lorsqu'ils viennent des confins de la fédération et enfin l'économie russe résiste au FMI. Et ce même FMI prévoit pour 2024 une croissance pour la Russie supérieure à celle de la zone euro. Comprenne qui pourra. Nos sanctions et nos moyens militaires contingenté même technologiquement supérieur suffiront-ils à changer la donne. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller face à une puissance dotée. Nous sommes désormais sur un terrain glissant. Les opinions publiques commence à s'interroger, y compris aux États-Unis. La question du contrôle des armes livrées et du bon usage des aides est aussi un sujet majeur. Par ailleurs, cette situation malheureusement fait le jeu de la Chine et des États-Unis. Je constate aujourd'hui combien il est judicieux pour les Chinois d'avoir mis en place des outils financiers alternatifs permettant d'échapper aux sanctions occidentales et qui peuvent être proposées à leurs alliés comme la Russie. De plus, les entreprises russes se tournent vers le One pour leur contrat et cette pratique pourrait durablement s'ancrer en janvier 2023, la Russie a annoncé que la relance du marché des changes allait permettre de privilégier le One pour ceux des de la risée je cite ces rapprochement russo-chinois dans de nombreux domaines doivent donc là aussi nous interpeller l'Europe pourrait se trouver cornérisé dans de grands axes, Chine, Russie, d'une part et États-Unis et leurs angles leurs alliés anglo-d'autre part, la Chine se garde bien de soutenir ouvertement la l'invasion russe, sans pour autant la désavoué non plus. Et déjà à travers ce conflit et la politique de sanctions qui ont d'école la division du monde prend corps entre le camp occidental et le reste du monde autour d'un pôle russo-chinois tandis que l'ONU et de plus en plus marginalisée. En raison des sanctions les difficultés financières de la Russie ses besoins en biens équipements haute technologie la rapproche encore plus de la Chine. Quant aux États-Unis après la période de Trump. Assez désastreuse pour leur image internationale l'évacuation difficile non concertée de Kaboul. Ils ont amorcé un réengagement en Europe malgré la primauté accordée à la zone indopacifique la faveur de la guerre en Ukraine dans toute l'Europe les achats sur étagères de matériel américain se multiplient à l'avenir. Ah la la terme l'avenir de l'abbaye aide européenne et notamment française est en jeu. Si les Européens à juste titre ont montré une certaine unité une vraie fermeté face à la Russie. Je ne suis pas sûr à ce stade qu'ils aient gagné en crédibilité dans la mesure où la plupart d'entre eux considèrent que seule l'OTAN et les États-Unis sont en capacité de les protéger l'Europe puissance est encore loin et Washington n'a aucun intérêt à une trop grande autonomie politique et militaire européenne. Alors pour la France, le chemin de crête est étroit, tout en gardant ouverts les canaux de dialogue, il semble important de maintenir une ligne de fermeté vis-à-vis de l'agresseur russe de poursuivre le soutien au peuple ukrainien, mais également de porter une attention plus soutenue aux actions indirectes menées par la Russie en Afrique francophone et dont nous sommes la cible, le moment venu il faudra aussi aider en lien avec nos partenaires à la reconstruction de l'Ukraine aux réformes nécessaires, notamment en matière d'état de droit et de lutte contre la corruption et aussi d'économie. Nous voterons donc cette proposition. Je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Cadic, pour le groupe Union centriste pour 4 minutes.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Voilà près d'un an. La Fédération de Russie a décidé d'envahir l'Ukraine. Mes premiers mots seront pour la population ukrainienne et sa résistance admirable face à la barbarie de l'envahisseur. L'occasion nous est donnée avec cette résolution transpartisane du président Maluret de réaffirmer le soutien du Sénat envers l'Ukraine. Une semaine après avoir ovationné ici. Le président de la Rada ukrainienne. Anne de Kiev reine des francs, il y a près de Milan aurait toute sa place parmi les femmes illustres qui ornent le jardin du Luxembourg. En érigeant sa statue. Le Sénat pourrait rappeler ainsi les Liens indissolubles qui unissent l'Ukraine à la France. Ce soutien à l'Ukraine. Nous avions voulu la portée avec le président Maluret en nous rendant à Kiev, le 20 avril dernier, quelques jours après que les Russes soient chassés de ses environs. À Irpin, Borodianka Boutcha. Ville martyre, où les Russes ont commis des massacres. Nous avions découvert un cadre indescriptible de ruines. Ou même les statuts avait reçu une balle dans la tête. À Boutcha, avec des enfants. Nous avions planter des arbres pour rappeler que l'espérance le bien et nos valeurs l'emporteront au final. Ces enfants ukrainiens connaissent désormais les abris la terreur des bombardements. Leur regard vide et triste me hante. Je suis revenu d'Ukraine avec la conviction que tout doit être entrepris pour arrêter cette guerre. En détruisant les infrastructures énergétiques, de nombreuses villes. L'armée russe utilise l'hiver et le froid comme une arme pour faire céder la population. Les frappes incessantes sur les immeubles, les hôpitaux ou encore les écoles et les crèches constitue une véritable stratégie de la terreur à l'encontre des Ukrainiens. Doux déplorons des dizaines de milliers de civils morts ou blessés. La cruauté de monsieur Poutine peine à trouver ses limites. Un Crime impuni est un crime récompensé selon la formule de mail M. Khalaf un député libanais, qui occupe son parlement depuis 20 jours aujourd'hui avec sa collègue Najat Saliba afin d'exiger l'élection du président libanais. Que prévoit le gouvernement et l'Union européenne pour que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par la Fédération de Russie soit jugé et leurs auteurs punis. Depuis un an, la France se tient aux côtés de l'Ukraine avec ses partenaires européens. Dès le début du conflit, des trains de sanctions ont été décidées à l'encontre de la Russie pour affaiblir sa base économique la privé de technologie et de marché critique et réduire sa capacité à faire la guerre à ce jour, l'Union européenne a décidé de 9 trains de sanctions intégrant également la Biélorussie et l'Iran pour l'aide qu'ils apportent à la Russie. Ce dont nous nous félicitons. Fidèle à sa devise Unie dans la diversité, l'Union européenne a démontré la volonté d'agir ensemble pour relever les défis. La Pologne a affirmé un rôle de Leadership avec les États baltes et la Roumanie pour mobiliser l'Union européenne et ne pas tergiverser. L'aide de l'Union européenne, que ce soit en matière de protection civile par son soutien aux forces armées ukrainiennes. A contribué à soutenir la résistance héroïque du peuple ukrainien face à son envahisseur. Soyons-en fiers. Nous pouvons également participer à la reconstruction économique ukrainienne en facilitant le retour des investisseurs. Il faudrait pour cela. Monsieur le Ministre, changer la couleur rouge à l'ouest du pays. De la carte conseils aux voyageurs. Pour accompagner la l'Ukraine dans sa lutte pour sa liberté et sa défense et la défense de nos valeurs. Nous devons aller plus loin dans nos livraisons d'armes. Le président a annoncé vouloir aider à renforcer les systèmes anti-aériens en Ukraine. Pouvez-vous nous préciser si le sujet a été évoqué lors du sommet Union européenne-Ukraine, le 3 février dernier. Comme vous l'aurez compris, le groupe Union centriste votera pour cette résolution. Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Becht. Ministre délégué chargé du commerce extérieur de l'attractivité et des Français de l'étranger. Merci beaucoup madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs. La proposition de résolution aujourd'hui débattue de votre assemblée porte sur un enjeu. Particulièrement important pour la France et pour l'avenir du continent européen. L'agression russe de l'Ukraine déclenchée le 24 février peu après 8 ans de conflit larvé. Et d'ingérence militaire russe en Ukraine a vu le retour de la guerre inter-. De haute intensité en Europe impliquant un État doté de l'arme nucléaire. Par cet acte, d'une extrême gravité. La Russie a franchi toutes les limites et violé les règles régissant les relations internationales depuis 1945. Notamment les principes fondateurs de la charte des Nations unies que sont la souveraineté des États et le respect de leur intégrité territoriale. Cette invasion les objectifs mis en avant pour Moscou. Pour justifier sa prétendue opération militaire spéciale et l'annexion illégale de quatre régions ukrainiennes à l'issue de simulacres de référendums démontre si besoin était, la volonté russe de nier l'existence d'une Ukraine en tant que nation indépendante et libre de choisir son destin. Alors que nous approchons du premier anniversaire de cette agression barbare injustifié et injustifiable. Force est de constater que la Russie n'a en rien abandonner ses objectifs et qu'elle cherche à soumettre la nation ukrainienne par la force militaire. Malgré les revers sérieux qu'elle a connu, retrait de la région de craie de Kiev au printemps dernier. Offensive ukrainienne réussie dans la région de Kharkiv en septembre. Abandon de Kherson en novembre, seule capitale régionale qu'elle avait conquise et prétendait avoir annexé la Russie poursuit son agression avec une violence sans limite. Elle exerce aujourd'hui une pression extrême dans le Donbass, où elle a réussi à progresser dans le secteur de Bakhmout, sans la moindre considération pour ses propres soldats qu'elle utilise comme de la Chair à canon. Seule la Russie est responsable de la poursuite des hostilités en Ukraine, alors que l'Ukraine a montré sa disponibilité à travailler à une paix juste et durable à travers le plan de paix en 10 points présenté par le président les Zelensky que la France soutient. La Russie poursuit par ailleurs sa stratégie lâche et cynique visant à détruire les infrastructures essentielles de l'Ukraine afin de mettre le pays à genoux. Depuis le début du mois d'octobre des salves successives de missiles et de drone visent les infrastructures électriques et gazières ou de distribution d'eau nécessaires à la survie de la population civile pendant l'hiver. La dernière salve a eu lieu le 26 janvier, le jour où la Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Madame Catherine Colonna visiter la ville d'Odessa, qui a été touché. L'objectif russe éclair. Désorganisé l'arrière-ukrainien et semer la terreur parmi la population pour infléchir la résistance de l'Ukraine à l'agression. Ce ciblage systématique de la population civile. La ministre la rappeler cela ne s'apparente pas à faire la guerre. C'est faire des crimes de guerre. Dans ces circonstances, la résistance dont font preuve depuis près d'une année. L'armée et la population ukrainienne forcent notre admiration. En conjuguant la bravoure et la détermination de ses soldats aux équipements sophistiqués que nous lui avons livré. L'Ukraine a montré qu'elle était capable de résister et de repousser l'envahisseur russe. Nous le redisons, la Russie ne parviendra pas à briser la résistance du peuple ukrainien. Celui-ci se bat pour sa liberté et dans cette lutte. L'Ukraine n'est pas seul. Nous nous tenons à ses côtés et nous continuerons de le faire pour l'aider à retrouver son intégrité territoriale et sa souveraineté. C'est ce message de soutien indéfectible qu'apporter aux autorités ukrainiennes la Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Madame, Catherine Colonna, lors de sa visite à Odessa, le 26 janvier. C'est ce même message que le président de la République a transmis au président de la Rada et au ministre ukrainien de la Défense la semaine dernière. Dès le début de cette agression que nous avons cherché à éviter jusqu'aux dernières heures, la France s'est placé du côté du respect du droit et de la liberté en apportant son plein soutien à l'Ukraine dans l'exercice de sa légitime défense. Ce conflit, nous le savons ne se réglera pas intégralement par les armes. Il faudra à un moment se mettre autour de la table et négocier. Mais ce moment n'est pas venu et ce sera à l'Ukraine et à l'Ukraine seule de décider quand et à quelle condition elle souhaitera le faire. Nous avons donc consenti un effort considérable de livraison et d'équipements militaires et nous continuerons de le faire afin de mettre l'Ukraine en position de force pour recouvrer son intégrité territoriale. La décision du président de la République de livrer des chars légers début janvier à initier une dynamique positive. Parmi nos partenaires et ouvert la voie à la livraison de matériel cruciaux pour les forces armées ukrainiennes. De nouvelles annonces françaises ont été faites par le président de la République et le ministre des armées. À l'occasion de la visite du menu du ministre ukrainien de la Défense à Paris, le 31 janvier. Nous allons fournir à l'Ukraine 12 canons Caesar qui s'ajouteront aux 18 déjà fourni. Nous allons poursuivre notre soutien dans le domaine anti-aériens fourniture d'une batterie ASM PTI conjointement avec l'Italie. D'un radar GM 20 et de missiles pour les batteries anti-aériennes Crotale. Essentielle pour protéger la population civile ukrainienne. Des frappes russes. Nous travaillons également à des solutions pour fournir à l'Ukraine des munitions de nouveaux véhicules blindés du carburant et pour assurer le maintien en condition opérationnelle des équipements livrés et assurer un ravitaillement en carburant. Nous avons participé au lancement de la mission militaire européenne eux-mêmes et le ministre Sébastien Lecornu a annoncé que nous formerions 2000 soldats ukrainiens sur le territoire français d'ici l'été tandis que 150 militaires français se rendront à la fin du mois en Pologne pour former jusqu'à 600 soldats ukrainiens par mois. Nous sommes également l'un des plus importants contributeurs à la Facilité européenne de paix qui apporte un soutien en équipement militaire létal inédit au niveau européen. nous avons mis en place un fonds bilatéral que vous avez porté à 200 millions d'euros pour que l'Ukraine puisse se fournir en matériel auprès de notre base industrielle et de technologies de défense. La France et donc comme les Ukrainiens le disent eux mêmes, un soutien de 1er plan à la fois par l'ampleur des montants mobilisés par la fiabilité du matériel qui est fourni et par la rapidité avec laquelle elle parvient à répondre aux besoins exprimés par Kiev. Mais notre. Ne se limite évidemment pas au domaine militaire. Nous consacrons au total plus de 2 milliards d'euros à l'aide civile à l'Ukraine. Face aux conséquences humanitaires dramatiques des frappes russes contre les infrastructures ukrainiennes. Nous avons organisé le 13 décembre à Paris la conférence solidaires du peuple ukrainien afin d'aider l'Ukraine à passer l'hiver 47 États et 24 organisations internationales ont répondu présents et ont promis plus d'un milliard d'euros d'aide d'urgence, qu'il s'agisse de dons matériels ou de financement dans les domaines de l'énergie de l'eau de la santé de l'alimentation et les transports. La France a pour sa part annoncé un effort total de 125 millions d'euros pour les seuls mois de l'hiver. L'intégralité de cette somme aura été engagées au 15 février, ce qui correspond, rapporté à la fenêtre calendaire à l'effort humanitaire le plus important jamais déployée par notre pays. Cette aide aura un impact concret sur la vie de milliers d'Ukrainiens victimes de la stratégie russe visant à faire de l'hiver, une arme de guerre. Pour vous donner des exemples concrets 63 générateur haute puissance sont en train d'être livrés en Ukraine. En plus des 100 déjà livrés début décembre, ainsi que 5 millions d'ampoules LED qui permettront de réaliser d'importantes économies d'énergie. L'effort total dans le secteur humanitaire s'élève à 200 millions d'euros en faveur de l'Ukraine et des pays limitrophes notre centre de crise et de soutien amener plus de 40 opérations pour un total de 2700 tonnes d'aide acheminée. Nous avons également apporter un soutien précieux aux juridictions ukrainienne et internationales en matière de lutte contre l'impunité. C'est l'une de nos priorités car il n'y aura pas de paix durable en Ukraine sans justice. Nous avons apporté un soutien aux enquêtes ukrainienne de la CPI et d'Eurojust afin de contribuer à la collecte des preuves de crimes de guerre. Nous avons aussi envoyer 2 équipes de médecins légistes et de gendarmes de lierre À Boutcha en avril et dans la région de Kharkiv fin septembre et fait don de de laboratoires d'analyses ADN nous participons, réflexion sur la poursuite du crime d'agression qui a initié l'Ukraine dans le cadre du corps, groupe qui s'est réuni à Prague, les 26 et 27 janvier dernier et nous accueillerons la prochaine réunion de ce groupe à Strasbourg fin mars. Nous sommes OPCI mobilisées pour apporter une aide financière à l'Ukraine, à titre bilatéral et au niveau européen et participer à l'effort de reconstruction à plus long terme qui se structure sous l'égide de la plateforme de coordination des donateurs mise en place à Bruxelles par le G7. Parmi nos 2 milliards d'euros d'aide nous avons octroyé un prêt budgétaire directe de 400 millions via l'AFD est fléché 1,2 milliard vers des garanties à l'export qui bénéficie à de large spectre de projets économiques. Essentiel à la reconstruction de l'Ukraine. Un exemple concret, celui de la plateforme numérique. De la modélisation de la reconstruction de l'oblast de Tchernihiv. Porté par 3 entreprises françaises. Enfin nous poursuivons nos efforts visant à accroître les difficultés de la Russie à financer sa guerre d'agression par l'adoption de nouvelles sanctions. Celles-ci sont une preuve de l'unité européenne, les États membres ont réagi avec une rapidité sans précédent. En adoptant les premières mesures. 48 heures après l'invasion russe. Nous avons depuis lors adopté neuf paquet de sanctions sectorielles comme individuel au niveau européen mais aussi bâtit des coalitions avec nos partenaires du G7 et l'Australie afin de plafonner le prix du pétrole russe. Ces sanctions ciblées et proportionnées portent leurs fruits. Comme en atteste la baisse du prix du pétrole brut russe depuis la mise en oeuvre. De ce dispositif de plafonnement. Dans la perspective de l'adoption d'un dixième paquets de sanctions dans les prochaines semaines. La France prépare de nouvelles initiatives visant à entraver le fonctionnement de l'économie de guerre russe et à sanctionner ces responsables. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Vous le voyez. Le soutien de la France est totale, il engage l'ensemble de l'État français mais mobilise au-delà des collectivités, les ONG, les entreprises et je le sais parfaitement votre haute assemblée. Le soutien que nous apportons à l'Ukraine. C'est notre devoir. C'est notre honneur et ce sont évidemment nos valeurs. Les valeurs d'une République qui s'est bâti sur la défense du droit et de ses libertés. Le vote de la proposition de résolution aujourd'hui soumis à votre examen le confirmera, j'en suis persuadé. Ensemble, nous tenons debout. Sans faiblir, aux côtés de l'Ukraine et nous continuerons aussi longtemps qu'il le faudra à le faire, je vous remercie. je vous remercie. Alors nous allons. Procéder au vote sur la proposition de résolution, la conférence des présidents, a décidé que les interventions des orateurs Valais. Explications de vote. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe les indépendants. Il va être procédé au scrutin public d'un conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter. Le scrutin clos. Ah oui.

Alors j'ai donné les résultats du du scrutin merci nombre de votants donc 344 un nombre de suffrages exprimés, 340 pour l'adoption 324. Contre 16, le Sénat a adopté. Je vais suspendre la séance quelques instants pour permettre à chacun de s'installer. Pour l'examen du prochain point à l'ordre du jour, la séance est suspendue.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème automobile tout électrique 2035 est réalisable. Et la parole et tout d'abord à l'orateur du groupe, qui a demandé ce débat.

vous avez la parole pour le groupe Les Républicains pour huit minutes.

Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. En juillet 2015 la commission d'enquête sénatoriale présidée par notre collègue le sénateur Jean-François Husson. Évalué le coût économique et financier de la pollution de l'air pour la France entre 67 et 98 milliards d'euros par an. À ce chiffre s'ajoute le bilan humain. Selon le ministère de l'Écologie. Il s'agirait de 48.000 décès prématurés par an 9% de la mortalité en France. En octobre dernier, le Conseil d'État a condamné l'État français a payé de nouvelles astreinte de 10 millions d'euros. En raison du dépassement des valeurs maximales fixées par les directives européennes. Le trafic routier et responsable de 28% des émissions totales de gaz à effet de serre en France, dont la moitié, proviennent des véhicules des particuliers. Aussi la transformation du secteur automobile est certainement un élément clé de la transition climatique. Encore faut-il que la restructuration de la filière soit réfléchi dans son ensemble et les objectifs assignés réalisable. Depuis les années 2000, la filière automobile française réduit ses capacités de production nationale, le solde commercial des échanges extérieurs du secteur est passée d'un excédent de 13 milliards d'euros en 2004 à un déficit de 15 milliards d'euros en 2019. Dans le même temps, l'industrie automobile allemande augmenté son excédent commercial de près de 30 milliards d'euros. La filière automobile a également subi une succession de crises conjoncturelles. Avant la crise sanitaire, la filière constructeurs comme l'équipementier fournisseur représenter environ 400.000 salariés. Plus de 10% des exportations de biens pour trois quarts à destination de l'Union européenne et plus de 20 milliards d'euros de valeur ajoutée. La crise sanitaire a eu un impact significatif sur l'industrie automobile, avec une diminution de la production en France et une chute des exportations en 2021, la sortie de crise a été perturbée par les difficultés des fournisseurs à s'approvisionner en matières premières et en composants électroniques. Cette année là 11 millions de véhicules n'ont pu être produit. En octobre dernier, le chiffre de avec le 5 millions était avancé pour 2022. Enfin dernièrement il y a eu la guerre en Ukraine et la crise énergétique. Parallèlement à ces crises conjoncturelles, la filière fait face aux défis de la décarbonation en développant depuis 2018 l'offre électrique le 8 juin 2022 a été franchi la première étape vers la fin au sein de l'Union européenne des véhicules thermiques. Le Parlement européen en effet voté la révision des normes d'émission de CO2 pour les véhicules particuliers et utilitaires légers neufs dans le cadre du paquet ajustement à l'objectif 55 pour 2030. Le texte adopté exprime le soutien des députés à la proposition de la Commission visant à atteindre une mobilité routière à émission nulle d'ici à 2035. Le 28 juin 2022 sous la présidence française, la 2ème étape était franchie. Les ministres européens de l'environnement ont en effet convenu de relever les objectifs en matière de réduction des émissions de CO2 pour les voitures neuves et les camionnettes neuves d'ici à 2030 à 55% pour les voitures et à 50% pour les camionnettes. Ils ont également approuvé l'introduction d'un objectif de réduction des émissions de CO2 de 100% d'ici à 2035 pour les voitures et camionnettes neuves. Fort heureusement une clause de revoyure a été ajouté pour tenir compte des développements technologiques. Selon Marc morte UE délégué général la plateforme automobile française. Les dépenses de recherche et le développement de la filière en France représente environ 7 milliards d'euros par an à l'occasion des travaux menés par la commission des affaires économiques sur la filière automobile c'est ce celui-ci nous a assuré que les choses sont lancés, il faut réussir, nous n'avons pas le choix, on lui et c'est irréversible. Les inquiétudes sont pourtant nombreuses. Le premier risque identifié touche à notre souveraineté. En France, les véhicules électriques et hybrides rechargeables ont représenté près de 18 pour 110.000 tracts immatriculations 2021 alors qu'elle ne représentait que 3% en 2019. Il y a actuellement 640.000 véhicules électriques en circulation en France alors qu'il en faudrait un peu plus de 15 millions en 2035. Comment s'assurer que ces véhicules seront fabriqués en France ou en Europe qu'ils ne seront pas importer de pays étrangers comme la Chine. Pourra-t-on produire en France les batteries et les bornes de recharge. Par ailleurs, la production de véhicules électriques est dépendante de l'approvisionnement en mais aura tels que le cobalt, le lithium ou le nickel. Or la France et l'Europe ne sont pas producteurs de ces métaux. À l'occasion de la séance de questions au gouvernement du 12 janvier dernier. Monsieur le ministre de l'Économie a évoqué son souhait de rouvrir une usine de lithium. Les Français sont-ils prêts à ouvrir des mines et accueillir ce type d'usine sur leur territoire. A-t-on les compétences pour le faire. Pourrons nous respecter les délais européen aura-t-on le temps d'implanter des entreprises de fabrication de bornes de recharge. Se pose également la question de l'énergie et du bilan carbone de véhicules électriques. Pour calculer la quantité de CO2 produites par une voiture, il faut tenir compte non seulement du CO2 émis pendant son utilisation mais aussi de émissions causées par sa production et ensuite sa destruction. La production et la destruction d'une voiture électrique sont moins respectueuse de l'environnement que la production et la destruction d'une voiture équipée d'un moteur à combustion. La manière de produire de l'électricité est donc crucial. Les atermoiements des précédents gouvernements sur le nucléaire nous ont conduit au risque de coupures d'électricité. Avec le zéro artificialisation nette pour nous mettre en oeuvre les projets de centrales nucléaires annoncé. En 2035, pour nous alimenter les 15 millions de véhicules annoncé avec de l'énergie bas-carbone ou serons-nous obligés d'importer une énergie carbonée produite à l'étranger. La France n'aimait qu'entre 0 9 et 1,5% des émissions mondiales de CO2. Quand la Chine est responsable de 29% les États-Unis de 14%, ce chiffre est en grande partie dû au fait que la France a délocalisé ses émissions de CO2. Il ne faudrait pas que la brièveté du délai imposé nuisent in fine et au bilan carbone des véhicules électriques. Sans compter que nous ne savons pas recycler les batteries de ces véhicules lorsqu'il y en aura 15 millions en circulation sur le territoire français quand ferons-nous. Enfin tous les citoyens entrepreneurs pour ont-ils bénéficier de cette révolution, il y a les barrières du coût d'achat et d'usage le déploiement des bornes de recharge mais aussi de l'évolution technologique, à l'instar des camions présents sur les marchés par exemple de nombreux véhicules utilitaires et professionnelle n'ont aujourd'hui pas leur homologue en électrique. Ces véhicules bénéficieront-ils de dérogation en cas de ZFE. Comme nous l'avons fait en matière d'énergie, ne faut-il pas accepter qu'il y a un mix je pense ici à l'hydrogène, mais aussi aux innovations sur le moteur thermique et il existe des études notamment australienne sur la dépollution du moteur diésel. Faut-il se priver de ces formes d'innovation, l'électrique est-elle la solution universelle. Toutes ces inquiétudes nous invite à ne pas confondre vitesse et précipitation. Cette politique doit être conduite au bénéfice de notre économie et de l'équilibre de notre société et être pensé avec les entreprises pour nos concitoyens. La lutte contre le dérèglement climatique doit être une chance pour l'économie française et non l'occasion de valoriser des économies étrangères. Avec mes collègues du groupe Les Républicains. Nous avons conçu ce débat comme un point d'alerte. Alerte à ne pas reproduire les atermoiements erreurs commises en matière du nucléaire. À l'air ça ne pas adopter des mesures qui enfermerait notre économie et exclurait toute forme d'innovation alerte enfin à veiller à la cohésion de la société sans marginalisés. Une partie de nos concitoyens. Le tout électrique soulève de nombreux enjeux en matière d'infrastructures de souveraineté industrielle et de lutte contre les inégalités socio- économiques le présent débat doit être l'occasion de réfléchir ensemble à une stratégie quelconque volontaire collègue je vous remercie. Ah bah c'est parfait, merci beaucoup. Merci la parole est à madame Olivier. Voir Ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme pour une durée de 8 minutes maximum. Madame la présidente, monsieur le président babary, mesdames, messieurs les sénateurs. La voiture de demain sera électrique, les voitures électriques continuent de se faire une place de plus en plus conséquente. Dans les ventes de voitures neuves de l'Union européenne. 1,1 million de véhicules électriques qui ont été vendus en 2022. Ces 28% de plus en une année. Elles représentent au total 12,1% des voitures neuves vendues en 2022 contre 9,1% en 2021. Ou encore 1,9% en 2019. Selon les chiffre publiés par l'Association des constructeurs, constructeurs européens en France, c'est même un taux supérieur avec 13,3% des véhicules vendus qui était entièrement électrique en 2022, soit 200.000 sur les 1,5 millions de véhicules vendus. Derrière ces chiffres. Je souhaite profiter de ce débat pour porter 3 messages clés sur le développement du véhicule électrique en France. La voiture électrique est indispensable. Essentiel pour décarboner notre secteur des transports. Dans son dernier rapport, le GIEC alerte sur l'urgence climatique. Il reste quelques années vous le savez pour agir. Éviter les pires conséquences d'un changement climatique non maîtrisée pour les générations futures les années qui sont devant nous sont décisives pour déployer des solutions qui nous permettent de contenir ce réchauffement en deçà des 2 degrés Celsius, le véhicule électrique en tant que solution d'ores et déjà disponible et mature fait partie des leviers absolument indispensable et d'ailleurs, d'après le GIEC je cite les véhicules électriques alimentés par de l'électricité à faible émission offrent le plus grand potentiel de décarbonation pour le transport terrestre. Les émissions du secteur des transports qui pèsent pour 25%. Des émissions en Europe et pour 30% des émissions en France ne baisse pas et même au contraire continuent d'augmenter, plus 12% entre 1990 et 2015 en cause, la dépendance aux carburants fossiles. Le maintien d'un niveau élevé d'émissions par véhicule, mais aussi la croissance des trafics. La fin des voitures thermiques et la conversion à l'électrique sont donc des leviers absolument essentiel. Une étape dans le chemin vers une mobilité décarboné. L'interdiction de la commercialisation des véhicules thermiques à compter de 2035 en Europe a le mérite de la clarté. Une voiture électrique acheté en 2022 et conduite en France émet 5 fois moins de CO2 que son homologue à essence grâce à une électricité produite essentiellement à partir d'énergie nucléaire mais aussi renouvelable source d'énergie bas-carbone. Ailleurs en Europe. C'est également en moyenne 3 fois moins. D'ici 2030 l'empreinte carbone des véhicules électriques est amené à se réduire encore grâce à une électricité de plus en plus produite à partir d'énergies bas carbone mais aussi de l'amélioration de la performance environnementale des batteries. Le gouvernement travaille à bâtir une filière industrielle complète pour les véhicules électriques cette décarbonation vous l'avez mentionné monsieur le sénateur Babary ne doit pas se faire au détriment de l'industrie française, c'est une évidence, il faut que la France prenne sa part dans le renouvellement du parc automobile français. On ne peut pas importer massivement des véhicules électriques fabriquées dans d'autres pays. Le président de la République l'a rappelée encore lors du Mondial de l'automobile d'octobre dernier. Nous avons une stratégie pour faire de la France une grande nation de véhicules électriques, et pour maintenir une industrie automobile forte souveraine en France, produire 2 millions de véhicules électriques par an en France en 2030 ainsi que les composantes stratégiques de leur chaîne de valeur batteries électroniques mais aussi le logiciel bornes de recharge. Je parle ici de l'ensemble de la chaîne de valeur. Nous devons réussir à maîtriser les technologies de pointe qui vont des moteurs électriques jusqu'aux batteries en passant par les composantes électroniques de puissance et les systèmes qui vont servir aux véhicules automatisés. Par ailleurs, le maintien de la localisation sur le territoire national. Les usines d'assemblage de véhicules est absolument primordial pour notre filière automobile d'excellence et pour tout ce qui contribue, et lors du Mondial de l'automobile les constructeurs Renault et Stellantis ont ainsi annoncé l'affectation de 15 nouvelles modèles de véhicules électriques dans leurs usines françaises. L'État mais des moyens sans précédent pour atteindre cet objectif d'une production annuelle de 2 millions de véhicules électriques à horizon 2030. Nous mobilisons via le programme France 2030 pas moins de 5 milliards d'euros pour l'ensemble de la filière automobile à la fois pour soutenir bien sûr la recherche et le développement, mais aussi pour l'industrialisation des véhicules et de leurs composants en France 3ème, élément clé. Le gouvernement reste très vigilant sur les impacts industriels et sociaux de l'arrêt de commercialisation des véhicules thermiques en 2035 l'arrêt de la commercialisation des véhicules thermiques dès 2035 est un tournant majeur pour la filière automobile la décarbonation du parc automobile va dans le sens de l'histoire et nous sommes prêts évidemment à soutenir tous les acteurs dans cette mutation industrielle. Il est indispensable d'accompagner nos entreprises mais aussi les salariés, de les former dans cette révolution pour en faire pour faire en sorte, pardonnez-moi, que la France garde une industrie automobile performante et souveraine. Plusieurs activités liées au thermique vont naturellement décroître avec des impacts. Dans certaines filières de sous-traitance. Certains impacts majeurs le décolletage la fonderie fonte la forge. Sont par exemple des activités qui vont faire face à des baisses de commandes dans les prochaines années. L'État accompagne ces entreprises dans leur projet diversification soit vers le véhicule électrique soit en dehors de la filière automobile parce qu'il y a là aussi des reconversions possibles. Outre les entreprises sont aussi nos territoires qu'il faut accompagner dans l'évolution du tissu industriel et c'est bien pourquoi l'État a mis en place en lien, évidemment avec la banque des territoires. Un appel à manifestation d'intérêt dénommé rebond industriel dans le cadre du programme que vous connaissez bien territoires d'industrie une enveloppe de 100 millions d'euros et déjà dédié à aider les territoires impactés par les mutations du secteur automobile pour identifier des projets industriels dans les bassins d'emplois affectés mais aussi garantir à chaque salarié de l'industrie automobile des perspectives d'emploi dans son bassin de vie mais aussi dans des secteurs d'avenir. Vous le voyez donc, mesdames, messieurs les sénateurs. L'État est conscient de la révolution que nous avons à mettre en oeuvre ensemble et met tout en oeuvre pour accompagner la filière automobile dans cette décarbonation absolument stratégique bien sûr. L'objectif est ambitieux mais il n'est plus le temps de tergiverser, les décisions d'investissement des entreprises se prennent aujourd'hui et elles doivent être orientés clairement en faveur de l'électrification de notre parc automobile nous aurons loisir d'en parler lors de ce débat auquel je répondrai avec la plus grande acuité possible je vous remercie. Merci madame la ministre. Dans la suite du débat. Chaque orateur dispose de deux minutes maximum, y compris l'éventuelle réplique. Le gouvernement dispose pour répondre à une durée équivalente. Le gouvernement aura la faculté s'il le juge nécessaire de répondre à une réplique pendant une minute et l'auteur de la question disposera leur à son tour du droit de répondre pendant une minute. Et la première question est à monsieur Daniel Salmon. Merci madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. L'Union européenne a fait de la motorisation électrique. Un axe central de son paquet mobilité la fin de la vente de véhicules thermiques 9 et pour 2035 et 15 ans après en 2050 les émissions du parc effectif de véhicules devront être au régime de la neutralité carbone. Les batteries bien entendu sont une priorité de relance et de mutations de l'industrie automobile. Le marché de l'électrique d'école. Reste qu'au rythme actuel de leur renouvellement si l'équipement voiture restaient similaire à celui d'aujourd'hui nous ne parvient Drillon pas en 2050 à la neutralité. De plus, la seule conversion à l'électrique ne répond pas à tous les enjeux. En particulier la réduction de la pollution par les particules fines, liées à la précision des chaussées à l'usure des pneumatiques. Les enjeux de réduction de l'empreinte des matériaux employés pendant la pour la construction qui constituent 75% du bilan, leur durée de vie, leur recyclage leur empreinte sociale aussi. Dans les mines lointaines aux conditions indignes d'des enjeux sur la nécessaire mutualisation des automobiles pour accroître leur temps réel d'usage et diminuer leur nombre le nécessaire report modal vers les transports collectifs pour agir sur la congestion vers les mobilités actives aussi pour qu'elles donnent tout leur potentiel. Le gouvernement a-t-il donc au-delà de la mutation électrique des moteurs, la volonté de conduire en même temps la mutation des usages en se donnant les moyens de réduire la place de l'automobile et de de l'auto-solistes dans nos mobilités et puis ce que nos constructeurs sans faire en misant essentiellement sur et SQV laissant de fait l'espace à la con fulgurances étrangères pour les véhicules électriques légers qui s'imposeront. Demain, le gouvernement a-t-il la volonté de contrecarrer cette dérive qui minent l'avenir de notre compétitivité industrielle et de nos emplois. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur Salmon vous aborder plusieurs sujets au sein de cette même question d'abord. Rappeler que contrairement à d'autres secteurs. Je le disais en en discussion générale effectivement les émissions du secteur des transports continue d'augmenter. En cause, la dépendance aux carburants fossiles le maintien d'un niveau élevé d'émissions par véhicule et la croissance des trafics. C'est donc cette conversion à l'électrique est un levier essentiel et c'est bien l'objet de notre débat aujourd'hui des véhicules thermiques en Europe en 2035, il en restera et vous l'avez mentionné encore énormément en circulation. On estime d'ailleurs que la moitié du parc automobile français, soit 20 millions de véhicules sera encore carbonée. En 2035, il nous faut donc accélérer la. Pardon la décarbonation du secteur des transports par exemple et je pense qu'on en reparlera en misant beaucoup voire plus sur le rétrofit. C'est-à-dire notre capacité à remplacer un moteur thermique, par une propulsion à moindres émissions par exemple avec un moteur électrique ou à moteur à pile combustible à hydrogène. Cette opération reste encore cher, pas assez massifier nous sommes en train de travailler en ce moment même, notamment avec le ministre des Transports Clément Beaune à la à la démocratisation du rétro feed pour faciliter la conversion du parc automobile dans les prochaines années pour les 20 millions de véhicules qui resterait encore carbonée en 2035. Je précise d'ailleurs mais vous avez dû le voir que l'État a lancé entre novembre 2022 et janvier 2023 une consultation au sujet du rétro chiite pour récolter les propositions des industriels du rétro rétrofit de véhicules particuliers. Nous sommes en train, du moins le ministre de l'industrie, mais aussi le Ministre des transports sont en train d'étudier toutes ces propositions et vont bientôt communiquer sur un plan d'action courant mars ça devrait permettre ensuite à des particuliers comme nous le souhaitons de convertir à un coût moins élevé et de façon plus facile dans des garages sur nos territoires anneau particulier de pouvoir convertir leurs véhicules thermiques en véhicules électriques. Pour la 2ème, partie de la réponse, je suggère de vous faire une réponse écrite. Je vous remercie. Merci madame la ministre, on va respecter vraiment le temps parce que nous avons notre débat ensuite. Monsieur Salamon, vous avez 19 secondes. Merci madame la présidente. Effectivement, Madame la Ministre vous avez insisté sur les profil qui est fort intéressant parce qu'il permet de ne pas gaspiller l'énergie grise qui est contenu dans une voiture, c'est forcément un élément essentiel. Par contre, on ne pourra pas faire l'économie de la sobriété d'usage et de la sobriété de dimensionnement ainsi qu'un d'aménagement du territoire qui permette de revoir nos mobilités. Merci. Madame la Ministre. Le travail est en cours et Clément Beaune, le ministre des Transports a annoncé un plan à votre disposition si vous souhaitez qu'on en parle ensemble, en tout cas le plan est lancée et nous l'avons dans le viseur. Je vous remercie. Eh bien je, je me réjouis et je suis tout à fait. Enclin à participer et à échanger avec vous sur ce sujet du covoiturage puisque. Des comptages qui sont faits à l'entrée de Rennes métropole par exemple indique que sur 100 véhicules aux heures de pointe le matin il y a 102 personnes de transportées c'est-à-dire 98 véhicules avec une seule personne à bord, 2 covoituré pas tous les jours, mais simplement une fois dans la semaine, on n'aurait plus aucun embouteillage aux portes de la ville. Donc voilà il y a des solutions. Il va falloir faire en sorte que ce qui fonctionne bien sur le long, le long trajet avec Blablacar, pour le citer arrive à fonctionner au quotidien avec des lignes de covoiturage. Il y a des expériences qui sont en cours également. Sur cette métropole et j'espère que ça va se développer au niveau national parce que c'est une vraie solution pour limiter les embouteillages parce que la voiture électrique elle est comme les autres voitures elles provoquent des embouteillages et des problèmes de stationnement. Merci. Merci la parole est à monsieur Frédéric Marchand. et du savoir-faire reconnu des ouvriers cette ambition c'est notamment celle de Renault. Pionnier du véhicule électrique qui investit massivement dans cette solution. Confère le modèle vedette Zoé et 32.000 exemplaires l'an dernier, la marque française, se positionne également numéro un sur le créneau des utilitaires électriques avec la Kangoo produite à Maubeuge, dans le département du Nord. Corollaire indispensable du véhicule électrique, la batterie. La région Hauts-de-France n'est pas en reste dans ce domaine en particulier dans le département du Nord devenu The play-list oublié de la batterie électrique en quelques années en effet après le pôle Electricity de Renault et l'implantation du groupe chinois Envision et celle de Stellantis et de TotalEnergies à Douvrin Dunkerque accueillera la 3ème giga-usine française de production de batteries électriques avec l'implantation de Vercors qui permettra de faire des Hauts-de-France, la vallée de la batterie segments plus qu'indispensable pour produire sur notre sol les voitures électriques de demain. On ne peut que se réjouir de ce renouveau et la réindustrialisation des Hauts-de-France. Ces trois giga-factories. Ce sont, à terme, 7500 emplois Directs et 15.000 indirects qui vont être créés dans notre région, c'est un pari ambitieux qui passe par la mise en place d'un véritable écosystème notamment dans le domaine de la formation en amont des futurs salariés de ses usines. Celle-ci doit être anticipé pour pouvoir alimenter en personnel qualifié ces entreprises et notamment en favorisant la formation des personnels, locaux, dont le savoir-faire anciens n'est plus à démontrer. À cet égard les difficultés rencontrées par la filière nucléaire pour trouver du personnel à même de concrétiser ses ambitions et ses projets doivent nous servir de référence et de garde-. La perspective de ces employes est une véritable bouffée d'air pour ce territoire longtemps meurtri mais passe par un énorme défi dans le domaine de la formation, la réussite du tout électrique dans notre pays passe par une mobilisation qui doit embarquer tous les acteurs de la formation et notamment l'éducation nationale. Alors Madame la Ministre quelles sont les orientations retenues par le gouvernement pour réussir ce défi de la formation garant essentiel de la réussite du tout électrique. Merci madame la ministre. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, marchant, vous l'avez mentionné avec clarté. Oui le nord. Est au coeur du déploiement de l'écosystème. En faveur des de de l'automobile électrique, le constructeur Renault. S'engage fortement dans l'électrification de sa gamme avec notamment la constitution du pôle Electricity dans le nord de la France autour des villes de Douai de Maubeuge, de Ruitz avec un objectif d'un million de véhicules produits par an en 2031. En parallèle, 3 entreprises ont des projets de construction de méga-usines de batteries de véhicules électriques dans les Hauts-de-France a cessé à Douvrin Vercors à Dunkerque et and Vision à Douai. Ces usines devraient créer. Au moins 6500 emplois Directs à l'horizon 2030 vous mentionnez monsieur le sénateur, 7500 emplois, c'est à peu près l'étiage que nous avons et comme vous nous nous réjouissons des perspectives de constitution en France d'une filière complète des véhicules de demain mais aussi et surtout de la création d'emplois que cela va susciter vous avez et je vous en remercie la question fort légitimes de la formation. Il nous faut apporter une réponse rapide et formé à ces métiers dont certains sont quand même non pas des métiers de l'automobile classique mais les métiers de l'automobile de demain. Vous le savez à travers. France 2030 nous mobilisons pas mal de moyens et je vous rappelle que 2 5 milliards d'euros sont mobilisés sur la formation et les compétences rien qui va à travers pardonnez-moi. France 2030. Je ne parle même pas des efforts réalisés pendant le précédent quinquennat à titre d'exemple, ça va permettre et ça a permis surtout à l'état de soutenir le projet Que vous connaissez à hauteur de 14 millions d'euros, ce projet lauréat de l'appel à manifestation France 2030 accélère la structuration de nouvelles formations autour de technologies automobiles d'avenir. L'école de la batterie porté par Vercors à Grenoble a reçu 14 millions d'aide dans le cas de cet appel à manifestation d'intérêt. 2 autres projets sont également lauréat dans les Hauts-de-France pour répondre aux besoins à court terme en matière de formation d'Envy Vision, nous travaillons aussi et je vais vite au niveau des comités stratégiques de filière du Conseil national de l'industrie pour aussi identifié plus les compétences dont nous aurons besoin. Je ne serai pas plus longue, la présidente m'en voudrais je vous remercie. Merci, merci, la parole est à madame Martine Filleul. Si madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues, le les hasards de la vie font que ma question est assez proche de celle de Monsieur Marchand. Vous allez donc pouvoir approfondir votre, votre réponse, madame la Ministre décarboné au plus vite le parc automobile afin de respecter nos engagements environnementaux est un impératif. Reste à savoir comment nous allons atteindre cet objectif en aucun cas nous ne pouvons mettre sous le tapis. Les implications sociales et économiques pour les personnes les plus vulnérables concernés par cette mieux incontournable, je pense évidemment à nos compatriotes aux fins de mois difficiles, pour qui l'achat d'un nouveau véhicule électrique est hors de portée. Malgré les aides déjà mises en place mais je pense aussi comme sénatrice du Nord à mon territoire qui vous le savez a particulièrement souffert d'une désindustrialisation massive depuis la fin des 30 Glorieuses constructeurs ou équipementiers. Ce ne sont pas moins de 50.000 employés qui travaillent aujourd'hui dans le secteur automobile. Le président de la République a prévu la production de 2 millions de véhicules électriques et hybrides en France l'horizon 2030 et 3 projets de gigafactories à Douai, Dunkerque et Maubeuge ont été annoncés, mais un chiffre m'interpelle en raison d'un nombre de pièces inférieure là où il fallait 5 ouvriers pour produire un véhicule seuls trois suffisent désormais pour un véhicule électrique vous évoquez seulement 7006 1500 emplois nous assurer qu'au 1er janvier 2035, à la fois que la filière automobile française sera prête et que nos territoires industrialisés ne seront pas une nouvelle fois sinistrée. Que prévoit l'État pour prévenir la disparition de certains postes dans l'industrie automobile et assurer la conversion des salariés et avec quelles dispositions. Merci. Madame la Ministre. Merci madame la présidente, je réponds à la vie à l'invitation de la sénatrice filleul et si vous m'autorisez, je vais poursuivre ce que je n'ai pas pu dire juste avant. Au-delà de tous les projets que le Territoire du Nord a réussi à, à remporter puisque quand même rendons. Hommage au territoire c'est le territoire qui gagne. Et qui est lauréat de ses nombreux appels à manifestation d'intérêt je je voulais aussi ajouter que nous sommes en train de travailler j'allais trop vite au niveau des comités stratégiques de filière au Conseil national de l'industrie pour identifier justement les compétences dont nous allons avoir besoin dans le cadre de ses nouvelles productions et donc de ces nouveaux métiers, je veux aussi ajouter un mot sur le fait que Bruno Lemaire vous le savez présentera d'ici quelques mois un projet de loi très important de réindustrialisation verte. Je tiens à vous dire qu'il abordera très clairement avec un axe entiers du projet de loi, madame la sénatrice. La question majeure de la formation des compétences et des talents. On a donc missionné de pilotes pour le chantier spécifique de la formation au sein du projet de loi réindustrialisation verte, madame la députée, Astrid Panosyan-Bouvet que vous connaissez sûrement et monsieur Moussa Camara président fondateur des déterminée, ils travaillent ensemble depuis quelques semaines et sont si vous souhaitez échanger et on peut organiser la mise en relation en organisant justement des échanges précis pour faire remonter des propositions concrètes en matière de formation et notamment pour les personnes les plus éloignées ou les plus fragiles en matière d'employabilité, celle que vous mentionnez, madame la sénatrice, ses propositions que vont porter ces 2 personnalités ont vocation justement à venir nourrir le véhicule législatif qui arrivera dans quelques mois sur le sujet de la formation professionnelle de l'enseignement aussi professionnel aussi professionnel mais aussi supérieur et c'est l'ensemble du gouvernement au-delà de Bruno Lemaire mais avec aussi le ministre de l'éducation, le ministre du Travail qui va s'atteler à au sein d'un axe entiers du projet de réindustrialisation verte a essayé de, de renforcer au maximum l'employabilité. et la qualité des formations en faveur de de l'industrie de l'automobile électrique, c'est une invitation là aussi peut-être à ce que vous voulez nourriciers. En tout cas on en a besoin. Je vous remercie madame la sénatrice. Merci la parole est à monsieur le président, Pierre Laurent. Merci madame la présidente, madame la Ministre, l'objectif. 2035 a été entériné son véritable étude d'impact et sans planification globale sur le mode décidons l'un dans l'intendance suivra. Dès lors nous avançons sans stratégie claire on laissant la main aux industriels pour définir nos objectifs de production et en courant le risque de ne soit de ne pas réussir, soit de le faire dans les pires conditions avec inégalités manque de souveraineté à la clé. Parmi les problèmes mal maîtrisé. Je souhaite vous interroger sur les perspectives d'approvisionnement en matières premières critiques composant les batteries au titre desquels figure la volonté déclarée du retour des mines en Europe et la constitution de stocks stratégiques, le principal projet de lithium européen a Jada en Serbie. Donc devait exploiter le tristement célèbre Rio Tinto a été pour l'heure abandonnés par ce pays pour des raisons écologiques. Quant à l'Union européenne, elle s'apprête à assouplir dans l'urgence les règles environnementales pour faciliter l'implantation des mines. Je souhaite donc vous poser plusieurs questions à ce propos disposeront nous et quand, d'une véritable étude d'impact sur les besoins en matériaux critiques pour satisfaire la demande européenne en véhicules électriques. Comptez-vous renforcer le soutien public dans le cadre du plan France 2030, dont 132 millions d'euros ont été décaissés en un an dans le volet matières premières en garantissant que cet argent serve en France à des projets d'exploration et de raffinage conforme à nos ambitions industrielles et écologique. Enfin, quelles nouvelles règles. De commerce international, la France entend-elle promouvoir contre logiques de rentabilité prédatrice de quelques grands groupes mondiaux qui domine aujourd'hui pour garantir et sécuriser l'approvisionnement des matières premières critiques nécessaires au transition écologique. Dans ce cadre, êtes-vous prête avec le gouvernement à agir pour sortir d'une logique de souveraineté égoïste fondée sur la guerre concurrentielle entre États et entre filières

Merci madame la présidente. Monsieur le sénateur, Laurent. Sur la filière automobile en France vous et sur le L'objectif européen que nous nous sommes fixés votre jugement et le vôtre mais il est dur. Je ne crois pas que nous puissions dire que nous n'avons aucune stratégie claire en la matière bien sûr le la bascule est majeur, elle peut être anxiogène, mais. Je pense que nous avons une stratégie et d'ailleurs il est prévu des points d'étape avant 2035 vous le savez la stratégie, elle est assez claire pour donner de la visibilité aux industriels et aux consommateurs. Je vous l'ai dit produire 2 millions de véhicules électriques par an en 2030. Une mobilisation massive des moyens de l'État. Pas moins de 5 milliards d'euros dans le cas du plan France 2030 et ce hors du sujet compétences, formation dont nous venons de parler, qui sera lui-même abondé par ailleurs et le soutien est massif du côté de l'État pour justement accompagner cette mutation vous me questionnez. J'ai à coeur d'y répondre sur le sujet majeur des. Des matériaux critiques. Je veux. Rappeler que d'abord il est possible de recycler les métaux des batteries et je pense que vous le savez, jusqu'à 99%. Que ce soit le lithium, le nickel ou encore le cobalt. Et en plus ça conduirait si on parvenait à les recycler plus par construction à en extraire moins du sol, ce qui serait moins délétères pour notre planète. Des projets d'ailleurs émerge beaucoup en France pour bâtir Cécile de recyclage des batteries de véhicules électriques. Nous disposons par ailleurs en France de gisements de matériaux constitutifs des batteries, le groupe par par exemple le groupe il mérite ce qui a annoncé en octobre 2022, lancement d'un important projet d'exploitation de lithium dans l'Allier qui représentent une capacité d'équipements de 700.000 véhicules en batterie Lithium, Ion par an. J'ajoute qu'il y a à peu près un mois, un délégué interministériel aux métaux critiques, a été nommé. Benjamin Galles Qui est à votre disposition et à la diffusion de l'ensemble des parlementaires pour aborder le sujet que vous avez pointé sur les matériaux critiques, je vous remercie. Merci la parole est à monsieur Patrick Chauvet. Merci madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Le 20 octobre dernier durant la séance de questions d'actualité j'RT, le ministre délégué chargé des Transports au sujet des dangers d'une interdiction pure et dure des véhicules thermiques à partir de 2035. Je ne suis pas certain qu'elle soit souhaitable au regard des investissements colossaux consentis par nos constructeurs pour améliorer les performances écologiques des moteurs thermiques. De plus, la montée en charge du véhicule électrique interroge également quant à la pérennité de notre souveraineté industrielle. En effet, nous sommes aujourd'hui dépendant de certaines filières d'approvisionnement, notamment concernant l'importation de Terres rares. Ces précieux métaux décisif pour le fonctionnement des batteries en cas de conflit géopolitique d'ampleur nous serions ainsi vulnérable. Quant à notre capacité à continuer de faire fonctionner notre filière automobile en dépit de cela, il est impératif que nous soyons compétitifs sur le Merchet du véhicule électrique à l'horizon 2035. Mes chers collègues, nous sommes tous conscients, je crois que la concurrence internationale ne nous fera aucun cadeau. La Chine a ainsi fait très tôt le pari de l'électrique contrôlant 56% de la production mondiale des batteries. Pékin s'est doté d'une industrie de l'automobile électrique ultra-compétitive ou les véhicules chinois coûte jusqu'à 30% moins chers que ceux de leurs concurrents européens. De leur côté, les États-Unis soutiennent massivement leurs constructeurs et leur industrie verte avec 370 milliards de dollars avec nos partenaires européens et nos constructeurs automobiles. Nous devons donc dessiné les contours d'un nouveau pacte industriel pour relever le défi du véhicule électrique. À ce titre je salue les annonces de la présidence terre Leyen en date du 17 et du 31 janvier dernier, de la mise en place d'un plan industriel européen pour la compétitivité de nos, de nos industries vertes. Pourtant les récentes prises de position de certains dirigeants des États semble mettre en péril cette initiative je terminerai juste par ma question. la règle elle est comme ça pour tout le monde à partir du moment où je commence à donner 10 secondes à quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir le nombre de messages que j'ai, donc je suis désolé, la règle elle est comme ça, il faut voir par groupe politique hein mais ça a été décidé avec vos président. Donc on ne va pas changer la règle aujourd'hui Madame la Ministre et vous qui avez la parole. Merci madame la présidente, exercice périlleux. Je vais essayer de répondre à une question que j'imagine et je vous demande. De la bienveillance, il se peut que je réponde à côté mais je veux quand même vous dire un mot sur le fait que évidemment c'est un. Un mouvement majeur. Mais je pense que nous en sommes parfaits, enfin je pense. Le gouvernement pense que nous en sommes capables et et l'Europe se met en position, et je voulais peut-être faire un, un focus sur ce que nous faisons en France justement. Et les efforts considérables que nous mettons en place pour aussi accompagner bien sûr les acteurs mais aussi tous les sous-traitants qui sont au coeur de la filière puisqu'on se les dit et le président Babary a dit dans sa discussion générale. L'enjeu n'est pas que la question des batteries électriques, l'enjeu est bien plus largement. La question de la chaîne de valeur. D'abord rappeler que. Comme dans, dans chaque mutation du. Ariel majeur bien sûr certaines certains savoir-faire et certains emplois disparaîtront. Mais il y a aussi de nombreuses innovations et de nombreuses opportunités industrielles qui sont en train de se créer dans notre pays. Qui sont autant de secteurs de croissance et création d'emplois. Ensuite dire que les sous-traitants de la filière automobile traditionnels sont en train de se diversifier. Bien sûr l'empreinte carbone des véhicules thermiques que vous mentionnez. Monsieur le député diminue pardon excusez-moi, autant pour moi. Voilà la je perds du temps. Non non non les sous-traitants la filière automobile se diversifie, soit vers des segments de la filière non exposés aux motorisations thermiques, soit vers de nouveaux secteurs, je le disais hors automobile pour accompagner ces changements, l'État accompagne les sous-traitants directement en leur dédiant pas moins de un 5ème des 5 milliards du soutien de la filière automobile, c'est un milliard d'euros pour nos sous-traitants qui va permet de soutenir leur croissance qui va permettre de faciliter la transition des sous-traitants historique d'accompagner aussi la reconversion des salariés des sites et des territoires impactés et vous dire aussi que Bercy a mandatée aussi le Conseil général de l'économie mais aussi l'Inspection générale des finances pour évaluer les conséquences sur le tissu industriel français de l'arrêt du moteur thermique et proposer aussi des actions très spécifiques, les résultats sont attendus à la fin du 1er semestre 2023. Je vous remercie. Merci la parole est à monsieur Jean-Pierre Corbisez. Madame la présidente madame miss mes chers collègues si la vente de voitures électriques a connu un bond sans précédent pour atteindre 12% en 2022. Notre pays accuse un retard sérieux sur nos homologues européens notamment nordiques avec par exemple un taux de 9 véhicules Avec un Pack de voitures circulent en Europe de près de 300 millions de véhicules. Je vous épargne le calcul, il nous faudra beaucoup de temps, énormément de temps pour aboutir à une conversion à au tout électrique. De surcroît le développement intensif de la voiture électrique pose de nombreuses questions économiques en 1er lieu le véhicule électrique coûte cher à hauteur de 20.000 euros pour les premiers prix, là où le thermique coûte parfois moitié prix tous les automobilistes ne peuvent se le permettre, sans compter les inquiétudes légitimes des consommateurs sur le niveau du prix de l'électricité dans les années à venir. Industriels, ensuite la crise de la Covid 19, a mis en péril les circuits d'acheminement des matériaux nécessaires à la fabrication des batteries. Des gisements ont été découverts en Europe mais il faudra des années avant de pouvoir en tirer les fruits. Quant au déploiement des bandes de chargement sera-t-il en mesure de suivre le rythme de la progression attendue des voitures électriques et leur peu probable que l'objectif de tout électrique en 2035 atteignable. D'autant que les fabricants autorisés déjà atteint leur 1er objectif de réduction de gaz à effet de serre et serait peut-être tenté de mettre la pédale douce sans mauvais jeu de mots sur la production électrique pour écouler leurs stocks de véhicules thermiques. Partant de là, n'est-il pas au portable le Ministre de miser aussi sur l'hybride en relançant par exemple le dispositif fiscal qui a été supprimée et qu'en est-il de l'hydrogène, ne faut-il pas par ailleurs accompagner la transition énergétique et la conversion de notre parc actuel de véhicules thermiques afin qu'ils soient moins émetteurs de gaz à effet de serre. Enfin, pouvez-vous rassurer l'inquiétude légitime de nos industriels de l'automobile au regard du plan d'aide américain massif qui risque de le fragiliser et bien à présent je vous offrent mes 15 secondes. Quelle générosité. Oserais-je dire au sénateur Corbizet qui en plus en moins de deux minutes. Me pose pas moins de 6 questions quel challenge donc je vais. Obligatoirement, Monsieur le Sénateur, être obligés de concentrer un peu ma réponse et je m'en excuse, ça n'empêche pas des réponses par ailleurs aux autres points que vous abordez un aide à l'acquisition de véhicules électriques. Évidemment, vous l'avez dit, elles sont encore plus cher parfois même bien plus cher que les véhicules thermiques rappeler quand même que plus d'un milliard d'euros de crédits budgétaires ont été consommés au titre du bonus écologique en 2022. Plus de 325.000 dossiers traités depuis le 1er janvier 2023, comme vous le savez, monsieur le sénateur, le bonus écologique. Voit son montant maximal diminué de 6000 à 5000 euros pour les particuliers mais il pourra être majoré de 2000 euros. Comme vous l'arrêt ça avait pour près de la moitié des ménages rappeler aussi que le leasing social à 100 euros par mois sera aussi proposé courant 2024, comme nous nous y étions engagés aux ménages les plus modestes. Rappeler enfin que s'agissant de la prime à la conversion. Elle exclut les ménages les plus aisés, elle peut aller elle aussi jusqu'à 6000 euros en fonction des revenus de l'acquéreur. c'est important de le mentionner le rétro feat. On ne le sait pas assez est éligible à une aide allant jusqu'à 6000 euros en 2022, les constructeurs français sont concernés par près de 50% des bonus octroyés. Nous devons néanmoins réfléchir à des critères. Je ne doute pas que vous serez force de proposition au Sénat, dans le cas du projet de loi réindustrialisation verte qui sera le vecteur de cette évolution. Je voudrais aussi quand même rapidement vous répondre sur les bornes au 31 décembre 2022, la France dispose de plus de 82.000 points de recharge, plus 53% sur les 12 derniers mois. L'objectif des 100.000 bornes. Devrait être atteinte à train atteint bien sûr, on a pris un peu de retard. Je ne le nie pas. Le contexte a été aussi difficile ça nous place quand même la France au 3ème rang des pays les mieux équipés dans l'Union européenne. Donc certes derrière nos voisins du nord, les Pays-Bas et les Allemands, mais nous ne sommes pas en reste et nous allons continuer à en installer. Je vous remercie. Merci. non mais parce que moi je, je vais vous réexpliquer parce que je pense que les gens ne comprennent pas bien, si vous prenez même ne serait-ce que 5 secondes, vous rendez aussi une minute à Madame la Ministre qui peut passer un peu plus de temps pour vous répondre

Et ça, sur les bornes. Oui mais c'est, vous savez que j'aime le Sénat. Monsieur le sénateur. Juste vous dire que sur les les recharges, plus de 90% des recharges c'est on le sait pas non plus elle s'effectue à domicile. Et 20% des Français vivant résidentiel, collectif disposant d'un Parking et vous dire que dans ce contexte, l'État soutient beaucoup les dispositifs facilitant l'acquisition l'installation de matériaux de recharge dans les logements collectifs. En plus du crédit d'impôt. De la prime à devenir et d'un taux de TVA réduit pour les bornes achetés par les particuliers. Plusieurs outils de financement sont mises à disposition des bailleurs et des particuliers par la banque des territoires, ces outils doivent nous permettent d'atteindre un objectif de 16.000 copropriétés privées accompagné d'ici 2024 pour plus de 125.000 points de recharge. Merci madame la présidente. Merci c'est bon Monsieur Corbizet très bien sinon vous aviez encore une minute hein. La parole est à madame Françoise Dumont. Madame la présidente Madame la Ministre l'Union européenne a donc acté la fin de la vente des véhicules neufs à moteur thermique à compter de 2035. Les ZFE pleurer fleurissent pardon dans les métropoles européennes sur le papier ce changement complet de façon de penser la mobilité pourrait sembler intéressant du point de vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre mais le diable se cache dans les détails. Premièrement comment rajouter le raccordement d'un parc automobile sur notre production vacillante. Pour quel prix de rechargement avec l'augmentation des coûts de l'énergie, sans même parler du retard pris par le déploiement des bornes de rechargement, vous venez de l'évoquer. Enfin les entreprises automobiles françaises et européennes ne sont pas en capacité à ce jour de répondre à l'immense vague de demandes qui va se mettre en place dans toutes les prochaines dans les toutes prochaines années, ce sont donc les entreprises chinoises qui bénéficieront de cette nouvelle manne financière puis en cette période de forte inflation, comment des familles devant changer un voire deux véhicules pourront-elles le faire en effet, même avec des aides ciblées de l'État, le reste à charge pour les particuliers mais aussi pour les artisans sera très conséquent de plus s'agissant d'une technologie assez récente. La question du recours à l'achat d'occasion ne pourra pas forcément être une option pour l'ensemble des acheteurs. Enfin il y a la question de la gestion des incendies de véhicules électriques et qui n'est pas des moindres, qui impose beaucoup de contraintes pour nos services de secours. En effet, lorsqu'un véhicule lorsqu'un feu de véhicule électrique se produit les sapeurs-pompiers doivent refroidir le véhicule brûler voir donc l'immergé dans de l'eau pendant des dizaines d'heures d'affilée pour éliminer le risque d'un nouveau départ de feu depuis une batterie en surchauffe. Or nos SDIS ne sont pas tous équipés pour répondre à un risque, il ne fait que s'accroître avec l'électrification du parc roulant aussi Madame la ministre au regard de tous ces points, comment le gouvernement envisage-t-il d'accompagner cette révolution de la mobilité sans abandonner les particuliers, les artisans, voire même un grand. Entrepreneur français et. Merci, madame la Ministre. Nous ne disons pas que ce sera facile, nous disons que là où il y a une volonté, il y a un chemin on peut regarder toutes les complications. Il y en a beaucoup. Mais je peux pas laisser dire. Sur les recharges par exemple. Bien sûr on a pris un peu de retard hein. Je ne nie pas le fait que ça devait être ces chiffres en fin d'année 2022, il s'est passé pas mal de choses vous le savez comme moi, mais les chiffres sont quand même assez encourageant, plus 53% en 12 mois la France 3ème pays dans l'Union européenne en matière d'installations de recharge. Pour les véhicules électriques. Voilà je vous passerai le pessimisme d'humeur et l'optimisme de volonté mais je pense qu'il faut qu'on y croit et même s'il y a pas mal de difficultés, les ZFE en font partie. Je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal et les chiffres en matière d'installation. De bornes le démontre sur les ZFE. Je veux rappeler 2 choses, d'abord le gouvernement a mis en place des aides substantielles, vous le savez pour aider les. Professionnels à remplacer leurs véhicules thermiques par un véhicule électrique aide quand je dis substantielle qui peut aller jusqu'à 13.000 euros de subventions pour l'achat de véhicules utilitaires électriques selon leur masse en incluant la prime à la conversion, c'est important, notamment pour les artisans et les indépendants. Sur lesquelles je suis évidemment particulièrement vigilante. Ensuite même si l'objectif est clair, je comprends très bien mais alors très bien qu'il puisse soulever certaines aux interrogations voire plus. Il est important que ces ZFE soit mise en place de manière concertée concertée avec toutes les parties prenantes. C'est le cas dans un certain nombre de métropoles. Je ne saurais qu'appeler la concertation dans toute et notamment dans celles dont j'ai l'honneur d'être élu. Le gouvernement a ainsi mis en place un point d'entrée unique. Par ailleurs, avec la nomination d'un coordinateur interministériel aux ZFE monsieur Qui est à la disposition des parlementaires qui souhaiteraient le soumettre. Le soumettre ou pas du tout le rencontrer mais Paul soumettre du tout vous enfin ou pourquoi pas enfin ça c'est à vous de voir madame la sénatrice. Non. En revanche, blague à part vous mentionnez en tant que sénatrice du Var, le point important des incendies sur lequel, je vous le dis, je n'ai pas de réponse. Je comprends votre sensibilité et donc je suggère qu'on y réponde. Je n'ai pas la réponse à cette heure mais on vous doit une réponse. Merci, merci, la parole est à monsieur Pierre Jean Verzeletti. Madame la présidente, madame la Ministre. Je vais vous permettent de reparler des des des bornes électriques. Sur le débat qui nous est posée. Vous avez donné les chiffres, aujourd'hui il y a 80.000 bornes qui sont installés. Retard qui a été pris et à la fin de la décennie, on devrait en théorie atteindre quasiment 500.000 bornes de poser. Sachant qu'on se bat sur un calcul qui fait qu'il faudrait une borne électrique à peu près pour 10 véhicules. Il y a les nouvelles qui vont être installées il y a celle qu'il faudra changer puisque la technique, la technologie évolue pour permet de recharger les véhicules plus vite. Alors il y a le sujet du nombre et après il y a le sujet du lieu où est-ce que nous allons mettre ces bornes et pour un certain nombre de villes et de centre-, bourg. Ça va être une révolution en termes d'organisation de de la commune. Vous disiez tout à l'heure 80% des recharges se font à domicile. C'est ce qu'on observe aujourd'hui, le problème c'est que tout le monde n'a pas un garage, tout le monde n'a pas un terrain. Il y a ceux qui sont dans l'habitat collectif. Je ne doute pas que dans des parkings. On va réussir à s'organiser et cetera mais il y a tout le reste qu'on connaît dans les villes et j'allais dire même plutôt dans les centre-bourgs ces rues où vous avez un habitat qui est contigu où les gens n'ont pas de garage, non pas de Parking non pas de places qui sont définis devant chez eux. Et là les choses vont être beaucoup plus compliqué. Donc je voulais savoir où en était l'état des réflexions. Pour ces endroits plus complexe pour installer les bornes savoir où en était l'état des discussions. Avec les maires, mais les associations qui sont censés les représenter et si le sujet du coup été abordées puisque cette nouvelle organisation dans les communes et dans les villes, va coûter aux uns, aux autres beaucoup beaucoup beaucoup d'argent. Merci de votre réponse. Merci, madame la Ministre. Merci madame la présidente. Sur les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Effectivement diversité. De de du territoire des centre-bourgs de nos villes de de villages. Rend le le sujet. Important je veux quand même rappeler. D'abord, vous l'avez dit. Une part significative du territoire et. Est ainsi couverte puisque en milieu rural, dans les départements ruraux. Vous avez pas mal d'habitat individuel je ne mentionne pas les centre-bourgs que vous avez mentionné mais avec la une possibilité de se recharger sur une place privée. Loin de moi l'idée que tout le monde aurait un garage, un jardin et une maison. Donc dans ce contexte, l'État soutient de nombreux dispositifs pour faciliter l'acquisition l'installation de matériel de recharge dans les logements et je pense ici au crédit d'impôt mais aussi au taux de TVA réduit à 5 5 pour les bornes acheter pour des particuliers. Pour ceux qui hier. De nos collectivités territoriales plusieurs mais juste sur une mise en place pour soutenir ce déploiement en dehors des noeuds urbains à hauteur de collectivités territoriales. L'appel à projets stations de recharge autre puissance qui est dotée à cette heures d'une enveloppe de 300 millions d'euros dans le cas de France 2030 prévoit une une intensité des aides plus importantes pour le déploiement de stations situées en dehors des 10 principales métropoles urbaines. cette enveloppe de 300 millions et dans le, l'appel à projets stations de recharge autre puissance la banque des territoires et l'interlocuteur qui aujourd'hui proposent des dispositifs d'accompagnement de financement aux collectivités locales aux délégataire de collectivités au bailleur mais aussi aux propriétaires en copropriété. L'État est aux côtés des acteurs locaux. Plus de 60% des bornes aujourd'hui ouverte au public ont été installés sous la maîtrise d'ouvrage de collectivité ou d'établissements publics et la réalisation de schéma directeur dédié doit permettre aux acteurs locaux, d'être légitimement moteur dans le déploiement de ses infrastructures, avec un financement bien sûr faciliter auprès de la banque des territoires. Je vous remercie. Monsieur Woerth de laine merci. La parole est à monsieur Hervé Gillé. Merci madame la présidente, madame la Ministre, la décarbonation des transports routiers, la dépollution des milieux urbains nécessite une adaptation volontariste des flottes de véhicules professionnels et particuliers. La fin de la production et de la vente des moteurs thermiques en 2035. Interroge la capacité des constructeurs à réorienter leur gamme, notamment au niveau européen à la recherche de plus Value plus conséquente. Ces derniers produisent des véhicules électriques de plus en plus lourd, de plus en plus cher et de plus en plus consommateurs d'énergie. Les véhicules d'entrée de gamme et donc plus facilement accessibles pour les ménages modestes sont de moins en moins nombreux. Au bénéfice d'une concurrence internationale et notamment chinoise plus adapté et plus attractive. Qu'elle soutient la filière française. Pourriez-vous envisager pour faciliter la production de véhicules d'entrée de gamme. Avez-vous des exemples concrets ainsi vouloir réserver des primes d'aide à l'achat au constructeur européen. À l'instar des États-Unis, reviendrait à empêcher les ménages modestes de s'équiper, afin de ne pas être pénalisé par l'alourdissement des fiscalités sur les aires Nýherji carbonés et la mise en place des ZFE. En d'autres termes, toujours plus de discrimination. Envisagez-vous ce ciblage des primes vers les constructeurs européens et donc une forme de protectionnisme. Pour accompagner les ménages les plus modestes. Où en êtes-vous du lancement d'un dispositif de leasing social facilitant l'accès aux véhicules propres, notamment pour faciliter l'accès aux ZFE par ailleurs de nombreuses études confirment l'intérêt de développer une filière de production de véhicules intermédiaires donc léger pour les mobilités du quotidien nécessitant moins de puissance et donc plus accessible pour l'ensemble des utilisateurs. Quel intérêt portez-vous sur ces nouveaux concepts. Le gouvernement serait-il favorable à soutenir et développer ces filières à l'échelle nationale. Je vous remercie. Merci madame la ministre. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, Gilles. Si vous m'autorisez, je commence déjà par répondent sur le leasing social. Oui. En 2024. C'est loin mais ça suppose aussi qu'on s'en parle enfin du moins que vous en parliez j'imagine et que vous soyez au côté. Du du ministre bonne en charge des transports. Moi c'est l'information dont je dispose et ça suppose aussi qui est sûrement une concertation en amont, ce qui me semble de bon aloi pour nourrir le projet. Mais il sera mis en oeuvre en 2024. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas y travailler là au 2ème semestre par exemple, pour ce qui est ensuite du sujet absolument majeur de la concurrence internationale. Oui vous avez raison, vous avez évoqué l'inflation réduction Act américain. L'IRA prévoit un crédit d'impôt pouvant atteindre 7500 dollars pour les particuliers achetant un véhicule électrique assemblé en Amérique du Nord et dont les batteries satisfont une exigence additionnelle de contenu local. Cette mesure, c'est une aide publique. Manifestement incompatible avec le droit de l'Organisation mondiale du commerce qui comme vous le savez aussi bien que moi interdit une manière générale à ses membres de favoriser leurs produits nationaux par rapport aux produits importés. Nous n'avons pas du tout l'intention de rester inactif face à l'IRA. Bruno Le Maire est en train de travailler en ce moment même. Avec le ministre de l'Industrie Roland Lescure à la préparation du projet de loi réindustrialisation verte dont je ne doute pas, pour avoir le plaisir de travailler avec lui depuis maintenant 3 ans qu'il associera en amont tout à la fois les députés mais aussi évidemment les sénateurs. Nous travaillons très sérieusement à des critères. Notamment environnementaux. Qui permettrait de réserver nos aide à l'acquisition aux seuls véhicules fabriqués en France ou en Europe. C'est donc une invitation. Qui sera d'ailleurs conclu et conclusif dans les prochaines semaines à travailler si vous le souhaitez et être force de nos de propositions sur ce sujet dans le cadre du projet de loi réindustrialisation verte. Les critères sont en cours. Merci. Merci Monsieur Gillet. Vous avez 16 secondes. Merci madame la présidente. Mais vous voyez bien l'objet. Pour que les gens qui ont des faibles moyens puissent acquérir des véhicules encore Fourtic que ces véhicules ne soit pas trop onéreux. Or, à l'heure actuelle, on a une dérive. Donc comment fait-on pour que les producteurs français produisent des véhicules qui sont pas chers.

Conseil et Parlement européens ont entériné la fin de la vente des véhicules à moteur thermique dans l'Union européenne pour 2035 au profit de véhicules 100% électriques. Ce choix politique suscite des interrogations légitimes. À titre d'exemple, la massification de la voiture électrique entraînera une hausse significative de la consommation d'électricité en France. Or notre consommation électrique a stagné pendant 20 ans, en dépit des aléas conjoncturels. Par conséquent, je me demande si notre système de production électrique peuvent vraiment monter en puissance. Nous avons tous encore en tête les exhortations du gouvernement à la sobriété pour éviter coupures des délestages cet hiver. Cela ne rassure donc pas sur cette question. Alors certes, le gouvernement semble avoir pris la mesure de l'urgence avec 2 projets de loi visant à accélérer l'un la production. Et l'autre les procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires, mais les premiers mettront sans doute plusieurs années avant de fonctionner. Quant aux secondes, elles ne seront jamais prête à avant 2035. Par conséquent, je voudrais savoir comment le gouvernement compte-t-il résoudre l'équation d'une consommation électrique augmentant plus rapidement que la production d'électricité ne serait-il pas pertinent d'envisager d'autres solutions comme le biogaz qui présente un intérêt certain pour décarboner la beau mobilité des poids lourds. Je vous remercie. Merci madame la ministre. Merci madame la présidente, madame la sénatrice Sempé. Merci pour votre question, vous vous interrogez le gouvernement sur le risque de notre système énergétique d'un accroissement. De la consommation d'électricité en France. D'abord une étude que j'imagine vous connaissez, publié en 2019 par RTE a démontré l'impact de la mobilité électrique sur la consommation électrique française. J'ai perdu quatre secondes pardon. Pardonnez-moi, madame la présidente. Cette étude désolé confirme. Que le système électrique français peut absorber le développement du véhicule électrique avec pilotage limitée de la recharge la consommation totale d'électricité des transports individuels et collectifs. Pèserait au plus un dixième de la consommation d'électricité totale en France à échéance 2035. C'est moins que la consommation du chauffage résidentiel. C'est moins que l'augmentation de la consommation électrique de la France entre 2000 et 2010. ne voudrais pas que le sénateur Babary. Tout ceci, on ne va pas y arriver. Pardonnez-moi, j'ai une quinte de toux. Désolé. Je suis désolé. Non non mais. Il va retrouver mon souffle ma voix et je suis là pour répondre aux questions, pardonnez-moi. Je vous remercie. Donc c'est moins que la consommation du chauffage résidentiel, c'est moins que l'augmentation de la consommation électrique de la France entre 2000 et 2010. Par ailleurs, la consommation énergétique additionnel qui est nécessaire à l'électrification du parc pourrait en grande partie être justement. Par les gains d'efficacité énergétique dans les autres secteurs comme le logement par exemple puisque nous menons en parallèle comme vous le savez une vaste politique de rénovation énergétique. Par ailleurs le pilotage dits intelligents de la recharge peut permettent de lisser les besoins de consommation pour éviter les pointes de consommation qui sont gourmandes en énergie et qui entretiennent le besoin d'importation ou la nécessaire production d'énergies fossiles. Le développement d'outils intelligents de recharge sera une des clés de la soutenabilité des véhicules électriques et pourraient apporter un élément de réponse aux besoins grandissants de flexibilité du réseau électrique. Vous questionnez enfin à madame la sénatrice, la possibilité d'utiliser le biogaz pour la mobilité. Le bilan carbone du biogaz peut certes concurrencer celui des véhicules électriques. Mais l'analyse du cycle de vie a ses limites. Elle ignore la disponibilité concrète et les coûts liés aux technologies. Or le biogaz à une disponibilité actuels et futurs limité. et sa large distribution n'des investissements forts ces de contraintes ne permettent pas à cette heure d'en faire une alternative à l'électrique pour décarboner les voitures ou les utilitaires légers. C'est donc pourquoi nous recommandons de réserver les ressources limitées de biogaz pour des secteurs qui sont déjà dit pendant du gaz plutôt que de créer une demande supplémentaire dans un secteur du transport où il existe des technologies plus adapté, plus mature, pardonnez-moi.

de ne pas utiliser le biogaz, qui est une ressource présente sur les territoires. Je vous remercie. Metz. Même la nuit. Pas de réponse pour l'instant.

Soit connu pour sa propension à d'utopie mais. Je je je comprends vos doutes encore une fois le la bascule. Elle est elle est majeure et le doute et et salutaire mais je me permets de vous vous renvoyer à cette étude. Pour ce qui est du bogue Objection retenue du moins entendu. Et et je suggère peut-être qu'avec la ministre de l'Énergie auquel je peux tout à fait faire un message vous vous en discutiez plus profondément. Je ne suis peut-être pas aussi spécialiste que vous madame la sénatrice, je vous remercie. Merci, même. C'est bon.

Merci madame la présidente, madame la Ministre, la France nourrit comme d'autres pays des objectifs de développement des véhicules électriques. Plus qu'une promesse, c'est un incontestable défi pour la filière automobile mais qui cache mal aujourd'hui un certain nombre de difficultés. Première difficulté, ça a été dit dans le contexte délicat d'abandon manifeste du nucléaire, la puissance électrique en France et de plus en plus questionné. Il y a aujourd'hui en France environ 44 millions de voitures concernées après 2035 pour l'électrification le remplacement massif de véhicules thermiques par des véhicules électriques va démultiplier la consommation électrique qui va accroître d'environ 25% par rapport à aujourd'hui, mais pas seulement. Seconde difficulté, nous avons aussi à faire face à des très fortes tensions sur certains matériaux. Je pense notamment semi-conducteurs nous avons enfin face à la radicalité à la généralisation des ZFE, un problème de souveraineté industrielle alors qu'il faut accompagner les Français massivement vers la transition électrique les aides actuelles pour ceux qui peuvent se permettent d'acquérir une voiture électrique bénéficie très majoritaire Ritter ment à l'achat de voitures étrangères alors que notre pays, clame l'urgence de s'en doter la France et même l'Europe sont littéralement à la remorque de la Chine de sa puissance de frappe actuelles sur la construction de voitures électriques et de batteries. Madame la Ministre force est de constater que ce sujet vire au casse-tête retard sur les bords de retard sur le matériel coût prohibitif empreinte carbone de la production. Coût de l'énergie, rejet des ZFE aussi fort de tous ces éléments, les objectifs de fin de vente des véhicules termine après 2035, vous semble-t-il et s'il vous plaît, répondez-moi sereinement objectivement et honnêtement toujours. Pouvoir être atteint. Merci madame la ministre vous avez la parole. Avec beaucoup de questions. Merci madame la présidente, et je prends volontairement 4 secondes pour remercier très honnêtement, très sincèrement, parce que c'est quand même ma façon d'être et d'être honnête et d'être sincère. La bienveillance de madame la présidente, qui m'a permis de retrouver mon souffle et la gentillesse des sénatrices qui m'ont offert quelques pastilles et de quoi reprendre mon souffle. Je ne vous cache pas qu'en 6 ans. De parlementaires et de ministres je j'ai rarement été. Entouré d'autant de bienveillance. Donc je prends 15 secondes et pas 15 minutes pour vous en remercier très sincèrement. mais c'est, qu'est-ce que vous voulez, c'est je perds mon souffle à les idées qui met juste merci pardonnez-moi. Non non mais c'est pas parce qu'on n'est pas toujours d'accord qu'on est obligé en plus humainement d'être dur les uns avec les autres donc, merci. Bon sur le le le constat. Je je l'ai dit à la sénatrice du Var. Il y a quelques instants, ça n'est pas parce qu'on a pris un petit peu de retard sur l'installation des bornes dans un contexte assez difficile, liées et vous l'avez mentionné monsieur le sénateur aussi à la pénurie de semi-conducteurs à une Inès complexe d'ailleurs surtout les entrants, que ce soit dans le milieu artisanal, comme dans le milieu industriel. Qu'on n'arrivera pas. Viser l'objectif d'ailleurs, je partage avec vous le faites que sur la pénurie des semi-conducteurs. Et le ministre de l'industrie et de l'économie s'y sont attelés. Il y aura, il y a déjà du mieux. Il y aura du mur en 2023 On s'y atteler. Tout au long de l'année précédente et je rappelle quand même sur les bornes que nous sommes le 3ème pays d'Europe. Vous m'avez demandé une réponse. Sincère, honnête et. c'est un, c'est un autre débat. Surtout quand on a un peu un problème de souffle mais je suis sereine sur le fond, pour vous répondre. Sur les chiffres-clés. Je pense qu'on peut. On peut y arriver. On a aujourd'hui. En 2022, 1,5 millions de véhicules particuliers vendus. Et 1,3 millions de véhicules particuliers. Dont 100.000 véhicules électriques. L'objectif en 27 million de véhicules électriques fabriquées en France en 32 millions de véhicules électriques fabriquées en France. L'estimation d'un parc électrique à 20% en 2030 avec 8 millions de véhicules et à 45% en 2035 avec 18 millions de véhicules me semble possible. Sans faire référence à d'autres débats en cours pour le coup, à l'Assemblée avant qu'il arrive ici. Je crois qu'en matière de flux. Nous pouvons y arriver si on n'oublie pas ce que j'ai dit au tout début, qui est le rétrofit, c'est-à-dire notre capacité à transformer aussi des véhicules thermiques en électriques pas uniquement à construire de l'électrique mais aussi à investir sur le rétrofit et la transformation donc honnêtement sereinement, j'y crois. Merci. Monsieur Tabarot. Vous avez 11 secondes. C'est, c'est bon. C'est bon je. La la ministre m'a pas répondu sur les ZFE mais de toute manière c'est un, un sujet qu'on aura dans les mois et les années à venir, malheureusement quand leur mise en place particulièrement difficile sur les territoires. Merci. accord. Je vais donner la parole à monsieur Joël Bigot. Madame la présidente, madame la Ministre, la décision de l'Union européenne d'interdire la vente de véhicules thermiques neufs à horizon 2035 est en train de bouleverser le marché automobile. Selon un rapport récent de la Fédération des acteurs de la mobilité électrique. Les prévisions de croissance sont exponentiels électrique passerait de 1,5% du parc français roulant à 24% en 2035. Néanmoins cet engouement est tempéré par le déploiement difficile des bornes de recharge qui sont toujours en deçà de l'objectif des 100.000 fixé par le gouvernement pour 2022. Mais vous avez répondu tout à l'heure à monsieur Corbizet que cet objectif serait atteint en 2023. Dont acte. À l'heure de la planification écologique. Où est le rôle de l'État dans le déploiement des bornes de recharge et de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire. C'est une condition sine économe du développement de l'électrique quand on quand l'autonomie des véhicules électriques ne dépasse pas les 300 kilomètres. C'est un véritable enjeu en région Centre Val de Loire ou encore en Pays de Loire où cette dernière ne compte que trois 86 points de recharge pour 100.000 habitants, ce qui est très en deçà de la moyenne nationale. Comment l'entend l'État entend-il assurer une répartition équilibrée du réseau sur l'ensemble du territoire, y a-t-il une attention particulière portée aux territoires peu denses afin de garantir l'égalité territoriale et un maillage intelligent, 83% de nos concitoyens vivent en zone rurale et sont donc par le manque d'offre de mode et mobilités alternatives pour. Utiliser quotidiennement leur vie leur voiture individuelle aussi, le gouvernement prévoit-il un plan spécifique de soutien à l'électrification des mobilités du quotidien pour ces zones rurales, une enveloppe de 10 millions a été débloqué en fin d'année dernière, mais on est encore bien loin des besoins locaux identifiés par l'Insee dans les zones rurales et périurbaines. Contrairement aux idées reçues. Je vous remercie. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur. Nous aurons-nous 100.000 bornes en fin d'année 2023. Dans un contexte que vous connaissez aussi bien que moi. C'est un retard je reste honnête. De sénateurs sénateur. Je pense que c'est un retard qui peut s'entendre si ce n'est se comprendre. Ce qui est important c'est qu'on arrive à l'objectif, voir qu'on le dépasse le plus vite possible et quand on voit les chiffres on y arrivera. Le sujet que vous mentionnez est absolument majeur et j'en ai, j'ai essayé, du moins de commencer à y répondre. Lors d'une question précédente. Il est indispensable que les collectivités locales jouent leur rôle dans cette planification territoriale. d'abord sur le volet recharge stations de recharge rappelle que là on ne parle pas 10 millions d'euros. L'appel à projets qui a été lancée dans le cas de France 2030. Ces 300 millions d'euros pour justement assurer une intensité d'aides plus importantes dans les territoires pour pour les installer des stations dans les territoires qui sont situés en dehors des 10 principales métropoles urbaines. Par ailleurs, je le redis, la banque des territoires est aux côtés des collectivités territoriales et propose différents dispositifs d'accompagnement financier pour justement accompagner nos collectivités territoriales les délégataires de collectivités, les bailleurs, notamment dans cette planification territoriale. Enfin, l'État est aux côtés des acteurs locaux, dont l'engagement a été son ciel. Plus de 60% des bornes aujourd'hui. Ont été installés. Je le répète, sous la maîtrise d'ouvrage de collectivité ou d'établissements publics et la réalisation de schéma directeur dédié va permettre aux acteurs locaux, d'être moteur dans le déploiement de ses infrastructures. Vous ne le connaissez. Le fonds Vert doté de 2 milliards d'euros. Dont. Nous pourrions imaginer si les par si la volonté de la représentation nationale et celle-ci qu'on isole, peut-être une petite partie sur cette masse des 2 milliards d'euros, peut-être pour renforcer. La problématique de de du développement des recharges mais aussi des infrastructures dans les collectivités territoriales. Pourquoi pas en parler directement avec le ministre Béchu. C'est une option qu'on pourrait regarder je vous remercie. Merci. Alors vous avez. 12 secondes. Monsieur Bigot. Oui, je vous remercie madame la présidente, donc j'habite pas très loin de chez le ministre-Béchu donc je pourrais vous lui poser directement la question mais en tout cas quand vous avez une course de plus de 300 kilomètres à faire et que vous habitez une zone peu dense. Vous hésitez à prendre votre véhicule électrique. Donc c'est une urgence. Merci. Alors la parole est à madame Véronique Del Fabro. Merci madame la présidente, madame la Ministre, comme l'ont dit précédemment, mes collègues en 2035, les concessionnaires automobiles ne pourront plus maître de véhicules thermiques neufs en vente je m'aurait eu jury pour 2 raisons, la première écologique et la seconde est que cette mesure répond aux attentes des territoires ruraux que je me permets de représenter aujourd'hui à condition qu'il y ait des infrastructures. Les habitants des zones rurales sont fortement dépendants de leur voiture. La crise des gilets jaunes nous a bien démontré le lourd tribut payé par les usagers dépendants des énergies fossiles rouler à la campagne coûte plus cher qu'en ville, sauf peut-être si on dispose d'un véhicule électrique à la campagne, le développement des infrastructures de recharge. Va jouer un rôle majeur en matière de mobilité. Or force est de constater que le déploiement des bornes de recharge et laborieux dans nos régions rurales. C'est pourtant une condition sine qua donne du développement de la mobilité, nous voyons certes fleurir des initiatives, territoire par territoire par l'action de l'ensemble des collectivités parfois de concert, je vous l'accorde la France des 35.000 communes ne doit pas devenir celle des 35.000 habitants abonnement nécessaire pour accéder aux 35.000 bornes de recharge des véhicules accessibles au public. pensez-vous que le déploiement des bornes de recharge constitue le véritable enjeu de développement et d'aménagement du territoire. Si oui, quel rôle et place l'État entend-il tenir dans la question majeure de l'interopérabilité, notamment en matière de transport de Merci, madame la Ministre. à l'aune de la générosité des sénateurs et des sénatrices et de leur bienveillance. Le reste de mon temps parce que je j'ai déjà répondu sur les bornes. Et et je j'ai pas beaucoup d'éléments à ajouter. Merci madame Delph, à Bron. Il vous reste 32 secondes. Sauf à répondre sur la transparence. Je vais juste vous. Vous parlez de mon expérience puisqu'il y a quelques semaines on va dire au mois de décembre, j'étais encore maire d'une commune rurale de 360 habitants et vice-, présidente d'une communauté de commune. Dans un souci écologique. J'ai acheté un véhicule électrique oh regardez il me faut, je ne sais pas combien de carte pour pouvoir recharger mon véhicule sur le territoire de plus sur une même bornes avec 3 cartes. J'ai dit à totalement différents qui vont de 35 centimes

Non non même. Les enjeux sont trop importants pour que nous ne fassions que jouer au jeu de la minute. J'en dis que ce n'est pas une option, madame la sénatrice, j'en dis que je comprends. Votre agacement fort agréable d'ailleurs et je vous remercie d'être resté agréable. en parlant de transparence, vous êtes. Très sympathique. C'est un vrai sujet. J'ai pas l'expérience que vous avez, j'ai, je ne suis que député de Paris et je n'ai pas l'expérience de la commune rurale que vous avez c'est pas normal et ça doit être un sujet, je n'ai pas en charge cet immense périmètre le mien est déjà. Maousse costaud pour la référence mais je pense que c'est un sujet qui doit être urgemment traiter et je suis à votre disposition pour le faire passer à notre ministre de la transition énergétique, madame Agnès Pannier-Runacher. Ça n'est pas un sujet. Une option qui est autant d'opacité et surtout autant de cartes et autant de manque de praticité dans ces pratiques. On veut développer. Si je peux me permettre à Madame la Ministre alors Madame madame. C'est c'est moi qui qui redonne la parole. Juste. Donc. Vous, si vous voulez, vous avez une minute pour répondre. Excusez-moi madame la présidente. C'est ma première question. Donc il faut que je me plie à l'exercice. Madame. Madame la ministre, lors de votre venue en Meurthe-et-Moselle, je serai ravi qu'on échange sur ce sujet. Merci madame la présidente, madame la Ministre. Carlos Tavarès, directeur général de Stellantis tente depuis de nombreux mois de casser les idées reçues sur les voitures électriques. Il n'est pas le seul mais nul ne semble l'entendre d'abord en raison de la très mauvaise empreinte carbone liée à la fabrication des batteries électriques, un véhicule électrique doit rouler 70.000 kilomètres pour commencer à être positif sur le plan environnemental, par rapport à un véhicule thermique ensuite la production d'un véhicule électrique est plus onéreuse que celle d'un véhicule thermique environ 50% de plus avec aujourd'hui un minimum quasiment de 30.000 euros, la différence n'est pas l'épaisseur du trait, les classes moyennes françaises ont-elles vraiment les moyens de supporter cette différence. Nous ne pourrons continuer à faire des chèques qui bénéficie à notre essentiellement à l'industrie automobile chinoise, nous l'avons dénoncé lors de l'examen du PLF. La question du réseau de bornes électriques, elle a largement été évoquée reste aussi un grand sujet d'inquiétude, partout en France bien sûr mais peut-être plus encore sur les aires d'autoroute pour accueillir simultanément beaucoup de véhicules. Enfin, et sans parler de notre production électrique, tant en quantité que au niveau du cou. Il y a le sujet de l'emploi et de la mutation profonde et rapide de notre industrie automobile avec tout ceci on prépare un gigantesque plan social pour l'industrie française. Il y aurait donc beaucoup de questions, je vais me limiter à deux. Que comptez-vous faire pour défendre nos entreprises et nos emplois par rapport à la à l'avancée du monde du véhicule électrique qui est aussi une opportunité, j'en conviens et surtout même si je suis un élu de la ruralité. Comment envisagez-vous l'accueil d'un parc tout électrique sur les aires d'autoroute. Demain je vous remercie. Merci, madame la Ministre. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur Sautarel. Première question. Déjà un, un soutien massif de l'État. Je, je le rappelle, même si. si. Peut se lasser. En sortant de la période du quoi qu'il en coûte mais ça n'est quand même pas anodin. 5 milliards d'euros dans le cadre de France 2030 dont je le redis. Un milliard d'euros directement fléchée pour soutenir nos sous-traitants et pour certains l'évolution de nos sous-traitants qui vont être aussi impacté. Par le développement des véhicules électriques. 2ème réponse monsieur le sénateur. À l'aune de ce que j'ai dit il y a quelques instants et vous aurez ce débat et je sais que vous serez force de proposition. Il nous faut trouver les voies et moyens pour que ce soit nos entreprises. Européennes qui bénéficient du développement de ces véhicules électriques. Bruno Lemaire prépare en ce moment avec Roland Lescure. Le projet de loi réindustrialisation verte hein on n'est pas ici dans, de l'utopie. On est vraiment sur le réel du semestre du 1er semestre 2023. Je ne doute pas que vous serez. Très prochainement, si ce n'est pas déjà le cas. Ceci pour pour y travailler et nous travaillons à des critères, je ne rentrerai pas plus dans les débats dans le cadre de cet échange, mais je ne doute pas que Bruno Lemaire le fera, nous travaillons à des critères pour faire en sorte que, comme les Américains le font comme l'Asie ne se prive pas de faire on puisse aussi encourager l'achat de nos véhicules européens sur le territoire européen. Il me semble que c'est la meilleure façon aussi de soutenir nos entreprises au-delà du soutien Direct de l'état du plan France 2030 aux autoroutes et installation de bornes de recharge. Sur le réseau routier national. D'abord on on a à consacrer une enveloppe de 100 millions d'euros au développement des stations de recharge, vous le savez. Ce dispositif a permis d'équiper 3800 points de recharge tout au long du réseau routier national en visant une station tous les 60 kilomètres sur le réseau concédé sur le réseau routier national concédé environ 85% des aires de service sont d'ores et déjà équipés et elle devrait toutes lettres à 100% courant 2023. Merci monsieur Sautarel, vous avez 23 secondes. Merci, madame la Ministre pour ces éléments de réponse, effectivement je reviens pas sur le la dimension industrielle qu'on aura l'occasion de de révoquer par ailleurs. Je, je me posais juste une question sur les aires d'autoroute, au-delà de de de leur équipement. C'est sur les surfaces qui seront nécessaires parce que je m'interroger sur le calcul avait été fait par rapport au nombre des véhicules en période de pointe et le temps de recharge par rapport au au temps de remplissage d'un réservoir et les objectifs de la zéro artificialisation nette par ailleurs si elle est pas falloir étendre considérablement nos aires d'autoroute. Merci.

à tout. Pas très la plus compétente mais je pense que c'est un point important. Alors je ne sais pas si vous habitez comme Monsieur le Sénateur, pas très loin de Christophe Béchu pour le poser la question, mais ce que je sais c'est que le ministre des Transports et ministre de la transition écologique travaillent main dans la main, ce que vous pointez monsieur le sénateur est un vrai sujet possiblement même un, un, un, un angle mort et je suggère que la question et je suis à votre disposition si il faut faire passer la question mais soit posé assez rapidement au cabinet des ministres que je viens de mentionner, c'est un vrai sujet. Merci monsieur Sautarel.

Il a affirmé que l'offensive chinoise était attendue et qui, c'est l'Europe qui a provoqué les conditions d'une très rude bataille. Ses propos ont été les suivants. Si l'Europe ne veut pas que son industrie automobile disparaissent d'ici 2035. Il faut la protéger. Nous ne refusons pas la compétition, nous voulons uniquement à des conditions équitables pour se battre contre les Chinois. En fait travailler sur la production vers d'électricité en Suisse sur les réseaux puis alors seulement sur les véhicules totalement électriques. Il a ajouté la décision dogmatique de ne vendre que des électrique en 2035 a des conséquences sociales inacceptable la couche de doit être complétée par la couche de pragmatisme même Thierry Breton, commissaire européen mis en doute la faisabilité de l'échéance 2035. Sénateur du tout territoire particulièrement impacté. Je m'interroge sur cette échéance. Les conséquences économiques et sociales comme d'autres régions ne sont pas réellement mesurer. La fragilité de tous les prévisionnel est l'absence d'étude publique d'impact sérieuse ajoute à ce grand point d'interrogation. Une telle marche forcée ne peut avoir pour conséquence une destruction massive d'emplois. Je passe, je parle en particulier pour le Doubs et le bassin automobile historique Sochaux-Montbéliard c'est dès aujourd'hui qu'il faut s'interroger dans 10 ans elle sera trop tard. Le défi est immense coup fabrication chez une des valeurs métaux rares. Je vais témoigner ici au Sénat, la grande inquiétude de tout un territoire et de leurs habitants, ainsi que du monde économique des sous-traitants mais aussi des élus. Le gouvernement ne peut se satisfaire devant ses inquiétudes de quelques aides ponctuelles et inaccessible à beaucoup ou d'Assystem subventionné trop complexe. Comment Madame la Ministre, pouvez-vous Merci madame la présidente, monsieur le sénateur. Il y a des éléments. Et il y a effectivement les prises de parole que vous êtes nombreux à citer de président Carlos Alvarez. Il y a des doutes que vous mentionnez et j'en parlais il y a pas si longtemps avec le commissaire breton. Aujourd'hui on a un taux de pénétration des véhicules chinois. Estimé à 18%. En 2025. À 805% aujourd'hui, 18% en 2025. Donc les chiffres corroborent. L'analyse pour autant et c'est l'objet de tout ce que j'ai essayé de partager avec vous on est en train pas demain, pas en 2025 mais on est en train de travailler, à bâtir une toute une filière. Avec des des soutiens massifs d'État. je le redis. 5 milliards. Directement dans le cas de France 2030. Dont encore une fois un milliard spécifiquement dédiés. Monsieur le sénateur, à nos sous-traitants dont je sais que. Dans votre circonscription, ils sont nombreux. Par ailleurs, compte tenu de, de l'ampleur du mouvement a opéré, compte tenu de l'ensemble de ses effets de bord des effets d'aubaine et des risques que je ne nie pas que le gouvernement ne nie pas. Je rappelle. Qu'une clause de revoyure est prévue en 2026. Aussi pour d'autres technologies à faibles émissions comme les carburants alternatifs qui pourrait. Comme certains d'entre vous l'ont suggéré tout à l'heure peut être aussi renforcer un peu le mix énergétique et ne pas le laisser uniquement reposer sur l'électrique, donc la clause de revoyure, elle est prévue en 26 et. En attendant 2026, nous avançons, nous bâtissons. Véritablement, pas uniquement sur les batteries et c'est aussi le sens de mes interventions, mais sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de lithium. Il y a quelques minutes sur les métaux critiques, nous nous dotons au sein de l'état aussi d'une organisation et on verra à la clause de revoyure mais je j'entends vaudou. Merci. Vous avez 7 secondes, pas une de plus. je remercie la milice pour sa réponse mais ça monte véritablement que l'Europe a fait tout à l'envers en imposant l'industrie automobile de produire des véhicules électriques si rapidement. Merci. La parole est à madame Laurence Muller-Bronn. Merci madame la présidente, madame la ministre. L'Union européenne a interdit à partir de 2035, la vente de véhicules neufs à moteur essence ou diésel. 450 millions d'Européens sont concernés. Nous sommes les seuls à avoir fait ce choix. Ni les États-Unis ni le Japon ou la Chine ne se fixe de tels objectifs en misant tout sur l'électrique. Carlos Tavarès, encore lui, directeur général de Stellantis a lui-même déclaré la voiture électrique. C'est un choix politique qui aura des conséquences économiques, sociales et même environnementale négative. Nous refusons d'être tenu pour responsable. Dans 10 ans pour un choix que l'Europe nous a imposé. La solution réaliste réside selon lui dans le véhicule hybride. Avis partagé par le patron de Toyota, qui nous alerte également sur les chimères du tout électrique. Sur le plan social d'abord, nous l'avons vu le véhicule coûte trop cher et sa production entraîne la disparition des activités sous-traitante artisanal ou industriel. Ensuite, sur le plan économique, cette industrie implique un investissement public lourds nous l'avait entendu pour équiper le pays à la mobilité tout électrique. À cela il faut ajouter les subventions à l'achat enfin avec la flambée du prix de l'électricité, les concessionnaires nous le confirme la chute des ventes a été brutal au cours du 3ème trimestre 2022 sur le plan environnemental. Enfin, il s'agit d'une fausse promesse pour obtenir une tonne de lithium, il faut un million de litres d'eau. Plus grave, nous savons que les conditions d'extraction, loin de l'Europe sont inhumaines, dangereuses et polluantes alors Madame la Ministre pour les alternatives sérieuses existent comme l'hydrogène, les biocarburants ou le carburant synthétique décarboné qui permettent de conserver les moteurs thermiques en 2035, elles seront viables. Pourquoi ne pas avoir laissé le temps aux industriels européens de les développer. Merci madame la présidente, de multiples questions. Abordées je. Je rappelle quand même ce que je disais dans ma. Dans ma prise de parole initiale. Aujourd'hui si on veut. Si on se refixe. l'objectif de neutralité carbone à 2050 qu'on peut aussi d'ailleurs remettre en question tous tes a vocation à être possiblement remise en question. Il y a un moment où. La planète. Elle ne se posera plus de questions. Et les les futures générations non plus. Mais je suis et je sais pas si vous me connaissez plutôt modéré en la matière mais je rappelle quand même l'ampleur aussi du de la bascule qu'on a à mener ensemble et, et comment arriver à cette neutralité carbone européenne en faisant fi. Dans le secteur des transports. Qui est massivement émetteur. Jour là appels d'au moins 30% des des des émissions de gaz à effet de serre. Les commentaires. Des présidents de structures automobile. Relève des commentaires et je n'ai pas à les commenter en l'occurrence et chacun a son point de vue moi j'ai à coeur de vous rappeler quand même que. Même si elle pollue moins. La voiture hybride elle elle pollue quand même elle pollue tout de même. J'ai aussi à coeur de, de rappeler que. Les porteurs. De messages parce que tout transport motorisé pollue, vous le savez, quel que soit son mode de propulsion mais les porteurs de messages négatifs sur le véhicule électrique ne prennent souvent en considération qu'une partie du cycle de vie et non pas sa globalité se centre uniquement sur le CO2. La fabrication d'un véhicule électrique, elle demande plus d'énergie, vous l'avez mentionné, du fait de la production de la batterie pour l'instant et vous avez été nombreux à lire les batteries sont majoritairement produite en Chine, mais aussi en Pologne. Pays dont le mix énergétique resterait carbonées et donc c'est pourquoi on se bat, on construit les j'usine de batteries électriques. C'est pourquoi d'ici 2027 on devrait être autosuffisant pour équiper nos véhicules électriques fabriquées en France et qu'on pourra ensuite possiblement les exporter je je vois pas bien comment on arrive à une neutralité carbone horizon 2050 sans s'attaquer au sujet du véhicule thermique et donc sans fixer des ambitions que j'entends que vous jugez irréaliste et encore c'est la liberté de commenter et d'avoir son avis, je vous en remercie.

On aurait pu changer un terme en disant est-ce souhaitable. Tant les points de vue. Je veux remercier les différents intervenants et évidemment bien sûr Madame la Ministre puisqu'on a eu à la fois des points de vue très concret des questions et des réponses. Les questions pertinentes et des réponses étayées. Mais on voit que dans le double objectif d'avoir une production automobile décarboné et de lutter contre la pollution automobile. Il y a encore un vrai travail, y compris en terme de meilleures connaissances et je terminerai par là de mon propos, dans quelques instants sur l'analyse du cycle de vie, à la fois de la production automobile et de son utilisation. elle concentre aujourd'hui les défis les plus important me semble-t-il de la transition écologique, économique et du lien avec la liberté. Auquel nous sommes partiellement attaché de pouvoir nous déplacer en conséquence de quoi, oui bien sûr il faut verdir le parc automobile. Vous avez, vous êtes tous rentrer dans cette logique avec. Plus ou moins d'envie en tous les cas. Certain étant moins jusqu'au-boutiste que d'autres, notamment par rapport à la date couperet de 2035 ou je crois. Nous devons entendre d'ores et déjà les interrogations. Je ne crois pas effectivement a-t-il persuadé non plus qu'il faille s'orienter vers une seule technologie ça n'est jamais bon notamment lorsque. Cette technologie vient à rencontrer des difficultés. La création d'une filière industrielle. Avec différentes étapes et notamment en espérant un bonne aménagement du territoire par les unités de production a été madame la Ministre, à mon avis à juste titre, rappeler avec, d'une certaine manière un triptyque besoin de formation. Qualifiée à tous les échelons, une production automobile si possible française et européenne et donc une capacité d'exportation de notre production pour servir évidemment notre balance commerciale qui soit dit en passant on a grandement besoin et la filière automobile perd des parts de marché actuellement et puis c'est un enjeu de mobilité propre qui passe par je je le l'exposé par cette liberté à laquelle nous sommes attentifs mais notamment par un maillage territorial ou à la fois il faut disposer d'unités de recharge à travers le pays, là où il y a de grands flots de circulation, on pense aux aires d'autoroutes, mais également un peu à l'instar de ce qui existait il y a quelques décennies à travers la France où il y avait beaucoup de stations essence, nous avons besoin de nous aurons besoin, pour la mobilité électrique d'être au plus près des territoires pour ça la date, je l'ai dit, de 2035. Plusieurs d'entre vous, je pense notamment aux sénateurs Chauvet qui a été le 1er à nous alerter. Attention de ne pas en faire une date couperet par un choix technologique exclusif qui pourrait d'ailleurs être hâtif, raison pour laquelle je veux le redire. Il faut regarder de près à la fois les biocarburants, le rétrofit de vous l'avez dit, mais également l'hydrogène. Un panel de solutions me semble préférable. Et puis le défi qui est devant nous, il est, il est aussi je le disais, celui de la, de l'aménagement du territoire qui doit concilier la transition écologique, la justice sociale mais aussi la réussite économique dans tous les territoires. Ça ne veut pas dire qu'il faut des unités évidemment vous l'avez compris, j'entends le nord mais voilà chacun défend à la fois son territoire et je crois que là aussi il faut, il faudra imaginer. Avec une certaine forme d'Intelligence collective. Enfin je voudrais. Peut-être rappeler que. Dans ces filières autour de l'automobile, il y a pas que la. Production il y a ensuite la mise sur le marché et l'entretien et il va falloir déployer sur le territoire là aussi formation unité pour pouvoir entretenir et réparer ce sont des formations nouvelles, on n'y est pas, aujourd'hui, donc il y a un travail à faire et, enfin je l'avais dit je veux terminer sur le sujet qui à mon avis, résument parfaitement au final. Derrière l'enjeu économique qui est l'enjeu écologique de l'analyse du cycle de vie de la production des véhicules électriques et des batteries c'est majeur. Le gouvernement ne peut pas s'exonérer aujourd'hui de mettre ses réflexions en partage avec la représentation nationale de telle manière que les orientations qui seront définitivement arrêtées répondent aux besoins d'aujourd'hui madame la présidente, je voulais enfin vous remercier de votre rigueur souriante. Vous avez une parfaite maîtresse des horloges. Un grand merci. merci. Beaucoup c'est pas la peine de me dire ça pour me prendre quelques secondes quand même. Je. Vais suspendre quelques instants la séance pour permettre. À chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour, la séance est suspendue.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions. sont en discussion du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. La parole est à monsieur Didier Mandelli rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire et pour cinq minutes. Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Il y a plus de trois mois, notre assemblée a adopté à la quasi-unanimité le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. En complétant largement le texte du gouvernement. Après la lecture à l'Assemblée nationale. Une commission mixte paritaire conclusive. L'heure est venue de transformer l'essai. Le chemin que nous avons parcouru depuis l'Automne dernier n'a pas été sans écueils et sans difficultés notamment dans cet hémicycle. Mais à l'heure du bilan. Je pense pouvoir dire que cet effort collectif n'a pas été vain. J'ose le dire, le texte qui vous est soumis aujourd'hui fait largement honneur à notre travail à votre travail. Avant de présenter les évolutions notables apportées par la CMP j'aimerais rappeler les objectifs qui ont été ceux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable au nom de la laquelle je m'exprime aujourd'hui. Le renforcement de la planification territoriale. Du ration de la concertation autour des projets afin de passer d'une logique descendante à une approche ascendante, nous avions ainsi instituer un dispositif global de planification territoriale du déploiement des énergies renouvelables, mettant les élus locaux, au 1er rang desquels les maires à la manoeuvre pour définir les zones d'accélération des énergies renouvelables. Dans la même logique, nous avions proposé une planification spatiale dédiées à l'éolien en mer, notamment avec le principe d'une localisation prioritaire des parcs éoliens au sein de la zone économique exclusive soit à plus de 22 kilomètre du Rivage afin d'améliorer l'acceptabilité des projets de négociations qui ont été réalisées. En Direct dans cet hémicycle. Après une suspension de 2 séances en de la simplification des procédures applicables aux projets ENR pour réduire les délais de déploiement des projets des mesures destinées à simplifier le cadre des autorisations administratives avaient été introduites. Nous avions également mis en place un fonds de garantie pour couvrir les risques contentieux pesant sur les porteurs de projets. On prend la libération de surfaces artificialisées nous avions renforcé la couverture en énergie solaire des bâtiments non résidentiels et faciliter l'installation d'ouvrages renouvelables sur les bâtiments. la sécurisation juridique des dispositions du projet de loi par exemple en s'assurant que l'ensemble des énergies renouvelables soient bien incluses dans le Champ du texte ce qui. N'était pas le cas à l'origine. Force est de constater que le texte issu des négociations que nous examinons aujourd'hui conforte largement ses axes de réflexion. La grande majorité de nos produits, de nos propositions ont été conservés par l'Assemblée nationale la CMP. Celle-ci a permis des compromis confortant les positions exprimées par le Sénat. Ainsi, sur les 108 articles du texte final. 39 ont été introduits par notre chambre. Quelques suppressions d'articles et dispositions votées par le Sénat sont certes a déploré comme c'est toujours le cas. On a une c'est une CMP équilibré. Je note toutefois que la balance penche très nettement en notre faveur. Sur le fond, la version finale du texte et plus ambitieuse que le projet qui nous était soumis il y a quelques mois le texte Offres d'une part plus de leviers d'accélération pour le développement des énergies renouvelables. Il donne d'autre part des garanties qui favoriseront une appropriation territoriale des projets. Le dispositif de planification territoriale dans la version qui vous est proposé aujourd'hui répond tout particulièrement à cette double exigence d'accélération du déploiement et d'appropriation territoriale. Les négociations ont permis à notre initiative, de donner plus de corps aux zones d'accélération qui seront identifiés localement. On y prévoyant des mesures de simplification procédurale spécifique. Les négociations nous ont également permis de pérenniser plusieurs mesures de simplification administrative visant à accélérer l'instruction des projets d'énergies renouvelables. Nous avons aussi pu rétablir l'article 5 dans une version très proche de celle adoptée par le Sénat qui nous permettra aux côtés du fonds de garantie créatrice à notre initiative, de limiter le risque contentieux. Par ailleurs, la commission mixte paritaire, nous a permis de rétablir des apports importants qui contribueront à la solarisation des toitures des bâtiments non résidentiels existants de plus de 500 m2 devront par exemple être couvert par un dispositif de production d'énergie solaire ou un dispositif végétalisée avant 2028. Enfin les bâtiments neufs devront être prêts à accueillir des énergies renouvelables et les collectivités, collectivités territoriales, pourront déroger aux règles d'urbanisme pour les installations en toiture. En guise de conclusion. Il me reste à remercier les présidents de commission pour leur implication tout au long aux travaux. Sophie et. Jean François le rapporteur à Patrick Chauvet, ainsi que l'ensemble des groupes pour le travail collectif qui nous a permis d'améliorer le texte qui nous était proposé mes remerciements vont également aux aux administrateurs. Du Sénat. Et au rapporteur de l'Assemblée nationale pour la qualité des échanges préparatoires à la commission mixte paritaire et à vous Madame la Ministre pour le sens du dialogue dont vous avez su faire preuve dès l'origine et tout au long de l'examen de ce texte formons le voeu que la loi de programmation quinquennale que nous aurons à examiner courant 2023 nous donne à nouveau l'occasion devrait collectivement à l'atteinte de nos objectifs climatiques et énergétiques. Merci. La parole est à madame Agnès Pannier nager Ministre de la Transition énergétique.

Madame la présidente. Madame la présidente de commission. Monsieur le président de commission chère Sophie cher Jean François messieurs les rapporteurs chers Didier cher Patrick mesdames et messieurs les sénateurs. Le projet de loi sur l'accélération de la production des énergies renouvelables touche à sa fin au Sénat, là même où il a commencé. Ce projet de loi se veut une réponse à 3 chiffres que je vous avez exposé. 3 donnée qui souligne la nécessité d'agir trois données qui démontre à quel point notre pays se trouve à un tournant historique. 2 tiers c'est la part d'énergies fossiles dans notre consommation finale d'énergie. Deux tiers de gaz de fioul, de carburants dont nous ne pouvons aujourd'hui pas nous passer pour notre industrie pour nous déplacer et pour nous se chauffer. Deux tiers d'énergies fossiles importés au détriment de notre balance commerciale comme de notre souveraineté. 2035 c'est la date à laquelle, 26 de nos 56 réacteurs nucléaires arriveront au terme de 50 années d'exploitation. Tous devront alors passer le cap d'un contrôle de sûreté approfondie pour être. 10 années de plus. Vous le savez en matière énergétique, 2035 c'est demain. 60%. C'est selon RTE, la proportion d'électricité que nous devons produire en plus à l'horizon 2050 pour répondre à nos besoins croissants d'électrification pour l'industrie, les transports et les bâtiments. Si nous voulons devenir le 1er pays industriel au monde à sortir des énergies fossiles et atteindre la neutralité carbone. Si nous voulons devenir enfin maître de notre destin énergétique, nous ne pourrons nous passer d'aucune énergies décarbonnées qu'elle soit nucléaire ou renouvelable tant la marche à franchir et autres. Nous devons accélérer. Accélérer, car nous sommes le pays européen qui n'a pas atteint ses objectifs de déploiement des énergies renouvelables. Car face aux règles dérèglement climatique. Tous les scientifiques nous le disent nos prochains objectifs seront encore plus ambitieux. Voici l'enjeu de ce texte lever tous les verrous qui retardent le déploiement des projets d'énergies renouvelables, ni plus ni moins. Il ne s'agit ni d'allouer des moyens financiers déjà prévu dans le projet de loi de finances, ni d'anticiper la future programmation sur l'énergie et le climat qui, nous le savons mathématiquement conduira plus de production d'énergie renouvelable. Pour répondre à cette ambition d'accélération. J'avais pris un engagement devant vous, celui de co-construire ce texte de le construire avec tous ceux qui veulent agir pour le pouvoir d'achat des Français et la compétitivité de nos entreprises. Tous ceux qui souhaitent défendre l'indépendance industrielle énergétique et donc politique de notre pays. Tous ceux enfin qui veulent lutter contre le réchauffement climatique. Cette méthode inédite a défini les grands équilibres de ce texte construit ces grands apports de manière consensuelle, il conduit à sa large adoption au sein de votre chambre. Je tiens à souligner la qualité des échanges et du travail conduit par les rapporteurs Didier Mandelli et Patrick Chauvet et par les présidents de commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Et de la présidente des affaires de la commission des affaires économiques. Jean-François Longeot et Sophie Primas. Je souhaite également remercier l'ensemble des responsables de textes dans chaque groupe avec qui j'ai eu des échanges continue nourri et c'est normal. Exigeant. Permettez-moi maintenant de prendre quelques instants pour souligner les avancées majeures qui ont permis nos débats. Sur la planification d'abord c'était une demande des territoires porté par le Sénat pour la première fois nous créons un système de planification qui met les élus locaux au centre du jeu qui leur fait confiance. La commission mixte paritaire a permis de préciser le dispositif en simplifiant le système et en conférant aux comités régionaux de l'énergie, un rôle de vigie sur les zones d'accélération et d'exclusion au regard des futurs objectifs de la programmation pluriannuelle régionalisée et je le rappelle, pas de zones d'accélération. Pas de zone d'exclusion. C'est un levier offert aux élus pour aménager leur territoire en décidant des zones où ils vont en priorité développer des projets d'énergies renouvelables. Les élus locaux proposent et ont le dernier mot sur le zonage aucune commune ne pourra se faire imposer une zone d'accélération sur son territoire mais la somme de ces zones doit permettre d'être à la hauteur des ambitions de la production de la production de la programmation pluriannuelle de l'énergie. 2ème. Sujet l'agrivoltaïsme. C'est une mesure issue d'une proposition de loi largement adoptés par le Sénat. Je tiens à saluer l'auteur Jean-Pierre de colle et le rapporteur Franck mine en ville mais aussi Jean-François Longeot Jean-Pierre Moga et l'ensemble des sénateurs qui ont travaillé sur ce sujet de nombreux mois. Notre objectif, je les maintes fois répété et de concilier souveraineté alimentaire et souveraineté énergétique. Il y avait que le texte que vous votez. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire que nous sommes à la hauteur de l'enjeu pour la première fois, nous donnons en droit une définition de l'agrivoltaïsme avec des conditions. Un encadrement qui garantissent la compatibilité des activités agricoles avec les activités énergétiques et le bénéfice des activités énergétiques pour les activités agricoles. Le texte vient également encadrer l'installation de panneaux faut écoutez vos voltaïque sur sols agricoles afin qu'aucune terre fertile ne soit sacrifiée et qu'aucune forêt ne soit inutilement défricher. En effet, c'est le 3ème. Sujet, nous favorisons l'accélération des énergies renouvelables dans les zones déjà artificialisées en matière d'énergies renouvelables et bâtiments constitue une priorité de mesures importantes avaient déjà été prises dans la loi climat résilience nous avons rehaussé les objectifs de développement de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments neufs et lourdement rénovée. Surtout, la commission mixte paritaire, à renforcer l'ambition du texte sur les bâtiments existants. Elle a introduit en effet une obligation de couverture des bâtiments non résidentiels ayant une emprise au sol au moins égale à 500 m2, soit d'un procédé de production d'énergie renouvelables, soit d'un système de végétalisation. Je salue cette avancée, qui était attendu par plusieurs groupes. Par ailleurs, nous avons également apporter des facilités pour implanter des projets d'énergies renouvelables sur tous les délaissés routiers, ferroviaires, fluviaux. C'est une avancée massive et inédite. Nous avons enfin retenu un seuil obligatoire pour l'installation d'ombrières sur Parking de 1500 m2, ce qui va considérablement augmenter le nombre de parkings ayant l'obligation d'installer des ombrière ces avancées. Elle n'était pas écrite, c'est grâce à vos propositions et à nos échanges que nous avons augmenté notre ambition. Autre sujet, celui du partage de la valeur, c'est un à mort un apport majeur de ce texte. Il doit permettre les que les habitants des communes tire directement partie des retombées des projets d'énergies renouvelables et qu'il soit associé associé à leur réussite et je remercie la présidente Sophie Primas et le rapporteur Patrick Chauvet qui ont pas. Particulièrement travaillé sur ce sujet. La création d'un fonds de financement d'actions locales pour les collectivités d'un second Didier à la biodiversité et si j'ose au Et l'ouverture d'un financement participatif des habitants au projet sur leur territoire sont des apports positifs que nous soutenons. Et car nous avons entendu certaines craintes. Nous avons complété ce dispositif en permettant aux collectivités locales de soutenir directement leurs habitants et notamment les ménages en précarité énergétique. Enfin je me réjouis que ce texte facilite le développement des énergies renouvelables dans les territoires d'outre-mer ce texte n'aurait pas été complet sans ces dispositions les énergies renouvelables étant stratégique pour l'autonomie énergétique de ces territoires qui sont mal interconnectés. Et alors que beaucoup connaissent des difficultés et des dépendances à des Je tiens à remercier les députés des Outre-mer et les sénateurs et plus largement des zones non interconnectées pour le travail collectif mené sur ces sujets. Les dames et messieurs les sénateurs, nous avons démontré que les chemins pour bâtir des compromis au service de notre pays existe. Il s'agit maintenant de les emprunter de les emprunter pour agir et lutter contre le dérèglement climatique pour construire notre indépendance énergétique pour protéger le pouvoir d'achat des Françaises et des Français et pour défendre la compétitivité de nos entreprises. Je vous remercie. Merci madame la ministre. Alors je rappelle qu'en application de l'article 42 alinéa 12 du règlement, le Sénat, examinant après l'Assemblée nationale, le texte élaboré par la commission mixte paritaire. Il se prononce par un seul vote sur l'ensemble de ce texte en ne retenant que les amendements présentés ou accepté par le gouvernement. En conséquence, le vote sur les amendements et sur les articles est réservée. Nous passons donc à la présentation des amendements du gouvernement avant d'en venir aux explications de vote, des groupes. Madame la ministre a hein si vous voulez bien. Accepter de présenter l'ensemble de. Voilà mais vos amendements merci beaucoup. Ce sont des des amendements rédactionnels ou de coordination comme il arrive souvent dans ce type de texte qui vont préciser des références juridiques changer hein ici un mot là. Assurer la bonne référence donc 18 amendements mais qui apporte surtout une renforcement de la la tenue juridique de ce texte. Merci beaucoup. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Bonsoir. Écoutez c'est madame la présidente, c'est un avis favorable sur chacun de ces amendements qui ont été vus ce matin en commission, il s'agit effectivement d'amendements rédactionnels après pour, pour l'essentiel après passage en CMP. Merci beaucoup. Alors nous allons passer donc aux explications de vote, des groupes. À raison d'un orateur

Mais vous allez avoir 5 minutes donc. Nous allons passer donc aux explications de vote, des groupes à raison d'un orateur par groupe. Et la parole est à madame Nadège avez pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants pour cinq minutes. Madame la ministre, monsieur le rapporteur. Monsieur le président de la commission. Mes chers collègues. Vous avez posé le cadre Madame la Ministre de tiers c'est la part des énergies fossiles dans notre consommation initiale finale d'énergie deux tiers importé en même temps, la proportion d'électricité que nous devons produire en plus à l'horizon 2050 est estimée à 60%. Disons-le, le défi à relever est immense pour à la fois respecter nos engagements environnementaux et préserver notre souveraineté. Il y a 2 semaines le baromètre Observer mettait en avant notre retard sur l'éolien, le solaire ou encore la géothermie au regard des objectifs de la PPE, la conjecture elle conjoncture économique mondiale mais aussi par la complexité de notre réglementation. Il s'agit donc bien pour nous de soutenir plus fortement la production d'énergies décarbonnées en France, qu'elle soit nucléaire ou renouvelable. Il s'agit d'aller plus vite et c'est ce que nous faisons. Il y a deux semaines toujours réunis pendant près de 5h en commission mixte paritaire avec nos collègues députés nous parvenions à un compromis sur le sujet de la loi, relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Les conclusions que nous examinons aujourd'hui sont le fruit d'un travail parlementaire de plusieurs mois d'une construction transpartisane alors que nous nous apprêtons à les adopter. Je veux saluer une nouvelle fois votre travail messieurs et Madame les rapporteurs et votre écoute votre méthode de coconstruction Madame la Ministre est également remercier toutes les équipes qui ont travaillé à la rédaction. Afin d'accélérer nos actions non dans ce texte. Tous les leviers disponibles en agissant sur la simplification des procédures, je l'ai fait OK précédemment en libérant du foncier et en partageant la valeur productive Les discussions au cours de la CMP auront beaucoup porté sur la planification territoriale du déploiement des énergies renouvelables et nous avons abouti des zones d'accélération non exclusive pourront être identifiés et le conseil municipal gardera un rôle clé sur l'agrivoltaïsme ensuite intégré au Sénat en première lecture une définition est désormais apporter un encadrement et fixé un nouvel outil au service des agricultures sont que la production d'électricité viennent concurrencer la production alimentaire avec des précisions aussi sur la comptable la compatibilité entre l'agrivoltaïsme et les aides de la politique agricole à plusieurs en droit du texte nouveau nom favoriser l'accélération des énergies renouvelables dans les zones déjà artificialisées, de même que sur les délaissés routiers et ferroviaires. Nous intégrons également dans la loi un seuil obligatoire pour l'installation d'ombrières sur les parkings de 1500 m2. Le partage de la valeur figure aussi parmi les apports majeurs de ce texte, la création d'une contribution territoriale permettra notamment de financer les projets des communes et de leurs groupements en faveur de la transition énergétique, telles que la rénovation énergétique et les les fichiers. Cacité et la mobilité propre je me fais Icitte également des avancées sur l'éolien pourra rude sur et un raccordement effectifs des éoliennes en mer. La CMP a autorisé l'implantation d'ouvrages de transport d'électricité par des goures rogations à la loi littoral. Le Sénat a été là encore entendu dans sa volonté de mieux associer les élus locaux à cette dérogation. De même qu'il a été suivi pour ce qui concerne la généralisation du dispositif de planification spécifique au projet éolien en mer à l'ensemble des façades maritimes. Enfin, concernant le rôle des ABF une voie médiane a là encore été emprunté. Il est, il est désormais prévu dans la loi que les ABF non plus une seule mission la protection du Patrimoine mais aussi la transition énergétique. Une circulaire viendra préciser cela et nous y serons attentifs. Je crois par conséquent que les équilibres ont été respectées par le projet de loi les sénateurs de mon groupe RDPI le voteront évidemment et avec ce texte, qui aura bientôt force de loi. La France fera mieux longeant premier je le rappelle, est celui de la défense de notre souveraineté et de notre indépendance future. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Hervé Gillé pour le groupe socialiste, écologiste et républicain également pour cinq minutes. Merci madame la présidente, madame la ministre. Les sénateurs du groupe socialiste, écologique et républicain s'engage depuis plusieurs années sur l'urgence à passer d'une écologie de principe à une écologie d'action. Avec ce texte nous touchons du bout du doigt. Notre objectif est une majorité arrive enfin une volonté commune. L'accélération du déploiement des énergies renouvelables. Ceci étant, nous continuons à nous interroger sur le calendrier de programmations des projets accélération des énergies renouvelables et nucléaire pour finir sur une loi de programmation énergie-climat qui cristallisera le choix de notre mix énergétique. Bref, nous mettons la charrue avant les boeufs, pour autant c'est parce que la France a été le seul pays de l'Union européenne à avoir manqué son objectif de production des énergies renouvelables en 2020 que le groupe socialiste a agi en responsabilité. Pour améliorer autant que possible ce texte nécessaire afin de trouver une issue favorable. Il conserve son objectif initial d'accélération des énergies renouvelables, tout en tenant compte du rôle central des collectivités territoriales et de la nécessaire préservation de la biodiversité. En effet plusieurs améliorations sont notables. Premièrement la CMP revenu sur la rédaction de l'article 4 en réintroduisant le fait que les projets d'ENR qui pourront bénéficier de manière automatique de la raison impérative d'intérêt public majeur devront répondre à des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ce que nous considérons comme une mesure de protection. Deuxièmement, elle supprime la modification de la répartition de la taxe sur l'éolien en mer entre les communes, sur la base de la population dite DGF c'est-à-dire en majorant la population d'un habitant par résidence secondaire. C'était quand même assez assez déstabilisant par après avoir certaines communes du littoral. Concernant l'accélération du développement de l'énergie solaire thermique et photovoltaïque depuis le début de l'examen de ce texte. Notre groupe a privilégié le développement d'énergies solaire sur le bâti existant plutôt qu'une augmentation de l'artificialisation le texte va au-delà de ce qui était initialement proposé par le projet de loi initial, c'est donc un grand pas. Nous avons défendu un encadrement des nouvelles dérogations la loi littoral et à la loi montagne pour éviter une accentuation du mitage des territoires, avec un risque accru de Roger par les habitants des projets sur ces espaces protégés. Aussi, le compromis trouvé en CMP qui permet de recueillir l'avis des associations représentatives des collectivités territoriales concernées, à savoir la neige ou la ANEM et donc satisfaisant. Nous avons été très attentifs. Madame la ministre et prenons maintenant acte du processus de planification partant des communes qui a été entérinée. Ils se concrétise par la définition de zones d'accélération pour l'implantation d'énergies renouvelables. que les communes ne pourront définir des zones d'exclusion des énergies renouvelables qu'une fois les zones d'accélération elles-mêmes défini et qu'elle soit suffisamment nombreuses, pour que les objectifs de la PPE puisse être atteint une mesure de bon sens qui évitera des vetos arbitraire qui était d'ailleurs rejeté par les associations d'élus locaux. Néanmoins, le processus de planification n'est pas suffisamment aboutis certes les Scott les PLU ils seront consultés mais l'approche territoriale permettrait une meilleure acceptabilité des mix énergétique et meilleure répartition de la valeur. Nous restons dans nous restons dans un entre-deux politique plus que que Un débat s'est instauré concernant l'avis conforme ou à vie simple des architectes des Bâtiments de France. Le consensus trouvé en CMP illustre surtout le manque de moyens alloués aux services pour accompagner au mieux l'implantation des projets en fonction de la réalité de terrain. D'autres points du texte final sont plus contrastées sur la grille vos tabagisme, nous avons été constants pour défendre la nature première du foncier agricole la production alimentaire. Notre devoir étant de protéger les agriculteurs et lutter contre les effets d'aubaine visant à transformer notre modèle agricole en de vastes champs de panneaux photovoltaïques. La plupart des arbitrages se décideront par décret et nous serons attentifs à suivre leur mise en oeuvre. Néanmoins, la recherche d'un modèle économique et en mental agricole mérite d'être retravaillé. Pour terminer nous déplorons la suppression de la disposition introduite par l'Assemblée nationale qui permettait d'interdire aux producteurs de suspendre à leur initiative leur contrat de compléments de rémunération, avant leur terme pour profiter seul au détriment de la collectivité de l'envolée des prix de l'énergie et donc des surplus de revenus engrangés ce processus rend l'État systématiquement perdant en le privant de recettes finalement à l'issue de nos débats, ce texte va néanmoins dans le bon sens même si des éditeurs que des interrogations demeurent à la fois dans la mise en oeuvre des mesures mais également dans les arbitrages qui seront décidées par décret. Il est néanmoins encore insuffisant voire trop complexe sur le plan de la planification territoriale, l'accélération des énergies renouvelables ne pourra se faire que dans le cas de projets de territoire cohérent permettant une répartition de la valeur équilibre Max les permettant à chacun de prendre sa femme objectif fixé Ouais j'ai demandé de respecter parce qu'il y a, on a encore un débat derrière. Donc si vous pouviez respecter votre temps de parole, ce serait formidable. Et maintenant nous allons monsieur Fabien Gay pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour cinq minutes.

Madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues. Après les énergies renouvelables. Début novembre, l'énergie nucléaire. Début janvier, nous discutons à nouveau suite à la commission mixte paritaire des énergies renouvelables. Le groupe communiste défend et nous l'avons dit un mix énergétique équilibré avec une part de nucléaire et une part d'énergie renouvelable. Mais nous voulons répétons il y a un problème de méthode et d'ailleurs une commission mixte paritaire avait 18 amendement en séance, pardonnez-moi, j'ai rarement vu ça, et il y a pas que des amendements de coordination j'invite chacune et chacun à lire l'amendement le 16 avant de se prononcer sur le vote. Il aurait d'ailleurs fallu privilégier une discussion d'ensemble pour que nous puissions justement de traiter de cette question du mix énergétique dans son ensemble. Preuve que tout cela est fait dans le désordre. Nous allons au bout d'un long chemin législatif discuter de plus en plus ouais annuel pour la politique énergétique qui arrivera cet été. Cette segmentation des débats à au moins une cohérence d'ensemble Madame la Ministre dans nos comme qu'en aucun cas vous n'agissez pour que l'énergie sorte d'une logique de marché, ni pour qu'elles soient vendues à des tarifs accessibles à toutes et tous, nous voyons bien ou sous la nous mène l'électricité, le gaz. Augmenter de 15% au 1er février et les tarifs réglementés du. Disparaîtront en juin prochain. D'ailleurs toujours pas un mot sur cette extinction. Madame la Ministre. En pleine crise énergétique. Êtes-vous prête. Pour livrer aux appétits financiers les 5 millions de foyers qui dépendent des tarifs réglementés du gaz, un jour il faudra nous donner votre position. Pire. Je ne sais pas si cette loi permettra l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Mais elle accélère a sans doute la libéralisation du marché de l'énergie à travers l'utilisation des pépés Haye comme on dit, ou encore le partage de la valeur qui vont se généraliser dans de nombreuses communes et intercommunalités. Tout cela est en opposition totale avec le service public de l'énergie que nous défendons. Ensuite, pas un mot sur qui développera ces énergies renouvelables. Le public ou le privé et puis si nous voulons accélérer encore faut-il des travailleuses et travailleurs formés des filières de formation et des filières industrielles pour construire, entretenir et démanteler les panneaux photovoltaïques et les pales des éoliennes concevez-vous cette accélération comme une énième dépendance face aux entreprises chinoises et à leur savoir-faire là encore, pas un mot. Alors je note et nous notons qu'il y a quelques avancées, nous voulons les souligner. Vous avez entendu le besoin d'associer les communes dans la définition des zones prioritaires est propice à l'installation de sites de production d'énergie renouvelable. Par ailleurs, plusieurs surfaces déjà artificialisées comme les parkings permettront la création de milliers de mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Ce sera aussi sur le toit des bâtiments non résidentiels et au total on peut supposer que nous doublerons notre capacité de production d'ici 10 ans. Toutes ces dispositions se feront pourtant au prix d'un contournement du code de l'urbanisme, du code de l'environnement est en contradiction avec les démarches de concertation promu dans tous les projets urbains que nous connaissons dans nos communes. Sous prétexte de rattraper un retard accumulé depuis des années, vous faites une croix sur des dispositions essentielles protectrice et utile. C'est notamment contre ces régressions que nous nous sommes mobilisés avec les collègues lors des débats en séance. Il est paradoxal de promouvoir des énergies dites renouvelables, censé être plus respectueuse de l'environnement en les accents au détriment des espaces naturels forestier littoraux. Le fait de limiter le dialogue et les recours possibles autour de ces projets n'offrira plus des possibilités suffisantes pour tenir un débat public utile et serait nous craignons si quand vous leur donniez quelques mois au détriment de l'accord certes station vous perdiez finalement plusieurs années avec des oppositions cristallisé enfin il y a un enjeu global, l'urgence climatique et l'absence de réponse pour laquelle la France est régulièrement condamnée ne se résoudra pas seulement par l'accroissement de la production d'énergies renouvelables. Il faudra aussi passer par la réduction de la consommation d'énergies fossiles que ce projet de loi ne nous a pas permis d'aborder, c'est pourtant une aspiration majeure de notre groupe qui doit passer par la lutte contre les passoires thermiques. La promotion du transport ferroviaire des mobilités douces ou encore l'accompagnement de notre agriculture. Ces considérations sont pourtant absents du texte, tout comme l'avait question d'une maîtrise publique de l'énergie en filigrane ce qu'il faut comprendre c'est plutôt que vous souhaitez accélérer la libération du secteur à l'heure où toute la crise que nous vivons nous prouve qu'elle un échec cuisant. C'est pour toutes ces raisons que nous nous abstiendrons. Merci cher collègue. Parfait. Je vais donner la parole au président Jean-François Longeot pour le groupe Union centriste pour cinq minutes. Madame la présidente, madame la ministre, nous retrouvons aujourd'hui pour examiner le fruit de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 24 janvier dernier sur le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Près de 3 mois après le début de son examen. Je me félicite qu'un accord était trouvé entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur ce texte, texte indispensable à la préservation de notre souveraineté énergétique et à l'atteinte de nos objectifs climatiques. Vous le savez, la France fait figure ne mauvaise élève dans le déploiement des énergies renouvelables, elle est le seul pays de l'Union européenne ne pas avoir atteint l'objectif qui lui était fixé à l'horizon 2020. Notre responsabilité était donc de taille dans l'examen de ce projet de loi notre commission s'est félicité du dépôt de ce projet de loi qui constitue le 1er texte intégralement consacré au développement des énergies renouvelables dans notre pays. Néanmoins, comme Didier Montlhéry et moi-même l'avons exprimée de concert lors de l'examen en première lecture sa version initiale nous a laissés sur notre faim. Outre les oublis, notamment s'agissant du gaz et de la chaleur renouvelable, nous avions en particulier déploré de lacunes. Un manque d'ambition simplificatrice, d'une part et le manque d'outils destinés à favoriser la Corsair stations locales. D'autre part. Nous avons donc aborder l'examen de ce projet de loi avec une ambition claire celle d'accélérer plus substantiellement la réalisation des projets. D'une part en instituant une démarche de planification territoriale afin de favoriser une meilleure approbation locale et d'autre part, en simplifiant plus amplement les procédures administratives applicables à ces projets. L'Assemblée nationale, a poursuivi le travail engagé par le Sénat en confirmant, nombre de nos âges joue comme la création d'un fonds garanti à compenser une partie des pertes financières subies par le porteur d'un projet d'énergie renouvelable qui résulterait d'une annulation, par le juge administratif d'une autorisation administrative. Et l'institution d'un référent préfectoral pour faciliter l'instruction des demandes d'autorisation et l'accompagnement des porteurs de projets pour n'en citer que de. Bien entendu, des divergences de vue se sont néanmoins en fait jour entre nos chambres elles ont donné lieu à de riches échanges échanges entre les rapporteurs de l'Assemblée nationale et ceux du Sénat en amont de la réunion de la commission mixte paritaire. Ce dialogue. Constructif a permis de trouver un accord ou une rédaction de compromis sur l'ensemble des dispositions restant en discussion je tiens à ce titre, a salué l'engagement important et le travail effectué par Didier Mandelli. Je remercie également nos collègues de la commission des affaires économiques pour leur contribution à ces travaux. Patrick Chauvet et Sophie Primas. L'esprit de coconstruction qui nous a animés. À n'en point douter, contribuer à l'issue positive de cette CMP. En définitive, le projet de loi qui nous est soumis est un texte de progrès par rapport au texte initial qui conforte de très nombreux apports ces sénatoriaux j'en citerai quelques-uns à l'article 1er la pénurie, la pérennisation de plusieurs mesures de simplification administrative et visant à accélérer l'instruction des projets d'ENR. À l'article 3, le dispositif de planification territoriale ascendante voulue par le Sénat a été confirmée en CMP et les travaux de la CMP ont permis de donner plus de corps aux zones d'accélération pour les énergies renouvelables qui seront identifiés localement en y prévoyant des mesures de simplification procédurale spécifique par exemple l'encadrement d'un délai de 3 mois de la phase d'examen des autorisations environnementales. L'article 5 visant à limiter les risques contentieux portant sur des projets de production d'énergie renouvelable a été rétablie dans une rédaction rédaction proche de celle du Sénat vous article 11 bis et austère introduit par notre assemblée. Un compromis a été trouvé sur la solarisation des bâtiments dont résidentiels existants et 9 qui permettra de développer des installations solaires en toiture. Enfin ce texte a permis d'avancer sur l'agrivoltaïsme ce donc je me réjouis tout particulièrement était à l'ayant été à l'origine avec mon excellent collègue et ami Jean-Pierre Moga, de la réflexion sur ce sujet dans notre assemblée. Tout compromis à un prix et certains de nos joue non pas passé le cap de cette navette parlementaire. Je pense par exemple à l'attribution au Conseil d'État de la compétence pour statuer en premier et en dernier ressort sur les litiges concernant les projets d'installations de Gaz renouvelables ces bémols sont toutefois marginaux au regard des nombreuses dispositions plus structurante qui ont été confirmées aussi je ne pense pas faire erreur en disant que l'équilibre final auquel nous sommes parvenus fait largement au travail. Honneur à notre travail sénatorial. Il me reste donc à vous remercier pour le travail accompli et à vous donner. Rendez-vous pour la loi de programmation quinquennale que nous aurons à examiner courant 2023. Je vous remercie. si la parole est à monsieur Jean-Pierre Corbisez. Pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour cinq minutes également. Si. On ne est pas. Madame la présidente, madame la ministre. Monsieur le rapporteur. Chez Didier madame la présidente de la Commission, monsieur le président. Chers collègues, 7 titres. d'une centaine d'articles, plus de 100 pages. Heureusement qu'il s'agissait de simplifier et d'accélérer. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui au sortir de la CMP particulièrement dense, dense, mais heureusement le manque d'ambition que j'avais regretté en discussion générale a été en partie comblé. Cependant Madame même liste pour remplir vos objectifs que vous vous êtes fixés ne voudra des textes supplémentaires dont on sait qu'ils mettent parfois beaucoup de temps à être publié, sans parler de la validation de certaines cartographie régionale et surtout les moyens budgétaires mobilisés devront être considérable. Si l'on veut donner un minimum de Cora ce texte. Ça lui ont néanmoins d'entrée de jeu l'instauration des zones d'accélération disposition absent du texte initial et que le travail parlementaire, à l'initiative du Sénat aura permis d'introduire. Preuve s'il en était de l'impérieuse nécessité de laisser aux députés et sénateurs, le temps d'exercer leur mission de législateur est d'encourager leur force de propositions. Mais un peu de temps une seconde lecture n'aurait pas été de refus, le Sénat n'a pas eu ce n'a pu se prononcer sur le nombreux articles introduits par l'Assemblée nationale. Ces zones d'accélération permettront, nous l'espérons une réelle planification et un rééquilibrage du déploiement des parcs éoliens et solaires et remplaceront les territoires au centre de la décision. Consultations concertations. Avis conforme 3 procédures qui redonnons aux élus leur rôle légitime de maîtrise de leur emprise territoriale tout en jouant la carte de la solidarité entre collectivités. La possibilité d'introduire au sein des PLU ou des Scott pour les communes soumises au règlement d'urbanisme. La définition de zones d'exclusion pour l'implantation des ENR conforte elle aussi le principe que les élus locaux sont bien les mieux placés pour organiser surtout validé les aménagements, les plus pertinents pour leur territoire. Je sais que certains représentants de l'industrie des ENR il voit une complexification du processus, il y a un risque de retard mais s'agissant de la transformation de nos collectivités. La concertation avec les élus et au-delà avec les habitants ne peut pas être sacrifié. C'est le contraire à gage de réussite. A-t-il personnelle parce que j'y suis attaché, que je crois dans cette énergie nouvelle. Je me félicite de l'intégration des installations d'hydrogène renouvelable et bas carbone dans le corps du texte. Il en va de même pour l'équilibre retrouvé dans plusieurs articles entre la volonté d'accélérer le déploiement des arts du renouvelable et celle de préserver notre biodiversité comme nos paysages. Pertinente également l'introduction de l'obligation pour les entreprises de plus de 250 salariés d'élaborer un plan de valorisation du foncier en vue de produire des ENR. Au regard des enjeux notre conversion énergétique, il est juste que tout s'qui contribue, y compris les entreprises. Toujours à titre personnel, je regrette que n'ait pas été retenu la proposition d'alléger les procédures d'avis des ABF pour faciliter l'implantation en ville des panneaux solaires, quand bien même il serait à proximité de sites classés Madame la Ministre panneau noir sur toi tu noir il y a désormais plus d'espoir. Plutôt que systématique et dans un périmètre classé le choix aurait pu être plus pragmatique. La toiture en question était réellement visible depuis le site classé. Sur le fond du texte et même s'il mentionne désormais des ENR qui en était absente. Il vote toujours pas assez loin sur la globalité de l'action à mener pour créer un véritable écosystème de la conversion bas-carbone depuis la formation jusqu'à la mise en place d'une véritable filière industrielle en passant par la transformation de notre économie basée encore trop massivement sur les énergies fossiles. Au final, nous sommes devant un texte qui était loin qui est loin de faire l'unanimité. Les professionnels du secteur des ENR le qualifient pour certains d'néfaste quand d'autres y voient si nous une accélération du moins signe et défenseurs de l'environnement le conteste pour les risques qui l'emporte pour nos paysages et la préservation de la biodiversité. Les associations d'habitants ne sont absolument pas convaincu, notamment celles mobilisées contre l'éolien marin. Seuls les élus locaux semblent rassurés puisque confortés dans leurs responsabilités, ce qui nous en conviendront réjouit les sénateurs que nous sommes cependant Madame la Ministre le verre étant plus qu'à moitié rempli là ce texte sera majoritairement voté par notre. Au groupe, je vous remercie. Si cher collègue, la parole est à madame la présidente, Sophie Primas. Pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes.

d'abord de consolider, de renouveler le parc nucléaire mais également de développer de façon extrêmement volontaire. La production des énergies renouvelables, la France faible d'une décennie d'atermoiements est aujourd'hui à la traîne à la fois dans le nucléaire, mais aussi dans les énergies renouvelables. L'objectif d'accélération qui sous-tend ce projet de loi et donc partagé car essentiels à notre souveraineté une fois de plus et ses moins regretté que nous soyons obligés de légiférer dans le désordre. Car oui, bien sûr, il aurait fallu commencer par la loi de programmation sur l'énergie. Mais plus encore nous légiférons trop à l'aveugle, puisque seulement 15% des 112 articles ont fait l'objet d'une étude d'impact. Enfin et pour en finir avec les regrets. Nous n'avons pas toujours les Ferré sur les véritables enjeux. Le texte initial était muet sur l'énergie hydraulique, il était muet sur les collectivités territoriales qui consacrent pourtant 5 milliards et demi d'euros à la transition énergétique. Le Sénat a corrigé le Tir et nous avons infléchie et enrichi le texte en premier lieu, ça a été dit plusieurs fois, nous avons associé les collectivités en respectant leurs compétences, leurs finances et en privilégiant une approche décentralisée en matière de planification, il faut bien avoir à l'esprit que nous avons garanti aux communes la maîtrise de la définition des zones d'accélération et de la réglementation urbanistique qui en découle. Nous avons permis à l'ensemble des communes de recourir au dispositif dis 3DS elle pourra ainsi réglementer l'implantation des types d'énergies renouvelables de toutes les énergies renouvelables et même les exclure sous conditions la vie des communes sera enfin requis requis en cas d'implantation de ces énergies en zone littorale. Alors oui, mes chers collègues, la planification demandera aux élus de plancher de nouveau sur leur document d'urbanisme, ce qui est complexe et souvent coûteux mais nous avons voulu donner la main aux élus plutôt que de se laisser imposer des schémas par notre cher État profond aujourd'hui rien ne protège les maires de l'installation controversée et parfois flibustières par exemple d'éoliennes demain après avoir travaillé et réfléchi sur les documents de planifications, ce sont les maires leur population et leurs conseils qui décideront. Dans le même esprit, nous avons appliqué une contribution territoriale au partage de la valeur à tous les projets d'énergies renouvelables électriques comme gazier lauréats d'un appel d'offres. Cette contribution sera allouée majoritairement aux collectivités. Nous avons également au Sénat assurer aux collectivités l'accès à plusieurs dispositifs les contrats d'achat de long terme qui leur permettront de mieux se prémunir contre les aléas des prix les prises de participation qui seront proposées aux communes et aux groupements d'implantation des projets d'énergies renouvelables. Les opérations d'autoconsommation qui seront facilités pour l'électricité renouvelable est institué pour le biogaz. L'objectif de notre groupe a été de faire en sorte que les collectivités s'approprie la transition énergétique et dispose des moyens de le faire. En second lieu nous avons garantit la neutralité technologique entre les différentes énergies et les différents équipements. C'est pourquoi nous avons fait adopter des incitations pour 3 secteurs l'hydroélectricité le biogaz et l'hydrogène. En 3ème lieu, nous avons permis l'accélération des projets par la simplification des normes par le financement des actions et la résolution des litiges. Enfin, nous avons essayé de combler quelques-uns impensé du texte qui sont aussi ceux en général de la transition énergétique. Le 1er c'est l'emprise foncière de cette transition et nous avons fait en effet prospérer la proposition. Cher Jean-François Longeot. Sur l'agro-voltaïques adopté au Sénat, qui fera l'objet ainsi pour la première fois d'une définition légale d'une planification et et d'une information légale d'appel d'offres dédié et de souplesse urbanistique. Le second a penser c'est bien sûr la dépendance minière de cette transition car les énergies de renouvelables sont de très grosses consommatrices de métaux critiques, pour tenir compte de cette consommation. Nous avons appliqué un bilan carbone à l'ensemble des projets d'électricité, de gaz et d'hydrogène renouvelable soutenue par appel d'offres. Cela n'épuise pas ce sujet qui est un sujet stratégique, mais nous ouvrons le débat, si ce texte laisse des regrets à certains d'entre nous au sein du groupe les républicains notamment sur l'éolien en mer. Nous proposons son adoption car la souveraineté énergétique de notre pays est un enjeu majeur que nous ne saurions balayé du revers de la main, le Sénat a imprimé sa marque en territorialisant les projets en remettant les élus locaux au coeur du projet de au coeur de la stratégie au coeur de cette stratégie nationale dont ils seront les premiers acteurs, je souhaite remercier tous ceux avec qui nous avons travaillé la commission du développement durable, les rapporteurs et le rapporteur Chauvet. Pour la commission des affaires économiques et vous remercier Madame la Ministre du travail en commun réalisé avec vous-même et vos certes. Merci beaucoup, merci, la parole est à monsieur Pierre mais deviennent pour le groupe les indépendants pour cinq minutes. Madame la présidente Madame la Ministre. Mes chers collègues. Après certaines turbulences lors du passage du texte à l'Assemblée nationale. La CMP a finalement produit un texte de raisons. Il nous paraît équilibré malgré le nombres d'articles ajoutés. Et répond ainsi à l'objectif principal fixé gagner du temps. Cependant, et je crois que c'est déterminant. Le vol réglementaire tout aussi essentiel que sont pendant législatif devra permettre rapidité et performances. Je connais votre engagement Madame la Ministre et je salue votre mobilisation ce projet de loi. Dès sa préparation. Je me félicite également du travail fourni par les parlementaires des 2 assemblées les commissions présidente Commission rapporteur malgré quelques incongruités que nous avons pu régler en discutant et des temps. Nos positions ne n'était pas toujours alignés. Mais nous avons largement enrichi le texte. Pour le groupe les indépendants, l'autre des principaux apports et bien sûr celui de l'agrivoltaïsme. Lors de notre niche parlementaire du 20 octobre dernier, nous avons mis ce sujet au débat grâce une proposition de loi qui a été largement adopté et qui a été insérée dans ce texte. Au moment de son examen au Sénat. J'avais déjà pu m'exprimer en pointant la nécessité de donner un cadre parfaitement défini à cette activité. Ainsi l'activité agricole restera l'activité principale la production d'énergie améliorera également notre mix énergétique et fournira revenus supplémentaires aux agriculteurs sans faire obstacle aux aides de la PAC. La précision de la définition de cette activité évitera les dérives que l'absence de règles aurait pu favoriser en ces temps de crise. L'agrivoltaïsme coche toutes les cases du bon sens. Un autre sujet qui me tient à coeur et que je crois satisfaits concerne la place de nos collectivités territoriales et de nos élus locaux dans le déploiement des énergies renouvelables. J'ai plaidé pour trouver un consensus entre un droit de véto excessif des maires et l'exigence de développement rapide et efficace des énergies bas carbone. Leur voix contents. Ils doivent rester des acteurs majeurs de notre transition écologique. Il connaissait parfaitement leur territoire et la pertinence des projets locaux, les associés, et le gage d'une transition réussie. J'ai le même avis sur les documents d'urbanisme et notamment ceux concernant les Scott. Les objectifs de développement équilibré du territoire ont été améliorés afin de prendre en compte les nouvelles installations de production et de transport des énergies renouvelables. Évoqué le transport d'énergie me permet de revenir sur la question du raccordement. C'est un élément absolument indispensable. On peut installer toutes les énergies renouvelables, que l'on veut, si elles ne sont pas raccordés l'effet un restreint, voire quasiment nulle. L'enjeu de l'intégration aux réseaux de transport et de distribution et principalement entre les mains du gouvernement et des gestionnaires de réseau. Enfin. Je salue la possibilité sous certaines conditions que le stockage d'énergie puisse répondre à une raison impérative d'amélioration de l'intermittence de certaines énergies. Je pense particulièrement au au station de transfert d'énergie par pompage. Dans le même domaine. Le procédé power to gas ce qui nous permettra aussi un autre mode de stockage de l'énergie produite. Nous pouvons cependant constater que notre bouquet énergétique de traite absolument compléter par le nucléaire qui fournit une électricité permanente. Madame la Ministre je conclurai mon propos en regardant vers le futur. Il est à la fois renouvelable et nucléaire. Le mois dernier nous avons examiné le projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires. J'évoquais alors le caractère pilotable de l'électricité produite en continu. De plus, le nucléaire. Et reste une filière d'excellence française. Si nous voulons amorcer sereinement ce virage de modification de nos consommations et de décarbonation. Nous avons absolument besoin de fortement augmenter notre potentiel de production de production d'énergie au carbone. Les 2 projets de loi d'accélération ne sont que les prémices de nos discussions sur le futur énergétique de notre pays et ils étaient nécessaires. Vu la situation d'urgence dans laquelle nous a plongé l'invasion de l'Ukraine. Ne compléteront de nos dispositifs lors des lois de programmation énergétique pour travailler très précisément selon futurs besoins et impulser les nouvelles orientations nécessaires. En attendant, le groupe les indépendants votera bien sûr en faveur de ce projet de loi, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Ronan Dantec. Pour le groupe écologiste solidarité et territoires pour cinq minutes.

Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs président et président de commission. Tout avait très bien commencé sur le principe tout d'abord 7 ans après la promulgation de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de Ségolène Royal. L'État et le gouvernement proposé enfin au Parlement. Une loi consacré au développement des énergies renouvelables permettant enfin à la France de tenter de crédibiliser un scénario à horizon 2035 de réduction de la part du nucléaire sous les 50%. Scénario affiché mais jamais encore décliné en politique opérationnel. Tout s'était bien poursuivi et évidemment il reste au Sénat une certaine nostalgie des années Pompidou d'un hexagone centralisé et un peu refermé sur lui-même où nos centrales nucléaires suffisait presque avec les barrages assurer nos besoins électriques et seulement électrique. Comme on pouvait un peu si attends l'offensive a donc bien eu lieu mais a échoué fauché par quelques pales d'éoliennes zoning, il s'est ainsi trouvé au Sénat une majorité claire pour refuser les 2 mesures qui auraient tronçonner les ma dédite éoliennes, le Sénat a ainsi refusé l'éloignement des parcs éoliens en mer à 40 kilomètres des côtes et rejeté l'instauration d'un droit de véto des maires sur les implantations une responsabilité non je le rappelle, il n'était pas demandeur mieux voire parfois à notre plus grande surprise plusieurs amendements importants du groupe écologiste ont été adoptés sur la planification régionale l'alourdissement des pénalités pour défaut d'équipement panneaux photovoltaïques ou la création d'un fonds dédié à la biodiversité. Je tiens d'ailleurs à remercier les 2 rapporteurs pour leur travail globalement et leur avis favorable assez nombreux qui nous ont délivré. C'est donc fort de ses avancées que le groupe écologiste avait très logiquement voté en faveur du texte amendé par le Sénat. Mais depuis les choses se sont un peu assombri. Un certain nombre de mesures, à notre avis importantes ont été modifiés ont purement et simplement disparu du texte lors de son passage à l'Assemblée nationale. Ainsi du niveau de pénalisation très insuffisant en cas de manquement aux obligations d'équiper les parkings en panneaux photovoltaïques. C'est dommage parce que là il y aura évidemment une baisse en terme d'équipements et de production ainsi aussi de l'affaiblissement des mesures sur l'autoconsommation pourtant demandé dans beaucoup de territoires, cette liste n'est pas exhaustive. Sur le fameux article 3 qui marquer la volonté unanime du Sénat de mieux associer les élus locaux l'équilibre final trouver équilibrant zones d'accélération et d'exclusion. Les deux allant de Pair pouvez paraissent six visant votre slogan était d'ailleurs percutant. Il y a quelques minutes. Madame la Ministre mais l'avis conforme des maires sur de, des étapes qui émaillent ce processus risque de le rendre au final plutôt bloquant et ralentissant c'est ce que craignent aujourd'hui de nombreux professionnels du secteur. Il ne s'agit pas pour autant d'ignorer les avancées de ce texte, l'évolution des procédures pour l'éolien en mer va permettent de gagner un temps significatif dans l'instruction des dossiers. L'ouverture des contrats de long terme aux collectivités est importante pour mobiliser l'épargne locale, enfin et nous y étions très attaché, la création d'un fonds pour la biodiversité. Dans le cas d'une loi sur l'énergie constitue en dépit des montants raboter en CMP également une évolution importante en élargissant pour la première fois à l'énergie et non plus seulement à l'eau l'assise des financements pour pour la biodiversité. Madame la Ministre, le gecko Vert de Manas. Vous remercie sincèrement pour votre attention sur ce point. Des plus et des moins, donc et à l'horizon surtout le retour du nucléaire sur lequel le président et le gouvernement multiplie les signaux en parallèle à la discussion de ce projet de loi. Il ne vous a évidemment pas échappé Madame la Ministre que la vie des filières productrices d'énergies renouvelables était quand même au final quant à l'impact de cette loi sur l'agro-Voltalis. Ça a été dit avant moi, ou l'éolien terrestre par exemple. Aussi, dans ce contexte, le vote du groupe écologiste sera lui aussi mesurer, nous nous abstiendrons sur ce texte qui ne suffira pas. C'est une évidence, à ce que la France respecte ses objectifs de développement des énergies renouvelables, telle que fixée par l'Union européenne, je crois. Merci Merci cher collègue. Alors nous allons passer au vote en j'ai été saisi. Une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur le traité là et sur le texte pardon élaboré par la commission mixte paritaire modifié par les amendements du gouvernement. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

plus personne ne demande à voter le scrutin est clos.

Pour permettre. Au ministre de Saint-de s'installer. La séance est suspendue quelques minutes.

La séance est reprise. L'ordre du jour un appel. Le débat sur les conclusions du rapport. Commerce extérieur. L'urgence d'une stratégie publique pour nos entreprises. Je vous rappelle. Que dans ce débat, le gouvernement aura la faculté s'il le juge nécessaire de prendre la parole immédiatement. Après chaque orateur pour une durée de deux minutes et l'orateur disposera alors à son tour du droit de répartis pour une minute. Monsieur le Ministre, vous pourrez donc si vous le souhaitez répondre après chaque orateur, une fois que celui-ci aura retrouvé une place dans l'hémicycle. Et la parole et tout d'abord aux orateurs de la délégation sénatoriale aux entreprises hein qui a demandé ce débat. Et le premier orateur c'est monsieur Vincent Segouin ou non donc de la délégation sénatoriale aux entreprises pour 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes heureux que ce débat sur le commerce extérieur puissent avoir lieu car il nous paraît essentiel de ne pas répéter les erreurs du passé. La plus importante d'entre elles fut le choix de la désindustrialisation pourtant assumé par les gouvernements successifs depuis des décennies. Personne n'a anticipé les conséquences de ce choix désastreux qui est à l'origine déficit abyssal de notre balance commerciale. Pour de nombreux commentateurs, nous avons touché le fond ou plutôt la bis en dépassant la barre des 164 milliards de déficit en 2022. Évidemment les dernières crises ont encore davantage creusé le solde des échanges de biens notamment à la avec la hausse du déficit énergétique. Mais cette dégradation conjoncturelle ne fait que renforcer une tendance structurelle observée depuis 20 ans. La situation est grave parce que nous nous sentons impuissants face à la détérioration conjoncturelle du commerce extérieur de la France. N'ayant plus de réserves pour faire preuve de résilience. Elle est grave car notre 1er partenaire commercial. L'Allemagne peut au contraire résister à la crise actuelle en effet, en 2021, d'afficher un solde positif de 178,4 milliards d'euros, selon Eurostat. Nous n'avons pas su tirer les leçons des choix économiques ayant placé nos deux pays sur des trajectoires diamétralement opposées. Depuis des années 90 en terme de compétitivité et nous sommes aujourd'hui les derniers de l'Union européenne derrière l'Espagne. La Roumanie et même la Grèce. Monsieur le Ministre, nous espérons aujourd'hui que nous partageons le même constat et les mêmes objectifs sur trois points prioritaires le 1er point. La Team France Export né de la stratégie dite de Roubaix de 2018 constitue un indéniable progrès. Mais ne peut à elle seule résoudre le problème du commerce extérieur de la France car nous ne pouvons pas changer la donne en nous focalisant uniquement sur l'export aujourd'hui l'ensemble des témoignages de notre mission convergent autour d'un constat d'une carence de vision globale stratégique intégrant des objectifs en matière d'importation. 2ème point réfléchir à une stratégie en matière d'importation. Et de relocalisation implique de s'interroger sur 2 éléments, ce que nous sommes en capacité de produire en restant compétitifs et ce qui contribue à notre souveraineté. Les Français ont découvert, conséquences des délocalisations de production avec la pénurie des masques pendant la crise du Covid. Ils vivent aujourd'hui dans l'angoisse de rupture d'approvisionnement de médicaments notamment pédiatriques on recense presse de 320 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur en forte tension. Conséquence des délocalisations massives de production. Nous ne pouvons plus attendre les prochaines crises pour réfléchir relocalisation. Nous devons impérativement nous demandons nous demander aujourd'hui quelles sont les dépendances qui peuvent porter atteinte à notre souveraineté et en tirer les conséquences en matière de relocalisation. Cette stratégie éminemment politique devrait faire l'objet d'une. Loi d'orientation économique pour la France. 3ème point qu'il s'agisse de relocalisation de réindustrialisation verte. Nous ne pouvons plus nous voiler la face. Rien ne sera possible sans accompagner ces projets d'une stratégie fiscale adéquate. La force de frappe, ce sont les outils. Or, elles ne peuvent pas se développer en France, notamment en raison d'une fiscalité de la transmission bien moins favorable qu'en Allemagne. Ça fait des années qu'on le répète. Résultat, nous ne comptons que 5400, OTI contre 12.500 chez nos voisins. Tous les économistes ont reconnu que le poids de la fiscalité de la complexité administrative avait conduit les entreprises françaises à créer des filiales à l'étranger plutôt que d'exporter. les importations des 46.488 filiale française pèse aujourd'hui sur notre balance commerciale. C'est cette logique cette spirale infernale à laquelle nous devons enfin mettre un terme. Je vous remercie. Alors la parole est à Madame, Florence. Compta au nom de la délégation sénatoriale aux entreprises également pour 4 minutes. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Comme le soulignait mon collègue Vincent Segouin à l'instant nous avons perçu tout au long de nos travaux une défaillance en matière de stratégie publique le commerce extérieur doit être appréhendée comme un écosystème. Et toutes les dimensions de la compétitivité nécessite que l'on se fixe des objectifs ambitieux. C'est vrai en particulier en matière de compétences, elle ne s'improvise pas et sont incontournables pour que les entreprises puissent s'emparer des marchés étrangers. Compétences linguistiques économiques mathématique doivent être renforcés pour accompagner l'Inter dossier réalisation de nos entreprises. Les compétences sont également au coeur de toute stratégie de relocalisation, relocalisation, voire de maintien dans nos territoires des productions qui sont aujourd'hui notre force. Prenons l'exemple du secteur des services dont les exportations ont augmenté de 142% depuis 20 ans pour atteindre un solde excédentaire de 50 milliards d'euros en 2022 soit une hausse de 14 milliards d'euros en un an ces services qui sont intrinsèquement liés aux biens industriels repose aujourd'hui sur des savoir-faire qui avec les nouvelles technologies connaissent un risque non négligeable de. Immigration, cette fuite des talents et donc des activités de services constituerait un revers fatal pour notre pays, s'il advenait malheureusement Nous constatons à la faveur des travaux en cours de la délégation aux entreprises sur les sujets de la formation des compétences que les entreprises sont obligées de s'organiser de créer leurs propres écoles pour pallier les carences de la formation initiale. Comme l'ont démontré de nombreux rapport de France Stratégie de la Banque européenne d'investissement ou d'autres. L'indisponibilité de travailleurs qualifiés, constitue une entrave à l'investissement et à l'émotion. Monsieur le ministre, il est temps que la stratégie publique prenne sérieusement en compte la question des compétences. Pouvez-vous nous indiquer comment vous organisez la coordination des actions avec vos collègues en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. La coordination encore sera également le maître mot pour appréhender les enjeux de l'Union européenne. Nous savons déjà que les sur-transpositions françaises de directives européennes constitue un handicap pour la compétitivité de nos entreprises. Mais sommes-nous réellement conscients des effets des sur-transpositions européennes d'accords internationaux. Ou bien du taux de recours dérisoire aux instruments de défense. Commerciale, les idées, c'est de l'Union européenne par rapport aux États-Unis, lors d'un récent débat sur les conclusions du rapport de la délégation aux entreprises consacré à la RSE. Nous avons souligné les difficultés liées à l'absence de réciprocité énorme applicables aux entreprises implantées en de l'Union européenne donc Monsieur le Ministre, comment la France, sensibilise-t-elle les autres États membres de l'Union aux effets néfastes de l'absence de clauses miroirs je sais que c'est un débat qui a déjà porté mais qui à mon avis méritent vraiment d'avancer. Vous l'aurez compris, l'enjeu du commerce extérieur dépasse largement la politique publique de soutien des entreprises à l'export, ce sujet ne sera appréhendée efficacement que lorsque les objectifs de compétitivité seront déclinés dans toutes. Les politiques publiques et partagée par tous les ministères concernés. Nous espérons que nos travaux trouveront un écho car nous devons rapidement changer de logiciel et définir ensemble les priorités de la France en fixant un cap pour les 20 prochaines années. Je vous remercie. Alors dans la suite du. Débat la parole est à monsieur Thierry Cozic pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour quatre minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. La France subit depuis le début des années 2000 une détérioration continue de sa balance commerciale avec un déficit écrasant évalué à près de 85 milliards d'euros en 2021. Cette situation est particulièrement inquiétante. Elle est d'autant plus que la crise énergétique actuelle est marquée par un grave dysfonctionnement du marché énergétique européen qui s'est traduit par une envolée historique des prix du gaz et d'électricité. Les dernières estimations font état d'un déficit qui pourrait atteindre plus de 150 milliards d'euros. Il est nécessaire de trouver rapidement une solution aux défaillances du marché européen de l'énergie qui plombent aujourd'hui la compétitivité de nos entreprises et grèvent le budget de l'nos service publics de nos collectivités et nos ménages. L'électricité que nous produisons en France et pourtant l'une des plus compétitive en Europe. Alors que la spéculation se déchaînent sur les marchés de gros, nos entreprises et notre tissu industriel. Ne peuvent pas directement profiter de cette compétitivité. Si les prix de l'électricité n'ont de cesse d'augmenter. On pourrait Cooney connaître une nouvelle vague de délocalisations et de désindustrialisation. Alors que dans le même temps, les États-Unis ont lancé un programme protectionniste à travers l'inflation, l'inflation l'Union européenne hésite encore à protéger de manière vigoureuse le peu qui lui reste de son industrie. Sans un grand plan d'aide pour la décarbonation notre économie. L'Union européenne peinera atteint les objectifs qui sont les siens. Cela pourrait la placer à la merci du secteur des nouvelles technologies dominé principalement par les firmes sino-américaine. Cela ne va pas dire pour autant que le repli sur soi et la solution. L'Union européenne doit prendre la mesure des phénomènes de reflux, la mondialisation. Et adopter une approche plus pragmatique et en phase avec les enjeux de la transition est né écologique. Notre dépendance aux importations chinoises ne se cantonne plus aux produits de faible valeur ajoutée, force est de constater que la Chine a désormais investi le marché des produits de la haute technologie. Cette dépendance n'est pas spécifique à la France, elle touche aussi nos partenaires européens et les États-Unis. Lorsque la Chine a commencé à les concurrencer sur des produits de haute technologie. Les États-Unis ont réagi auprès de l'OMC en dénonçant, d'une part, l'utilisation du statut de pays en voie de développement et d'autre part les nombreuses subventions et protection que la Chine déployés pour son tissu industriel. Comme par le passé. Les nations qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu sont celles qui ont réussi à protéger leur économie des règles du libre-échange. C'est se méprendre que de continuer à penser que l'on résoudra le problème du déficit commercial en diminuant le coût du travail. Cette course à la déflation salariale a maintes fois montré son inefficacité. Elle serait d'autant plus inopportune dans un contexte actuel de retour de l'inflation d'origine principalement énergétique. La solution pourrait être ailleurs. Les effets de bord d'un capitalisme devenu incontrôlée ont appauvri les couches populaires, les plus tributaire des secteurs industriels, marchands. Ce faisant, ces délocalisations sapé la confiance collective envers les décideurs publics et privés. Cette confiance est pourtant primordial afin d'engager des nécessaires et colossaux investissements que nous intime d'engager le climat. Monsieur le Ministre, je m'interroge le Pacte Vert européen présenté comme une réponse aux incursions protectionniste. De la Chine et des États-Unis sera-t-il suffisamment conséquent pour remettre sur pied une véritable politique industrielle capable de permettre à l'Union européenne de gagner en autonomie stratégique. Rien n'est moins sûr pourtant, le gouvernement devra trouver rapidement les réponses à cette question tant elle conditionne le retour à l'équilibre de notre commerce extérieur. Merci. Oui, Monsieur le Ministre. Vous attendez juste que notre collègue s'assied. Voilà. Voilà. Merci beaucoup madame la présidente. Mesdames, et messieurs les les sénateurs. Bien sûr je, je partage avec vous le constat. De l'aggravation de notre déficit sur la balance des biens. Qui a plus que doublé par rapport à l'année 2021. Ce doublement étant quasi intégralement du en fait. À la dégradation de la balance énergétique, c'est-à-dire que nous avons sur 2022. Été obligé parce que notre parc nucléaire était en grande partie indisponibles du fait du rattrapage de la maintenance, que nous n'avons pas effectué durant les deux années de Covid et donc au lieu d'exporter de l'électricité, nous avons été obligé d'en importer et nous avons d'autre part subit de plein fouet, comme la plupart d'ailleurs de nos partenaires. La hausse des prix du pétrole et du gaz qui, sur l'ensemble de l'année 2022 ont été multipliés par 2 quand on prend le gaz et même 248% d'augmentation. Donc nous avons cette situation très particulière. Nous sommes confiants sur le fait que elle va se résorber. de manière naturelle puisque le parc nucléaire aujourd'hui à est de nouveau disponible à plus de 75% et il le sera encore davantage dans les prochaines semaines, nous sommes déjà redevenu exportateur d'énergie qui a donc nous exportons de l'électricité, il y a. Ce qui est une bonne, une bonne nouvelle et puis pour le reste, bien sûr, nous sommes en train d'agir au niveau européen pour que les prix du gaz soit capé et que le prix de l'électricité soit recalculé selon une formule qui permette de rendre ces prix acceptable au MWh et donc je suis confiant sur les efforts que nous faisons avec nos partenaires européens pour que l'Europe soit particulièrement compétitive sur les prix de l'énergie, ce qui est évidemment une composante importante de notre balance commerciale. merci, la parole est à madame Marie-Noëlle Lienemann. Pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour cinq minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues rapporteurs. La chute de la balance commerciale de la France est devenue abyssale. Elle se poursuit en dépit de des discours martiaux du président de la République. Qui prétend que la réindustrialisation. Du pays est en marche. ne nous laissons pas égaré par une communication. Qui veut nous bercer de 12 illusion. La réalité que le compte n'y est pas. Et qu'il faut changer de cap. Car les faits sont têtus. La part de la production manufacturière. Dans le PIB. Ne cesse de chuter. Certes, il avait déjà chuté jusqu'à 13,5. En 2019, comme vous le dites, messieurs, mesdames messieurs les rapporteurs. Il n'est plus que de 9%. En 2021. Notre pays est le dernier de l'Union européenne à égalité avec la Grèce. Oui, la principale cause de la dégradation du commerce extérieur. Et la désindustrialisation. S'y ajoute certes désormais la forte dégradation de la balance énergétique. Il y a les hausses du gaz et d'électricité. Mais il y a le fait que la France était redevenue importateur d'électricité alors que jusqu'à présent elle était exportatrice. Qu'on le veuille ou non. C'est la conséquence de choix gouvernementaux calamiteux depuis 10 ans. L'horizon est loin de s'éclaircir. En particulier. Au regard de l'impact inquiétant de la hausse des prix de l'énergie. 42% des entreprises industrielles. Estime qu'ils vont doubler leur prix d'énergie qu'de en 2023. Et que la prévision de ce, il fait, c'est une baisse de 1,5% de la production industrielle du pays. Et les propositions de mesures du gouvernement. Ne sont pas de nature à inverser la donne. Nous considérons qu'il en faut davantage qu'il y a urgence. Comme il y a d'ailleurs urgence de s'exonérer de s'extraire de ces dramatique marché européen de l'énergie totalement absurde et dangereux. Mais le coeur de la acide, c'est quand même la désindustrialisation. Et nous partageons la proposition de des rapporteurs. D'une stratégie globale de long terme. Pour le redressement du commerce extérieur et la réindustrialisation. Mais pour ce faire, faut partir d'un bilan lucide et rigoureux. Et ce bilan c'est l'inefficience. Des politiques développées par Emmanuel Macron est largement soutenu par le MEDEF. On nous disait plus la France pour que la France retrouve sa compétitivité. Il faut baisser le coût du travail. Faut baisser les impôts. Voilà 10 ans que cette politique dite de l'offre. Et mise en oeuvre. 10 ans que la balance commerciale et notre industrie plonge. Ça devrait faire réfléchir. À des remises en cause. Eh bien non. Il y en a jamais assez. persévérer, persévérer. Diabolicos. Car excusez du peu. C'est 150 milliards annuels. D'allégements de cotisations et d'impôts. Pour les entreprises. Sans ciblage. On cible même pas les plus touchées vers le commerce extérieur l'industrie. Sans contrepartie on emplois ou un investissement. Et donc, nous estimons qu'il faut stopper ce gâchis d'argent. Public et réorienter ses crédits vers un soutien ciblé durable dans le cas de plans de filière et d'une véritable politique industrielle. Cette politique doit associer les partenaires sociaux. Les collectivités bien sur les régions mais les autres. L'éducation nationale, l'université, le Centre de recherche et de formation. C'est une mobilisation générale du pays qui s'impose. À une politique nouvelle industriel qui doit s'appuyer à. Sur la création d'un véritable ministère de l'industrie. Indépendant de Bercy. Aveugle avec une administration propre compétente orienté vers cet objectif. Et qui serait l'acteur de cette mobilisation et travaillerait avec le Commissariat général au Plan. Deuxièmement, nous croyons qu'il faut des plans de filière. Bien sûr, dans les domaines stratégiques mais pas seulement. Car la réindustrialisation doit se faire dans la plupart des secteurs de notre pays. Il faut donc évidemment par filière des plans qui gradue le soutient l'effort les aides. Mais ne négligeons aucun secteur. Car c'est bien la diversité du tissu industriel qui permet sa réindustrialisation,

Merci beaucoup madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs. Je partage avec vous un constat. Oui il a pendant plus de 20 ans depuis le début des années 90 jusqu'. Au début des années 2010. Notre pays a fait beaucoup d'efforts, il y avait de grands succès pour se désindustrialiser. Nous avons. Peut être cru. Tous gouvernements confondus d'ailleurs de gauche comme de droite. Au mirage de la Chine en disant ça va coûter moins cher, on sera plus compétitif fidèlement en allant produire ailleurs et et on a été pris par ce merveilleuse effet ciseau qui fait que quand on produit plus chez nous, non seulement on exporte plus nos produits mais on est en plus obligés d'importer ce qu'il nous faut dans notre propre pays et nous avons creusé. De manière constante notre déficit de la balance des biens.

d'un point de vue industriel et nous avons avec les gouvernements du président de la République lancé le plan France 2030 qui est un magnifique outil pour réindustrialiser, notre pays a et j'en veux pour preuve les usines qui aujourd'hui sortent de terre dans les semi-conducteurs près de Grenoble, dans la fabrication de paracétamol de sur les principes actifs avec séquences dans l'Isère ou encore en matière de lithium sur les matières stratégiques, que ce soit dans l'Allier ou dans le Bas-Rhin. Donc oui, la réindustrialisation est en marche. Oui, elle prendra du temps parce que on ne. n'inverse pas 20 ans de désindustrialisation. En 2 ans donc ça prendra une décennie. Mais elle est mise en oeuvre par les gouvernements du président de la République. Merci Madame Lienemann. Il nous faudrait du temps pour démonter le le discours mirobolants sur la réindustrialisation, je ne nie pas. Que grâce à l'intervention de l'État. On a réouvert certaines usines. Simplement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'que des secteurs entiers qui sont en train de distribuer et franchement la reconquête du du médicament par le paracétamol seul ne suffira pas. Nos collègues l'ont très bien exprimé. Je voudrais surtout dire que tout, tout le monde n'était pas béat devant la désindustrialisation. Les syndicats en particulier. Mais c'est la conséquence de cette vision de la mondialisation heureuse. Du libre-échange généralisé c'était pas grave de les prendre en Chine. Parce que ça coûtait moins cher. Hé ben justement aujourd'hui le temps est venu de rompre avec les politiques européennes qui font du libre-échange généralisé la règle et pas seulement dans les échanges internationaux

merci, la parole est à madame daphné Ract-Madoux pour le groupe Union centriste pour 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Face au retour en force d'un protectionnisme classique couplé à un réarmement commercial inédit. Il est plus que jamais nécessaire de bâtir une stratégie commerciale résolument ambitieuse afin de garantir la compétitivité à l'international de nos entreprises. Le travail prospectif menée par la délégation sénatoriale aux entreprises de ses rapporteurs et salutaire et permet d'inscrire ce sujet à l'agenda du débat. Du débat public. Je souhaite donc félicitée Florence Patrick compta Vincent Segouin Jean Grey pour la qualité de leurs travaux et de leurs recommandations. Un travail d'autant plus important qu'en matière commerciale, la sonnette d'alarme devaient être tirés depuis longtemps. Ainsi le déficit de la balance commerciale française s'est fortement aggravée en 2022 passant de 82 à près de 164 milliards d'euros en plus en plus d'un phénomène structurel connue connue de longue date le renchérissement de la facture énergétique associée à la forte dépréciation de l'euro face au dollar à se plonger notre balance commerciale. Chers collègues notre dépendance aux importations et nous le savons problématique et remet en cause notre souveraineté. Si l'on met de côté la question préoccupante de l'énergie notre déficit structurel s'est creusé dans des proportions inquiétantes. Fleuron français l'aéronautique vois ça balance excédentaire, passer de 31 milliards d'euros à 20 milliards entre 2019 et 2022, soit une chute de 35% sur 3 ans. Ah ces chiffres symptomatique d'une politique commerciale touchés par un mal profond s'ajoute une concurrence internationale acharnée. Avec la fin des restrictions sanitaires, Pékin renoue avec sa politique commerciale offensive en misant sur sa main d'oeuvre peu qualifiée et ces géants industriels ultracompétitif. Washington a récemment adopté une flèche réduction Act dotée de 370 milliards d'euros visant à soutenir des entreprises américaines produisant éoliennes, panneaux solaires et véhicules électriques. Avec nos partenaires européens. Nous devons agir rapidement pour permettre à nos entreprises de continuer à trouver des débouchés sur les marchés internationaux, tout en restant compétitives. Je salue à ce titre, l'action du gouvernement ayant conduit au niveau européen, à la mise en oeuvre un plan industriel communautaire pour un pacte Vert, présenté par la Commission, mercredi dernier. La création d'un fonds européen de souveraineté à destination de nos acteurs économiques est ainsi un signal fort envoyé par la commission. En complément, l'échelle nationale. Nous devons mieux accompagner nos TPE, PME et ETI à l'international. La mise en oeuvre de la Team France Export dans la lignée de la stratégie de Roubaix en février 2018 est à titre d'exemple, un véritable succès. C'est désormais un outil clé ayant accompagné. Plus de 10.500 PME et ETI françaises en 2021. Si nous ne pouvons que nous féliciter de ces réformes et de ces avancées. Il reste tant à faire. Mes chers collègues. 3 recommandations du rapport me semble devoir être soutenue à ce titre. Nous devons tout d'abord, continuer à investir dans la formation dans le secondaire et le supérieur afin de doter nos entreprises de professionnels Agile et à l'aise à l'international vous faciliter l'insertion nos entreprises sur les marchés. Nous devons ensuite mieux identifier les risques de vulnérabilité d'approvisionnement en utilisant les données douanières européennes c'est une condition impérative pour garantir notre souveraineté commerciale. Enfin. Il est urgent de définir une vision stratégique à horizon 2040 voire 2035 en matière de commerce extérieur avant de ça afin de s'attaquer aux racines structurelles de notre déficit. doit s'appuyer sur 2 piliers principaux, d'une part une meilleure synergie entre les nombreux et différents dispositifs existants. Pour une politique plus efficiente, et d'autre part, l'inscription dans une loi de programmation des objectifs précis de réduction du déficit afin de bâtir une trajectoire lisible et cohérente pour l'ensemble des acteurs. Mes chers collègues, nous le savons, le chantier est immense, il nous appartient désormais le mollet avec un engagement total. Merci. J'aurais éventuellement. La possibilité de reprendre après. Monsieur le Ministre.

Merci beaucoup madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs. Je partage évidemment avec vous un certain nombre de constats. En dehors de la situation exceptionnelle sur. La facture énergétique. Nous avons dans notre balance. Des biens. Un déficit structurel ce déficit structurel, on vient de le voir tout à l'heure. Répond pour une grande part à la question de la désindustrialisation et pour une autre part en réalité à la faiblesse de nos PME à l'exportation. Et ça c'est un sujet sur lequel nous travaillons avec la Team France Export. Vous parlez de la formation, je parlerai aussi de la culture de nos chefs d'entreprises à l'international, c'est-à-dire que nous avons en France cette particularité peut-être parce que notre pays est agréable et que l'on s'y sent bien. De ne pas être tourné instinctivement vers l'international et je pense qu'il y a là une véritable un véritable travail à faire, je me permettrai juste le temps mettant compter. Une remarque sur l'aéronautique puisque vous aviez pointé justement le fait que il manquait à peu près il y a. Aujourd'hui, un peu moins de 10 milliards d'euros par rapport au chiffre que l'on avait avant Covid sur la filière aéronautique. Nous sommes là véritablement dans un phénomène conjoncturel qui est celui. Évidemment de la baisse de régime du secteur durant le Covid et aujourd'hui surtout sur l'année 2022, j'avais le président d'Airbus au téléphone encore avant hier soir. Sur les semi-conducteurs. Il y a de très nombreux avions qui n'ont pas pu être livrés parce que les semi-conducteurs n'était pas là. Mais nous sommes très confiants sur la filière. On va rattraper ce retard. L'année 2023, on a plus de 7200 avions dans les carnets de commandes. Voilà donc on peut être tout à fait confiant sur le fait que la le secteur économique récupère. Le niveau d'avant-crise crise très prochainement. Merci. Merci Madame Ract-Madoux. Alors la parole est donc à Madame. Guilaine Pentel pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour cinq minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la délégation aux entreprises. Madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître la chanson d'Aznavour s'appliquerait bien à l'histoire de notre balance commerciale ces dernières décennies. Si les déficits de l'État, de la sécurité sociale bientôt un demi-siècle ah matière commerciale. La France était restée exportatrice nette de bien jusqu'au début des années 2000. À l'époque du gouvernement Jospin et de la gauche plurielle. Notre pays était encore une grande puissance commerciale en Europe et dans le monde. Depuis notre balance commerciale n'a cessé de se dégrader. Un cap supplémentaire a été franchi depuis la crise sanitaire, avec un déficit commercial qui a dépassé 80 milliards d'euros en 2021 et qui aurait explosé à plus de 50 milliards en 2022. En particulier, il est vrai à cause de la crise énergétique, entraîné par la guerre en Ukraine. Comment expliquer ce phénomène désormais structurelle, il faut mettre au crédit de la délégation sénatoriale aux entreprises de s'être penché sur cette question épineuse. Mais si important c'est importante Au sein d'une Union européenne qui équilibre à peu près ses comptes extérieurs, la France, à Paris, à la remorque de l'Allemagne et même de l'Italie qui ont su conserver une balance commerciale positive. Il y aurait des choses à dire sur le bien fondé d'un commerce demain aussi fortement excédentaire revers d'une consommation intérieure atone et des exportations parfois au détriment de ses partenaires européens. Ces questions sont débattues depuis des années avec les crises qui ont secoué la zone euro. Toutefois, cela ne nous empêche pas de regarder certaines réalités en face et de trouver des solutions aux faiblesses structurelles de l'économie française. Le Brexit a probablement renforcé ses difficultés car c'est avec le Royaume Uni que nous avions notre plus gros excédent commercial même si le coût principal du Brexit et bien sûr pour le Royaume Uni lui-même. Le déficit commercial de la phrase n'est pas due qu'à la facture énergétique. Cette dernière représente une part certes importante mais les pertes de parts de marché à l'exportation se sont accumulées dans de nombreux secteurs sur le long terme. cet affaiblissement touche aujourd'hui non seulement l'industrie mais aussi le secteur agroalimentaire. À neutre. Le rapport a mis à lumière les risques qui pèsent sur les services, avec le phénomène de télé émigra. C'est un phénomène qu'on a commencé à envisager avec la généralisation du télétravail mais mesure-t-on encore bien son ampleur. Le secteur des services et pourtant un domaine où la France reste exportatrice. Si l'on prend la balance courante et plus seulement la base de commerce de biens le déficit à 2021 et ramené à une vingtaine de milliards d'euros seulement. C'est une nuage intéressante face au discours souvent alarmiste malgré tout notre position extérieure nette n'a cessé de se dégrader sur une longue période. Les faiblesses de nos PME à l'export ne sont pas nouvelles. La France continue de manquer de grosses PME exportatrices, à l'instar de leurs homologues de leur homologue allemande ou italienne. Certains ont voulu incriminer la monnaie unique et l'absence de zone monétaire optimale, mais les difficultés similaires rencontrés par le Royaume-Uni qui n'a jamais été dans la zone euro montre que cette question est plus complexe. Face à tous ces défis, que faire. Indifféré 3 axes, d'abord, la remontée en garde de notre production. Nous devons impérativement, améliorer la qualité moyenne de nos produits dans nos nombreux secteurs, hormis quelques domaines d'excellence. L'économie française souffrent de se situer trop dans la moyenne gamme cette remontée nécessite d'importants investissements tant publics que privés. Ensuite le gaz. Le cadre réglementaire et fiscal. Un amendement proposé par mon groupe de la dernière loi de finances visait arbre à préserver la souveraineté économique dans le secteur des services numériques face au risque de prise de contrôle hostile. Le cadre concerne aussi les modalités de transposition des directives européennes. Dans ce domaine. Le Sénat pourrait, il pourrait lui-même lutter contre sa propre aux tendances à la surtransposition. A enfin et surtout la réindustrialisation doit aujourd'hui être le levier de la transition écologique. Dans ce domaine, les pouvoirs publics, États et collectivités entre. Collectivités territoriales hein. Rôle crucial à jouer. Voici les quelques remarques que je souhaitais faire au nom du groupe RDSE et qui sont loin d'épuiser ce vaste. Ce sujet merci. Merci cher collègue. Monsieur le Ministre. Dès que notre collègue a rejoint une place. Voilà. Merci. Merci beaucoup madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice. Vous me permettrez de ne pas être d'accord sur un certain nombre de points de votre propos. D'abord. Nous avons une situation qui est particulièrement conjoncturels sur l'énergie. Et qui est vrai d'ailleurs pour tous nos partenaires européens y compris l'Allemagne qui avait de très forts excédents et qui va voir ses excédents font de plus de 100 milliards d'euros et l'Italie qui était également habitué aux excédents et qui cette fois-ci, il va se retrouver comme nous comme nous dans un déficit commercial assez important. Donc on voit bien à quel point cette question de l'énergie, elle est conjoncturelle et elle emporte l'ensemble des pays européens. 2ème point de désaccord sur l'agroalimentaire, l'agroalimentaire. En France, est excédentaire. Nous avons plus de 10 milliards d'euros d'excédent sur l'agroalimentaire et ses 2 milliards de plus sur l'année 2022, c'est-à-dire que nous avons des filières sur les céréales et sur l'élevage tout particulièrement qui sont très dynamiques. C'est pas simplement les vins et spiritueux, donc ce sont des bonnes nouvelles pour le commerce extérieur français et. Un point évidemment sur lequel nous serons d'accord en revanche c'est. La question des des PME PMI. Nous avons effectivement à un tissu de PME PMI françaises plus faible que ce que nous avons en Allemagne et en Italie et surtout nos PME sont très faiblement. Vers l'exportation et c'est là le gros défi que nous avons devant nous, autant la la la réindustralisation ça prendra du temps. Je l'ai dit tout à l'heure, il faudra une décennie pour réindustrialiser notre pays en voir véritablement les effets autant les PME ne pouvons les pousser à l'exportation et c'est notamment le défi de la Team France exporte. Merci.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre, Madame et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le lent déclin de notre balance commerciale porte en lui. Nombre des maux qui affectent l'économie française depuis plusieurs décennies. Désindustrialisation, fiscalité écrasante sur la production et la transmission d'entreprise une structuration français qui peinent à installer d'intermédiaire entre petites et moyennes entreprises et entreprises du CAC 40. Lourdeur et complexité administrative. Bref nous traînons ses faire aux pieds depuis bien trop longtemps et je me réjouis que nos collègues de la délégation aux entreprises soient penchées. Je salue le travail des rapporteurs qui a pu aboutir à des propositions concrètes qui je l'espère seront entendus encourager car le constat est sévère mais hélas réaliste. La France n'exporte pas assez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et sont d'ailleurs particulièrement mauvais en ce qui concerne ces dernières années, le déficit commercial était de 84 milliards en 2021 pour atteindre le chiffre record de 160 milliards d'euros en 2022. Dans la période pré-Covid il était solidement ancrée autour de 60 milliards de déficit avec un plongeon significative de 15 milliards de déficits supplémentaires entre 2016 et 2017 à la racine de ce mal français la faible part de l'industrie dans le produit intérieur but brut qui n'a cessé de plonger aujourd'hui sa part dans le PIB n'est que de 13 et demi % quand la moyenne européenne et autour de 15%. Pour rappel, ces 24 deux en Allemagne, 19, 6 en Italie ou 15, 8 en Espagne. Vous trouverez tous ces chiffres dans le très bon rapport de mes collègues Florence. Compta Jean hein gré et Vincent Segouin. Revenons d'ailleurs quelques années en arrière lorsque sous l'impulsion de certaines théories économiques, nous pensions que ce monde qui vient serait celui des services et non plus de l'industrie, avec cette idée folle des mêmes auteurs. Les pays développés délocaliseraient leur production à l'étranger pour ne garder que les services malheureusement l'hémorragie qui s'en est suivi, chacun la connaît notre industrie a payé un lourd tribut à ses idées mortifères, perdant 10 points dans la part du PIB quel. Pour mémoire, chers collègues. Le déficit commercial de la France était jusqu'alors inférieur à l'Allemagne. Un exemple symptomatique. Comment expliquer aujourd'hui que les constructeurs automobiles français parmi les plus importants au monde pèse si peu dans les exportations nationales. C'est là particulièrement frappant notre industrie automobile s'est délocalisé depuis 20 ans. Attirés par le cou attractive de la main d'oeuvre étrangère. Dans le même temps, l'industrie automobile allemande s'est adossée sur les anciens pays d'Europe centrale et orientale comme arrière-boutique tout en conservant un assemblage final en Allemagne Made in Germany. Résultat notre balance commerciale automobile n'a plus été excédentaire depuis 2004 et comble de l'ironie, certains constructeurs français sont aujourd'hui devenus importateur sur le marché national. Nous devons être interpellé par ces exemples qui pourrait être multipliée s'appliquer à bien des domaines ces dernières décennies en partant de ce triste constat. Un autre émerge les productions étrangères afflux maintenant en quantité sur le territoire national. Nous sommes devenus un pays d'importation des denrées et des produits du bout du monde dans des emballages, du bout du monde. Notre notre déficit commercial ne l'évalue pas mais nous important en réalité les déchets de demain. Les mêmes qui n'ont créé ni emploi ni richesse ni savoir-faire dans notre pays. Monsieur le Ministre, je plaide pour que nos politiques publiques prennent conscience de ce fait d'. Soutiens de la création d'une puissante filière industrielle française de traitement des déchets compétitives et innovantes. Dans un contexte de rareté de diminution des ressources mondiales repensons notre rapport aux déchets. s'assurer aujourd'hui de leur valorisation c'est permettre demain de garder un levier important sur les ressources. Développer une puissante filière française du recyclage et du réemploi sera incontestablement également moyen de création d'emplois et de développement économiques dans nos territoires et nous aidera à changer notre rapport aux échanges commerciaux. Notre pays a de nombreux atouts à faire valoir qui nous permettrait de retrouver de la compétitivité et de garantir notre souveraineté nos politiques publiques doivent en tenir compte, valoriser et accompagner ses atouts pour que la France redevienne une grande puissance commerciale. Sortons de la mondialisation heureuse, qui nous a fait si mal par le passé redécouvrons un État stratège qui garantit notre souveraineté et notre autonomie stratégique. Je ne saurais pas plus longue chers collègue.

Je partage également votre préoccupation sur la question de la valorisation des déchets et du traitement des déchets. Nous avons besoin d'une politique industrielle dans ce domaine-là et ça fait partie des orientations du plan France 2030 notamment en ce qui concerne les matériaux. C'est d'ailleurs on va dire une étape indispensable pour la mise en place de cette économie circulaire que nous appelons évidemment. De notre voeu pour la défense de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Donc vous voyez qu'on a des des analyses extrêmement proches juste sur l'automobile. Nous avons des chiffres qui aujourd'hui sont plutôt encourageants puisque nous avons dans cette année très particulière, encore une fois où on a beaucoup manqué de semiconducteurs pour soutenir justement la production automobile en dépit de ça. Nous avons des chiffres dans le secteur automobile qui rejoignent la situation d'avant Covid. Donc nous avons rattrapé si vous voulez le retard que nous avions. L'année précédente et c'est aussi une bonne nouvelle pour ce secteur. Merci madame de Cidrac. Merci, monsieur le Ministre. Bien évidemment, je suis aussi d'accord sur ce que vous venez de dire, puisque vous étiez d'accord avec mes propres propos donc évidemment on est d'accord. Simplement je voudrais vraiment insister sur un aspect qui est important me semble-t-il, c'est que nous nous importons beaucoup nous n'exportons pas assez donc soutenons aussi des talents et des savoir-faire typiquement français. J'ai presque envie dire de fait même que nous sommes pays d'importateurs, nous pouvons aussi. Exporter ce savoir-faire dans beaucoup de pays y compris en Europe car nous avons de vrais talents en la matière et de très belles entreprises pas que de goût très grosse parfois les PME et les TPE sont très bonnes en ces matières là voilà. Merci. La parole est à Madame Vanina Paoli-Gagin pour le groupe les indépendants pour cinq minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, Madame et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le creusement progressif de notre déficit commercial dure depuis tant d'années que certains s'y sont presque habitué allant jusqu'à le qualifier de structurel. Chaque année plus le déficit tricolore s'enlise plus il devient urgent de redresser la barre. Chaque année. Les mauvais choix de ces 30 dernières années en matière de politique industrielle se Thanou. Pourtant les alertes se sont multipliées à l'instar du rapport déposé en 2018 par mon collègue Jean-Pierre de colle sur la pénurie de médicaments. Ils demeurent malheureusement. Toujours d'actualité. J'ai un petit problème. De papier. C'est vrai. La crise Covid a braqué un projecteur sans concession sur notre décrochage industriel et la perte de compétitivité de nos entreprises. Elle a posé une lumière crue sur le vieillissement de notre appareil productif sur les délocalisations de nos emplois sur la chute ininterrompue de nombreux de nos talents et sur l'inadéquation de notre positionnement milieu de gamme. Cela a déjà été dit. Alors que nous sommes confrontés de plein fouet aux pénuries au renchérissement du coût de l'énergie à notre dépendance aux importations les manquements de notre politique commerciale nous oblige à. S'accorder sur un même constat hein est un 1er pas réaliser un état des lieux des 900 postes et produits affichant un déficit supérieur à 50 millions d'euros, comme l'a fait. Le Haut Commissariat au Plan et déjà une bonne chose. Désormais, nous devons surtout agir et vite. L'étude de notre balance commerciale pose aussi la question de notre politique dédiée à la recherche. Lisbonne et mourir. C'est un peu ce que nous avons fait hélas Monsieur le Ministre. Je vous le rappelle, mes chers collègues, l'Europe devait être l'économie la plus compétitive du monde en 2010 et nous devions consacrer 3% de notre PIB à la R&D. La France est malheureusement encore loin du compte. Pourtant, les chiffres montrent bien que des entreprises actives en R&D exporte plus. Nos grandes entreprises impliquées en R&D réalise 31% de leur chiffre d'affaires à l'export. Contre 23% pour le reste des grandes entreprises. C'est encore plus flagrant flagrant pardon pour les PME, celles qui sont actives en R&D réalisent 29% de leur chiffre d'affaires à l'export, contre seulement 10% pour l'ensemble des PME. J'ai bon espoir Monsieur le Ministre, dans le prend le plan flanc France 2030 même si des lourdeurs bureaucratiques freinent encore son déploiement. Il met l'accent sur la formation et la recherche. Qu'on a aussi pris en compte dans la LPR. Dans des domaines stratégiques. Parmi eux le spatial décarbonation de l'industrie et la santé sont des secteurs dans laquelle la France doit rapidement se positionner. Développer une stratégie française en faveur de la recherche est un enjeu de souveraineté majeur et nous avons encore de bonnes raisons d'espérer dans certains domaines. La France, c'est même très bien positionnée le luxe ou l'agroalimentaire bien sûr ont été évoqués. Mais d'autres secteurs encore représente fièrement notre pays à l'international. Parmi eux, je voudrais saluer le secteur du jouet et du jeu de société tout un écosystème de talentueux professionnels dont on parle peu qui s'emploie à soutenir la dynamique de cette industrie qui, par la conquête des marchés internationaux. Dans l'Aube. C'est le cas par exemple de l'entreprise férié au CRIC à Mussy sur scène. international international des Jeux se tiendra à Cannes à la fin du mois, sa présidente édition avait réuni plus de 80.000 passionnés venant du monde entier. Une réussite du Made in France qui soulignent l'urgence du rapatriement de certaines productions comme les éléments magnétiques ou encore les puces électroniques, ces exemples redonne de l'espoir mais ne peuvent malheureusement faire oublier la gravité de la situation. Le statu quo n'est plus permis. Dans le rapport d'information transformer l'essai de l'innovation un impératif pour réindustrialiser la France, dont j'étais le rapporteur nous dénoncions le saupoudrage d'aides publiques, mais aussi les délais d'autorisation de mise sur le marché et caetera. Ces délais sont incompatibles avec le développement rapide des secteurs technologiques innovants. À titre d'exemple, sur les bio-contrôle qui vous le savez, sont des substituts. Aux. Pesticides ou la France et innovante. Il faut, c'est à 18 mois aux USA et 7000 dollars avec la procédure Fast Track pour homologuer un produit il faut 18. Voire Voire plutôt 36 mois auprès de l'EFSA a des coûts bien supérieur et encore en passant par la Belgique car nos 37 en France est submergé est saturé. C'est un vrai problème de commerce extérieur, Monsieur le Ministre indirect et c'est un vrai problème, ça coûte à nos entreprises elles subissent des décalages dans leur plan d'affaires. Elles perdent leur avance compétitive. J'espère que l'IRA européen viendra apporter les améliorations nécessaires pour stopper l'hémorragie. Je vous remercie. Si. Merci cher collègue. vous pouvez vous installer où vous voulez hein. Madame Paoli-Gagin. Bien sûr. Pas de souci. Bien. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. Je suis d'accord avec vous. Sur de nombreux points, notamment sur un il faut agir et vite. Et c'est ce que nous faisons, notamment à travers le plan France 2030 en matière d'innovation. Parce que vous avez parfaitement raison. Il faut relocaliser il a un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs stratégiques. On a parlé tout à l'heure des semi-conducteurs. On a parlé de la pharmacie avec un certain nombre de médicaments essentiels. On peut parler également. De composants nécessaires à la transition énergétique. Que les batteries et donc les matières premières dont on a besoin pour confectionner ses batteries mais on ne va pas tout relocaliser pourquoi parce que et ça a été dit très justement tout à l'heure. On ne va pas se lancer aujourd'hui dans une nouvelle compétition de compétitivité coût on trouvera toujours des pays. Dans le monde, si ce n'est pas l'Asie, demain ce sera l'Afrique. Où on arrivera à produire des produits à faible valeur ajoutée à des coûts bien moins important que ce que nous ferons en France et donc il est important. De d'accès aujourd'hui la réindustralisation. En dehors de ce que je viens de dire sur les matières stratégiques sur les questions. D'innovation, c'est-à-dire les produits qui porteront la croissance des prochaines décennies et c'est ce que nous faisons dans France 2030 à travers les énergies du futur à travers les biotechnologies travers les mobilités du futur. C'est ça le combat. Et vous pouvez compter évidemment sur le gouvernement pour agir et vite dans ces domaines. Merci. Même Paoli-Gagin, vous souhaitez répondre. C'est doux à mes oreilles. Monsieur le Ministre, mais j'avais quand même pointé le fait que. Nos réglementations ou aux délais d'homologation. c'est vraiment un caillou dans la chaussure des innovateurs dans notre pays. Ils partent en ce moment au Canada, aux États-Unis on leur construit des usines qu'qui sont payés à 80%. On leur garantit un prix de l'électricité sur 10 ans et on leur permet d'homologuer leurs produits, ils vont revenir via les procédures OCDE en Europe et en France, est-ce qu'ils vont revenir rapatrier la production chez nous, je le souhaite, mais c'est pas sûr. Merci. La parole est à Monsieur Daniel Salmon pour le groupe écologiste solidarité et territoires pour cinq minutes. Madame Madame la présidente. Monsieur le Ministre, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. Notre pays affiche un déficit record qui atteint désormais 150 milliards fin 2022, comme le souligne justement ce rapport les raisons des contre-performances ont déjà été évoqués et puis c'est des contre- performances à répétition du commerce extérieur, elles sont connues, il est déficitaire maintenant maintenant depuis près de 20 ans et l'envolée de la facture énergétique. Le ralentissement du commerce mondial et la dépréciation de l'euro face au dollar ont accentué son plongeon. Mais c'est bien évidemment les achats d'énergie d'hydrocarbures bien sûr et les importations d'électricité qui pèse le plus dans le creusement de ces derniers mois. Permettez-moi donc d'accès mon discours mon propos sur cet angle énergétique qui est l'une des raisons majeures de notre vulnérabilité et de notre déficit commercial. France. Qu'en France. Près des 2 tiers de notre consommation énergétique dépendent encore des énergies fossiles, dont une partie est toujours portée de Russie. Une situation de dépendance mortifère pour le climat pour la paix. Critique pour nos comptes publics et qui n'épargne pas non plus le pouvoir de vivres de nos concitoyens. L'objectif de la Commission européenne à travers le plan ripoux joueurs qui vise à se passer du pétrole, gaz et charbon russes d'ici à 2027 et bien sûr nécessaire mais le réveil hé bien tardif. Les importations d'électricité pèse également dans le creusement de ces derniers mois, nous l'avons dit, notamment du fait de l'indisponibilité de nombreux réacteurs nucléaires. Fait qui me permettent de rappeler l'impérieuse nécessité du déploiement des énergies renouvelables pour notre souveraineté énergétique en premier le premier lieu et pour contribuer de facto à la bonne santé de notre balance commerciale. Alors qu'elle représente la source d'électricité bas-carbone et compétitive pouvant être déployée massivement sur le territoire à l'horizon 2030. Nous ne pouvons que déplorer notre faiblesse en la matière et ceci à plusieurs niveaux importations d'électricité donc mais importations également des moyens de production et bien sûr faiblesses de nos exportations. Sur l'éolien, les Danois, les Allemands sont à l'avant-garde du marché mondial. Aucun constructeur français dans les 10 premiers sur le photovoltaïque c'est la Chine qui monopolise aujourd'hui toutes les étapes de la chaîne de production en pratiquant du dumping social et environnemental, sans que la Commission européenne n'y trouve à redire. En ayant investi 50 milliards de dollars dans le développement du secteur dès 2011 10 fois plus que l'Europe, sa part de marché mondiale dépasse les 80%, alors que l'Union européenne importe 84% de ces équipements. La Chine domine à présent les chaînes d'approvisionnement dans leur ensemble toutes sur toutes ces technologies essentielles à la transition. En plus du solaire. Nous pouvons également les véhicules électriques et le stockage d'électricité. Dans le domaine de l'hydroélectricité. La France ne tient pas non plus son rang au niveau de l'exportation de sa technologie. Alors que sur ces questions majeures, la France et l'Europe accumule un retard préoccupant. Le plan anti-inflation adoptée en 2022, États-Unis visant à combattre le changement climatique favorise la relocalisation industrielle dans des secteurs stratégiques de la transition. L'inflation réduction Act mettent en place un arsenal de mesures incitatives, notamment via des crédits d'impôt à l'investissement et à la production d'équipements de la transition énergétique pour une enveloppe de 369 milliards d'euros avec un objectif de relocaliser une capacité intégrée de 50 gigawatts par an d'ici 2030 50 gigawatts. Ce n'est pas rien. Face à ces subventions massives pour relocaliser la production des moyens de production d'ENR de la part des autres grandes puissances. Quelles initiatives, Monsieur le Ministre, la France va-t-elle engager pour une réelle relocalisation de la chaîne de valeur comment notre pays se donne-t-il les moyens de redevenir constructeur et exportateur dans ces filières qui hélas n'ont jamais été soutenu. Si la France veut sécuriser son découplage énergétique avec la Russie et les autres pays et garder la distance dans la transition vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Elle doit reconstruire une base industrielle sur son territoire en la tournant résolument vers la transition écologique. Cela passe par la fabrication des équipements au plus près mais aussi par la mise en place d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe en privilégiant l'industrie plutôt que la libre concurrence. Oui le combat face au changement climatique bah favoriser plus que jamais la recoller relocalisation de la production dans ces dans ces filières clé et là des industriels active dans la transition ont aujourd'hui besoin de visibilité pour démarrer des investissements très coûteuses en capital. Vous annoncer un projet de loi cette année pour une industrie verte qui devrait être l'occasion de répondre à ces défis majeurs mais sans amorcer un réel changement de paradigme dans des politiques publiques sans introduire la moindre conditionnalité à l'attribution d'aides publiques sans un Net investissement massif dans les ENR, le feu restera un voeu pieux. Ils vont bien.

Merci beaucoup madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. 1 point. Juste d'information sur le pétrole brut russe d'où sommes arrivés à 0% donc il y a plus d'importations de pétrole brut russe en France à l'heure à laquelle je vous parle de la même manière qu'il n'y a plus de soutien. Public. Que ce soit à l'export ou ailleurs sur les énergies fossiles. Nous partageons évidemment un constat. C'est que il n'y aura pas de réindustrialisation possible si il n'y a pas une énergie abondante et pas chère, pour avoir une énergie abondante et pas chère. Nous devons être à la fois dans les énergies renouvelables mais nous devons être aussi dans les énergies bas carbone. Parce que c'est ce qui permettra de répondre à la demande qui sera probablement croissante ces prochaines années en terme d'énergie. Et donc le plan France 2030. Qui soutient la réindustrialisation dont nous parlions à l'instant. A mis en place les soutiens nécessaires pour que l'on puisse à la fois dans l'éolien Offshore mais aussi dans les nouveaux réacteurs nucléaires notamment les petits réacteurs modulaires. Avoir un temps d'avance en matière technologique par rapport à nos principaux compétiteurs ça m'offre l'occasion très. Rapidement, puisque le temps m'est compté. D'aborder tchétchène ouais Duchesne acte. Il est évident que ce que nous lançons au niveau européen. Ne peut marcher que si nous avons une concurrence qui est qu'une concurrence équitable et loyale notamment vis-à-vis de nos alliés américains et donc nous sommes en discussion avec les États-Unis d'Amérique et en parallèle à ces discussions, nous avons également un plan européen qui est en train de se monter, qui sera au menu du Conseil européen qui se réunira en fin de semaine à Bruxelles et je suis particulièrement confiant sur le fait que nous arriverons à trouver ensemble les réponses pour assurer la compétitivité de nos entreprises dans ces secteurs là en Europe et particulièrement en France. Merci Monsieur Salmon. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre. Nous avons un désaccord de fond. Je pense que d'investissements dans le nucléaire clairement va nous donner plutôt un temps de retard. Encore une nouvelle fois sur les énergies renouvelables. Je vais vous donner aussi un exemple sur les problèmes sur le commerce extérieur. Je suis président du groupe d'amitié France-, Népal, je me suis rendu au Népal. En septembre dernier. Il y a un projet d'hydroélectricité. Vous savez que le Népal a un potentiel d'hydroélectricité gigantesque 50 gigawatts potentiellement et ils attendent des partenaires. La France avec EDF est engagé dans un projet, ça fait des années et ça patine, ça n'avance pas. Un autre exemple. Katmandou attends d'avoir un téléphérique. Il y a une société iséroise Poma qui est engagé sur ce projet, ça fait là également des années et on avance pas. Donc je pense qu'on a vraiment une nécessité d'être plus offensif et d'arriver à peser et arrivé à débloquer ces problèmes qui enfin c'est ces projets qui sont vraiment excellents pour le commerce extérieur français. Si. La parole est à monsieur Jean Baptiste Lemoyne pour le groupe. Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Bonjour et pour six minutes. Merci beaucoup madame la présidente, madame, messieurs les rapporteurs. Monsieur le Ministre, bon c'est pas la Saint-Olivier aujourd'hui parce que c'est le 12 juillet, je vous l'apprends. Mais c'est votre journée je crois entre ce débat ce soir les chiffres rendus publics par la douane ce matin avec effectivement ce nouveau record qui a été atteint en terme de de déficit commercial. Avec ses mois 163 milliards d'euros et et là ça devient un peu un marronnier en réalité. Et on a coutume effectivement chaque mois de février de verser des larmes de crocodile sur les chiffres du commerce extérieur depuis 20 ans parce que la tendance à Leila parce qu'elle est lourde. Mais l'examen attentif des chiffres je crois. Doit également inciter néanmoins à ne pas perdre espoir. Parce que le chiffre en pied de colonne il cache en réalité. Beaucoup de de nuances beaucoup de surprises. Et je crois qu'il faut voir tous ces éléments en tête pour effectivement bâtir une approche stratégique comme l'appelle de nouveau les rapporteurs et donc quelques éléments peut être que je voulais. Mettre à jour. À travers les chiffres rendus publics ce matin bon première chose, ça a été dit je paye revenir trop longtemps la part importante de l'énergie dans le déficit. 80% de l'accroissement du déficit lié au renchérissement de la facture énergétique et donc en mettant les bouchées doubles sur cette transition énergétique, on voit qu'on apporte une réponse structurelle à. Une partie ne d'autres déficits et imaginer le monde de demain avec une France autonome en énergie. D'ailleurs on on le voit hein. La Banque de France qui aussi publié ce matin un certain nombre de données le dit le déficit des biens hors énergie. Et stable, à moins 24 milliards d'euros. Donc je crois qu'il faut également pointé cet élément.

jusqu'en 2025. Capital 2ème point que je relève, c'est l'augmentation du nombre d'entreprises exportatrices est également l'augmentation des exportations et lorsqu'en 2018, nous avions lancé la stratégie Team France Export, le pari, c'était d'augmenter le nombre d'entreprises exportatrices, pari tenu, pari gagné. On en était à 123.000 entreprises exportatrices. En 2017, on en est à 144.000, plus de 21.000. Et donc c'est 17% de croissance et tiens d'ailleurs. La vie est bien fait, on est à 18% d'augmentation également des exportations. Alors il y a une part pris bien sûr mais également une part liée à à ces nouveaux exportateurs et ce qu'il faut c'est travailler au fait que, hé bien ses exportateurs. Le fasse pas un coup mais. De façon assez assez d'où le rôle des veilles j'insiste là-dessus véritable école d'application de l'export. Ces volontaires internationaux pour pour l'export. D'où le rôle également de cette TFE Team France Export. Je veux saluer l'engagement des régions de Business France des CCI à l'international de BPI. Des conseillers du commerce extérieur naturellement sans oublier. Les OACI et nos ambassadeurs. Parce que. Très clairement, là il y a une dynamique qui s'est mise en place et qui permettra de continuer à aller de l'avant. Parce qu'il va falloir faire encore plus, c'est encore mieux dans la mesure où les fantasmes au niveau mondial croissent plus vite que les exportations françaises et donc notre part de marché, elle a tendance à se réduire. 3ème point. À mon avis à relever, c'est que nous devons continuer à avoir une politique commerciale particulièrement exigeante vis-à-vis de nos partenaires. À la fois partenaires européens et partenaires internationaux réciprocité souveraineté c'était encore il y a quelques années, des gros mots dans les couloirs et les antichambres bruxelloise Georges ou que les choses et quand même évolué. Pour mettre plus d'équité dans un certain nombre d'accord et notamment commerciaux en juin 22. Les ministre de l'Agriculture sont tombés d'accord sur justement l'idée des clauses miroirs mais très clairement, il faut aussi que la partie commerce de la commission prenne en compte tout cela parce qu'un certain nombre d'accord modernisés, qui sont dits de nouvelle génération mais qui ne sont pas d'une génération à ces nouvelles pour nous Français, je le dis très clairement. Il faut être encore plus volontariste de cette façon-là pour que nos normes deviennent des normes non pas seulement européenne mais des normes qui s'imposent au niveau mondial. 4ème point peut être. Et beaucoup d'orateurs. Ont insisté également là dessus. Auparavant, la nécessaire relocalisation d'activités industrielles et la planification que France 2030 permet c'est vrai que post-Covid. On voit un ajustement dans les chaînes de valeur ces relocalisations. Qui sont à l'oeuvre et et pour lesquels d'ailleurs. Effectivement le gouvernement mais mais beaucoup d'impulsion. On a parlé des microprocesseurs. On peut parler aussi des membranes d'électrolyseurs pour produire l'hydrogène décarboné bientôt qui se feront en France et puis l'attractivité du site France à travers un certain nombre de mesures qui ont été prises depuis plusieurs années, sans être naïf parce que les investissements, il faut aussi regarder qui sont les investisseurs d'où le filtrage nécessaire aussi pour un certain nombre d'investissements stratégiques et puis on est dans un monde de re régionalisation des échanges, il faut le dire et de ce point de vue là, nous avons aussi la force. d'un certain nombre de filiales françaises établies à l'étranger et donc le Made in France doit être aussi complété par le Made by France si je puis dire tous ces entrepreneurs français à établir de France, les Français de l'étranger qui participent aussi. Hé bien à leur façon à notre présence à l'international qui est très différente de nos amis allemands ou italiens. Et puis enfin pour avoir une vue complète les services qui sont un vrai atout le tourisme, on le voit. Et donc, un seul des transactions courantes qui est. Qui était positif, mais en 2021 et qui sent le renchérissement de la facture énergétique de 2022 serait encore plus positif fois deux à 17 milliards d'euros et donc comme j'arrive presque au bout de mon temps, je laisserai le ministre pondre pour reprendre la parole est achevé mon propos. Madame la présidente. Parfait. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, D'abord je voudrais rendre hommage. Au travail que vous avez effectué, lorsque vous étiez. Au ministère, à ma place pour le lancement de la Team France Export parce que ce que vous avez dit est très juste. Si aujourd'hui nous avons une vraie dynamique. Notamment qui permet d'accompagner nos entreprises davantage à l'exportation, c'est parce que nous avons su rassembler qui a les acteurs à savoir Business France. Les chambres de commerce et d'industrie à la BPI. Les régions qui gèrent le guichet unique et derrière également d'autres acteurs que sont les conseillers du commerce extérieur de la France, les SCI. Et bien d'autres. Nous avons su les rassembler et les faire travailler en équipe, là où souvent ils étaient plutôt en compétition les uns avec les autres et donc c'est une très bonne nouvelle, la Team France Export, c'est une vraie réussite. Ça marche. 2ème point les VIE. C'est un vrai succès également. Il y a eu un petit. Creux évidemment au cours de la crise sanitaire, parce que les frontières étaient fermées, certains pays était tout simplement inaccessible. Aujourd'hui la très bonne nouvelle, c'est que les affaires ont repris, si je puis me permettre et nous avons 1000 départs de veille par mois par mois, donc ça aussi c'est une situation extrêmement. Favorable qui nous laisse. Penser que nous allons, là aussi avoir des succès futur avec nos entreprises qui se porte à l'international et puis le, le dernier point. C'est pour dire évidemment que je partageais totalement l'ambition du Made by France s'agit absolument pas d'encourager la délocalisation. Il s'agit de reconnaître les entreprises françaises de l'étranger qui a qui participent au rayonnement de notre pays et je souhaite que l'on puisse. Arriver à un concept dans le cadre de la marque France. Merci Pour poursuivre et terminer. Dire que on peut en termes d'accompagnement micro auprès des des PME effectivement conforter le rôle de la TFE, vous avez lancé l'ambassadeur et c'est et c'est très bien. Je veux dire aussi le rôle des salons très important. À la fois les salons en France et les salons hors de France. Très important d'aider les entreprises à y aller de faire venir des acheteurs internationaux. Et pour ça, hé ben voilà il faut effectivement des crédits. Et puis. Dire que il y a aussi ce beau projet des vitrines je sais à un jet de Pierre de Roissy que porte Évelyne Renaud va Garabédian et, et Jean-Pierre Bansard. Tout ce qui permet de mettre en avant ce Made in France où se by France et bienvenue. Et puis enfin ayons cet état d'esprit conquérant, une véritable démarche d'Intelligence économique, c'est un sujet cher également à Marie-Noëlle Lienemann et tout ça me fait dire que 2022 a peut-être le goût d'une bataille perdue mais que on va mener les combats à venir, et que la guerre économique on la gagnera je parle de guerre économique parce que c'est bien le climat actuel dans les rations commercial. Merci. La parole est à Madame, Florence. Compta. Pour le groupe socialiste, écologiste républicains pour cinq minutes, chers collègues. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cela a été dit la balance commerciale de la France est en déficit chronique depuis 2002. Devenu abyssal ces dernières années, et pire, au sein de l'Union européenne, la France se classe en avions le plus fort. Nous avions le plus fort déficit en 2021, donc la délégation aux entreprises dans son rapport à à tenter d'éclairer le sujet d'avancer des propositions et je remercie le président babary de nous permettre de débattre ce soir de ce rapport, oh oh combien stratégique pour notre économie. Je voudrais donc m'attacher maintenant au nom des sénateurs socialistes, écologistes et républicain, a souligné quelques-uns des aspects qui nous semble important. Cela a été dit la dégradation des performances de notre commerce extérieur est le fruit de la désindustrialisation de notre pays. En attestent les données récentes qui a relevé notre collègue Marie-Noëlle Lienemann sur la part de l'industrie manufacturière dans le PIB qui a été évalué à 9% 9% qui est passé sous la barre des 10%. Et qui nous relègue là aussi dans les tréfonds du classement européen. Et si on va à l'intérieur puisque je n'aurai pas une vision. Aussi rose que mon précédent collègues sur. Le. Le le notre commerce extérieur parce que on a quand même des points très négatif. L'automobile au début des années 2000, on avait un excédent dans ce secteur on a aujourd'hui un déficit de 18 milliards les autres biens industriels le déficit était d'une dizaine de milliards. Au début des années 2000 on était l'année dernière à 66 milliards, l'aéronautique, quant à elle n'a pas retrouvé sa dynamique d'avant crise et il nous reste bien que le secteur du luxe et des. Et des cosmétiques qui semble progresser, c'est quand même très inquiétant. On peut toutefois se rassurer en évoquant la balance des services qui existent et qui excédentaire mais qui ne parvient pas à combler le déficit grandissant des biens et on peut craindre pour l'avenir parce que si la production de bien a été. Délocalisée celle des services, enfin certains services pourront l'être à l'avenir et par ailleurs, le rapport montre que le le exportation de biens et de services sont intimement liés et donc face à cette dégradation continue. Il faut réagir et cela a été évoqué par plusieurs collègues à partir d'une analyse stratégique sérieuse il faut interroger nos choix de spécialisation et analyser nos avantages comparatifs dans un environnement certes incertain. Il nous faudra construire des avantages comparatifs porteur pour l'avenir. Nos collègues de la commission des affaires économiques ont déterminé 5 plan principaux pour reconstruire notre souveraineté économique en France, en Europe et c'est une piste qu'il faut à mon avis approfondir et mettre en oeuvre donc cette vision stratégique de moyen terme, nous devons la construire et si la compétitivité prix n'est pas à négliger. Elle doit bien entendu prendre en compte la compétitivité hors prix notamment l'innovation et le capital humain. La recherche constante de l'innovation tant dans les produits que dans les process est une dimension essentielle de la compétitivité est le tournant des transitions numérique et écologique doit être pris en effet alors ou le changement climatique et la transition énergétique qu'il implique percute nos 4 traditionnel de penser notre système productif une seconde transformation est à l'oeuvre la numérisation et la digitalisation et donc c'est transition écologique et numérique au Juan impact sur les formes des échanges économiques et sur la mondialisation et donc c'est dans ce nouveau contexte global qu'il nous faut désormais penser le commerce extérieur. Ce sont ces éléments qui doivent devenir demain des leviers de la compétitivité de l'économie française et européenne. Donc monsieur le ministre, est-ce que les services comment les services ministériels travaille-t-il sur une feuille de route géographique sectoriel pour anticiper ce que seront demain les échanges économiques dans le monde et donc notre commerce extérieur, alors qu'on envisage partout, ça a été peu soulever dans le débat mais on envisage partout et dans de nombreux domaines des circuits courts et des relocalisations donc quel. Commerce extérieur. Dans ce cadre là comment construire de nouveaux avantages comparatifs qui allient compétitivité et ambitions climatiques Les limites de la stratégie de Business France. Comment allez-vous faire évoluer les les actions de Business France et enfin comment envisagez-vous la place de nos PME ETI dans la nouvelle donne du commerce mondial. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs. Madame triste. Alors d'abord permis vois juste. Peut être de 2 nuancé. Sur votre propos. En ce qui concerne les grands secteurs exportateurs. Nous avons. Des grands secteurs qui continuent à avoir des excédents majeur. C'est le cas de l'aéronautique, c'est le cas de la pharmacie, c'est le cas de l'agro-alimentaire. C'est le cas des cosmétiques. C'est le cas de la construction navale encore 3 milliards. D'excédents cette année, donc nous avons. La chance d'avoir en France. Des champions des très grands groupes qui sont des champions mondiaux et qui porte. Ses exportations. La faiblesse. De nos exportations françaises c'est que derrière ces très grands groupes qui porte à peu près avec les uti. 87% des exportations françaises. Nos. PME PMI elle ne porte que 13% de nos exportations et c'est là que nous devons porter véritablement le combat parce que c'est là que nous avons des marges de manoeuvre. Importante en ce qui concerne la feuille de route sectorielles, elle existe et elle est portée par France 2030, ce sont les priorités de France 2030, ce sont les grands secteurs de croissance des prochaines décennies dans lesquelles nous devons investir pour faire en sorte que les industries que nous développons à travers France 2030 souhaitent aussi et ensuite sur la question géographique. Bien sûr l'analyse existe. Mais comme je dis souvent aux entreprises. Je ne veux pas les restreints dans leur choix géographique. Pourquoi parce que. Le slogan qu'elle devrait avoir. C'est à voir le monde comme horizon. Il y a des grands, c'est des des des grands secteurs de croissance aujourd'hui l'Asie demain l'Afrique très certainement, mais enfin ne pas négliger non plus l'Amérique latine. Il faut que pour une entreprise. qui soient performantes à l'export, il faut impérativement qu'elle est demain le monde que Morison merci. Merci Je vous remercie Monsieur le Ministre, le monde comme horizon certes mais je crois que c'était un élément soulevé par la Cour des comptes dans le dans son récent rapport sur. Notamment l'accompagnement à l'export que ce ne sont pas forcément les pays qui seraient les plus stratégiques qui sont les dans lesquelles nos entreprises sont les mieux accompagner donc je pense qu'on a quand même un vrai sujet à retravailler la su et compris sur la sectorisation. Il ne faudrait pas qu'on rate quand même le les les secteurs porteurs de demain je pense. on entend beaucoup parler, on en ce moment de tchatcher pythie mais de l'Intelligence artificielle du Cloud. Souverain qui est devenu un Cloud de confiance, il faut vraiment qu'on a des ambitions dans ces domaines là, je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Michel qui navette pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les et Madame les rapporteurs, chers collègues. Le groupe de l'Union centriste tiens à remercier la délégation sénatoriale aux entreprises d'avoir mené un travail sur cette question essentielle du commerce extérieur et aux 3 rapporteur d'avoir justement formulé 10 propositions qui doivent permettre. D'améliorer la situation parce que la situation, Monsieur le Ministre, cela a été dit par les précédents orateurs à la tribune. Elle n'est pas. Elle est pas très bonne il faut reconnaître avec 164 milliards de déficit en 2022. De la balance commerciale française, donc une augmentation très significative, c'est quasiment le doublement Hé bien sûr la facture énergétique n'est pas la seule raison de cette. Ah ah augmentation extrêmement significative, elle explique une partie de l'importance du montant mais pas seulement hein et ceci interroge d'ailleurs sur la stratégie. Énergétique, nous pouvons avoir sur notre pays Mais Monsieur le Ministre. Le groupe de l'Union centriste estime que ce n'est pas une fatalité et qu'il faut effectivement que nous prenions les sujets à bras le corps pour arriver à formuler des propositions. Alors les propositions. On les a vus il y a notamment la première proposition qui porte sur. Une loi d'orientation sur les questions de commerce extérieur nous pensons effectivement au niveau du groupe de l'Union centriste qu'il est important que la feuille de route soit particulièrement bien tracé bien définies que nous puissions la définir ensemble cette. C'est ainsi que le Parlement doit bien sûr être mobilisés sur le sujet, c'est je crois l'une des propositions importantes qu'ils font et nous souscrivons totalement à cela car si. Les objectifs de développement ne sont pas partagées par l'ensemble de ceux qui sont les acteurs de l'économie et les acteurs. Politiques de notre pays, je crois que nous n'arriverons pas au bout de nos, de nos peines. Il faut dire que. On a eu l'exemple de de la pandémie où. Beaucoup d'acteurs se sont mobilisés pour produire des masques par exemple dans notre pays. Vincent Segouin dans son propos liminaire l'a évoqué tout à l'heure. le résultat qu'on observe aujourd'hui c'est que la plupart de ces opérateurs sont dans la panade. C'est-à-dire que. Aujourd'hui, nous avons repris nos vieilles habitudes de recourir aux offres les moins chers, les moins cher, c'est bien entendu souvent ce qui vient de Chine et d'autres pays enfin d'Asie. Et donc, tous les opérateurs qui en France se sont mobilisées pour apporter des réponses nationales se retrouvent dans la difficulté et ceci n'est pas acceptable donc il importe que nous puissions apporter des des réponses les réponses seront aussi notamment par une action continue sur la compétitivité de nos entreprises, beaucoup a été fait est engagée par le gouvernement à ce sujet sur la baisse des charges, il faut que l'on continue et je ne partage pas les opinions qui tout à l'heure, ont été mises sur la gauche. Par des orateurs sur le fait que il faille arrêter la baisse des charges. Non il faut qu'on poursuive et en particulier qu'on puisse même les prolonger. Pour ce qui concerne les charges sociales qui constitue un handicap dans la compétitivité. Donc si nous pouvons travailler là-dessus et je formulerait des propositions dans le cadre du débat sur la retraite pour pouvoir substituer. Les charges sociales là à une autre ressource bien entendu et donc on, on voit qu'il y a. Beaucoup à faire là dessus. Voilà donc et puis. Il y a sans doute Monsieur le Ministre, un travail plus approfondi en synergie à mener avec l'ensemble des opérateurs je veux par exemple parler des des régions que la compétence économique. Je suis de Bretagne, nous avons en Bretagne commerce international en région. Mais il ne faut pas que Bretagne commerce international travaille dans son coin, il faut qu'il y ait une stratégie nationale bien définie qui soit élaboré ensemble et ceci doit être le cas dans toutes les régions. Merci de votre attention. Merci cher collègue. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur. J'ai déjà, je pense, répondu à à beaucoup de de 2. Qui. Structuré votre propos. J'aimerais peut-être juste faire. Une assise sur la question de la loi de programmation qui effectivement fait partie des très bonnes propositions qui sont incluses dans le rapport. Je ne sais pas s'il faut une loi de programmation. On est dans un domaine. Où les choses évoluent quand même très rapidement, on le voit aujourd'hui avec une fiche, une réduction Act américain qui vient en plus d'un allié. Traditionnel de. L'Europe et particulièrement monde de pays. En revanche ce qui est certain c'est qu'il faut une stabilité. Des dispositifs et des mécanismes et ça je crois je ne sais pas s'ils sont à inscrire dans une loi de programmation mais en tout cas si on veut véritablement relever le challenge à la fois de la réindustralisation et celui. De porter de PME PMI à l'exportation. On a besoin de dispositifs stable visible Claire et ça je crois que c'est le véritable enjeu sur lequel nous devons aujourd'hui nous engager. Merci.

pour notre pays parce que c'est ça qui est important, il y a bien sûr les acteurs économiques qui sont les principaux opérateurs mais on le voit bien qu'il y a un grand nombre d'intervenants aujourd'hui sur le sujet et que tout le monde n'est pas dans le même ordre de fonctionnement c'est vraiment par cette mobilisation. Je crois par cette loi. La mobilisation de tous, ce que l'on puisse définir là où sont les priorités et que les acteurs. Sur le terrain puissent savoir dès lors. Vers où aller et sur quel soutien ils pourront compter pour pouvoir. Continuer à à à activer. Mais comme on l'a dit tout à l'heure aussi la baisse des charges doit se poursuivre. Il avait engagé, merci. Merci la parole est à Madame, Evelyne Renaud Garabédian pour le groupe Les Républicains pour sept minutes, chers collègues. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre. Mesdames, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Les chiffres relatifs au commerce extérieur sont catastrophiques. Je ne les reprendrai pas ici puisque mes collègues, on en parlait tout à l'heure. Face à cela les plans des gouvernements successifs. Les rapports parlementaires et je tiens à saluer la qualité de votre rapport. Non, absolument pas inverser la tendance car nous n'avons pas appliquer les recommandations en partie car nous dépendons des mouvements internationaux en partie enfin car nous n'avons pas la culture de l'export comme vous l'avez dit, monsieur le Ministre, c'est en réalité sur. Dernier point. Qui à mon sens prend le dessus sur tout le reste je ne reviendrai pas sur les variables macro et micro-économiques du commerce extérieur. Le rapport le fait très bien. Je voudrais revenir sur un seul aspect qui est précisément la façon d'envisager le commerce extérieur qui passe en 1er lieu par l'étranger. Nous avons de grandes entreprises françaises qui exportent sans l'aide de l'État. Elles connaissent les pays, les dirigeants ainsi que les chefs d'entreprise, elles font leurs propres réseaux nous n'avons jamais compté autant d'exportateurs français depuis 20 ans, ils sont près de 140.000 les traditionnelles locomotives Airbus ou LVMH et les grandes entreprises de constitue de manière étonnante que 0,5% des exportateurs pourtant elles pèsent pour 52% de leur valeur, les PME/PMI et TPE qui, je le rappelle, constituent la majorité du tissu économique français représentent plus de 99% des troupes à l'export mais malheureusement seulement 48% de la valeur. Bien que de très nombreuses. Entreprises à l'export performants dans leur secteur respectif souvent de niche, elle n'exporte que de façon très ponctuelle. Faute paraît de maîtriser les règles de l'export, elles ne sont pas anglophone, elle ne se déplace pas, elle ne communique pas l'international et elles n'ont pas de stratégie globale à l'export. Elle constitue pourtant Monsieur le Ministre, la vitrine de la France. Ce sont elles qui ont besoin de nous pour augmenter leur chiffre d'affaires à l'export. Notre objectif doit donc être d'aider nos PME et PMI à généraliser l'exportation pour y parvenir, il faut développer une réelle culture de l'export auprès des étudiants, des futurs chefs d'entreprise avec des formations spécifiques. Il faut que les PME/PMI considère que l'international est une clé dans leur développement au même titre que le marché intérieur. Il faut faire la promotion des outils d'accompagnement à l'export et renforcer la coordination des acteurs Business France Bpifrance les régions. Je rappelle que la Cour des comptes a publié en octobre 2022, un rapport et a constaté que ces acteurs se trouvait dans une situation de de concurrence entre eux et non malheureusement de coopération. Il faut davantage s'appuyer sur une diplomatie économique parallèle que nous n'exploitons absolument pas les entrepreneurs français installés à l'étranger, je ne parle pas des entreprises françaises installées à l'étranger mais bien des des entrepreneurs qui ont créé une entreprise de droit local. Nous avons dans tous les pays du monde, des entrepreneurs français. Ces personnes sont françaises importe des produits et des services français dans leur pays de résidence. Ils connaissent l'économie locale comme personne les marchés qu'il faut exploiter et ce qu'il faut éviter ce sont eux qui créent une entreprise ce sont eux qui qu'on construit et établit des connexions avec des acteurs économiques locaux. Je suis chef d'entreprise et sénateur des Français de l'étranger en contact permanent avec ses entrepreneurs français qui participent au rayonnement de la France et qui peuvent être des puissants relais de croissance à double égard d'une part en facilitant l'export des entreprises. Je viens d'en parler longuement. D'autre part on important massivement des produits et des services français dans leur pays de résidence. Nous devons soutenir ses entreprises pour eux la France. Monsieur le ministre est une marque qu'ils vendent ce que les géants du luxe ont d'ailleurs très bien compris, il n'y a pas un pays au monde. Vous ne trouverez pas une référence à Paris ou une reproduction de la Tour Eiffel d'une baguette ou d'un camembert. C'est la raison pour laquelle je voudrais parler du projet de Label Made by France déjà évoqués par notre collègue et qui vendent et à l'étranger des produits et des services français ce Label vise à valoriser la fabrication, la conception française des produits, des services leur qualité, leur origine le savoir fait français artisanal ou industriel, le respect des normes, le terroir. En un mot l'excellence française. Ces entrepreneurs constitue le réseau des chambres de commerce France Internationale 120 chambres dans 94 pays, sans aucune aide publique. Nous ne les valorisons pas suffisamment. Or, le réseau c'est la base de tout projet entrepreneurial seul. Nous ne faisons rien. Ces chambres devrait être une partie essentielle de toute démarche visant notre balance commerciale. Je soutiens l'ensemble des recommandations du rapport de mes collègues en insistant sur le rôle que pourrait avoir au sein d'une stratégie du commerce extérieur efficace les entrepreneurs français à l'étranger. D'autre part, d'autres l'ont bien compris qui valorise bien plus que nous le potentiel économique de leur diaspora je pars d'ici de la Chine. Je présenterai dans quelques semaines, une proposition de loi visant à valoriser nos entrepreneurs français, cela n'est pas seulement dans leur intérêt, c'est dans l'intérêt de notre commerce extérieur, c'est dans l'intérêt de la France. La bataille de l'export. Ce gagnant pour moi d'abord à l'étranger merci d'autres. Merci cher collègue. Là, Monsieur le Ministre. C'est comme vous voulez, vous pouvez commencer et puis faire votre propos. Après. Bien sûr. merci beaucoup madame la présidente. Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. Votre engagement en ce qui concerne les entreprises françaises. À l'étranger. Nous avons et les entrepreneurs français de l'étranger, il y a nous avons besoin de pour le rayonnement de notre pays, ce sont également des acteurs et des supports pour doper l'exportation française. Et je voulais également vous dire que je partageais Votre analyse sur le rôle central que doivent avoir les chambres de commerce françaises. À l'étranger, il y a nous avons mis en place un pilotage fin de la Team France Export dans lequel nous avons inclus évidemment les CCI françaises à l'étranger, il y y a le Conseil national de l'export mais qui ne se réunissait à peu près qu'une fois par an. L'âge réunit l'ensemble des acteurs de la Team France Export. Tous les mois ou tous les deux mois directement au ministère pour faire le pilotage fin de ces dossiers dont je voulais dire que je partageais évidemment. Votre préoccupation et l'analyse que vous portez dans ce domaine.

j'insisterai sur quelque chose de savoir si on pourrait envisager de discuter en commun et de réfléchir, éventuellement un dispositif d'aide qui pourrait peut-être intervenir. Merci de votre. Merci. Alors la parole est à monsieur Olivier Becht un Ministre délégué chargé du commerce extérieur de l'attractivité des Français de l'étranger. Pour cinq minutes. Maximum. Merci beaucoup madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs. D'abord je voudrais rendre hommage à la qualité du travail. Des parlementaires qui se sont engagés dans ce rapport. Et dire que évidemment je partage le constat et nous le verrons. Une bonne partie des propositions qu'ils mettent aujourd'hui sur la table, j'en profite également puisque. À l'Assemblée nationale, un rapport a elle aussi été rendu la semaine dernière avec le député Charles Rodwell pour rendre également hommage à la qualité de ce travail et je voulais vous remercier, madame la présidente d'avoir rendu ce débat possible ici ce soir au Sénat le jour où nous rendons. Publics les chiffres du commerce extérieur de la France pour l'année 2022. Alors je voudrais simplement parce que c'est une précaution de langage qui me semble tout de même utile parce qu'on on parle de déficit commercial en parlant. Des 164 milliards. Dire que en fait les 164 milliards, c'est la balance des biens et que le, la balance commerciale, c'est aussi la balance des revenus et la balance des services quand on regarde ces deux autres balance on se rend compte que autant. La balance des biens à un déficit extrêmement important qui a doublé par rapport à l'année dernière pour les raisons qu'on a évoqué sur la question énergétique. Mais lorsqu'on regarde la balance des services. Nous avons annexée dans qui lui est aussi un excédent record record puisque nous n'avons jamais eu autant. Nous avons 50 milliards. D'euros, due à la reprise du tourisme du à la dynamique de nos transports est due également aux services financiers puisque nous bénéficions à la suite du Brexit du dynamisme de la place de Paris qui est devenu, il faut quand même le dire, la première place boursière en Europe en matière de capitalisation par action nous avons détrôné la City de temps à autre il faut aussi. Entendre la forêt poussé et pas simplement l'arbre tombé. Donc pour dire que nous sommes. Bon dans le domaine des services et nous sommes également bon dans le domaine des revenus puisque toutes les grandes entreprises qui travaillent, et aussi certaines entreprises françaises de étrangers qui travaillent à l'étranger rapatrient également les revenus en France 30 milliards d'euros d'excédents. C'est quand même. Considérable et là aussi c'est. Un record. Par rapport aux années précédentes et au 10 années précédentes où nous avions à peu près 8 milliards en moyenne sur cette balance. Alors après. Il ne faut pas se satisfaire évidemment de cette situation puisque sur la balance des biens. On est tout à fait d'accord, on a un vrai problème, c'est vrai problème il est lié à l'énergie c'est conjoncturel, nous allons le résorber. Il a et il y a un problème structurel qui est lié, nous l'avons dit dans le débat ce soir, à la fois à la fois à la désindustrialisation de notre pays que nous avons vécu au cours des 30 dernières années et à la faiblesse de nos PME/PMI à l'exportation, comparé à nos grands voisins et donc ce sont dans ces domaines-là qu'il faut agir et qu'il faut agir vite. Si la réindustrialisation que nous avons lancée avec le plan France 2030, 54 milliards d'euros qui sont posés sur la table avec des résultats qui sont déjà ce sont des usines qui se construisent au lieu d'usine qui ferme, ce sont des emplois industriels qui sont créés, ce sont des usines dans les domaines stratégiques que sont les semi-conducteurs comme STMicroelectronics à Crolles, dans le domaine de la pharmacie avec le paracétamol les principes actifs avec avec l'usine séquence dans l'Isère. Ce sont les usines qui se montent également pour raffiner le lithium, que ce soit dans l'Allier ou encore. Dans Dans l'exploitation du lithium dans le Bas-Rhin. Donc il y a de cela un certain nombre de choses qui sont déjà partis et qui sont positives et puis il y a le dernier domaine, qui est évidemment celui sur lequel on on doit agir rapidement également puisque la réindustralisation prendra du temps. C'est la question évidemment de nos PME PMI alors. Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne l'a rappelé tout à l'heure, nous avons déjà une satisfaction puisque nous avons de plus en plus d'entreprises exportatrices. On est passé de 120.000 à 144.400 entreprises exportatrices, l'année dernière ça reste cependant insuffisant par rapport à nos grands voisins et donc il y a une culture de l'exportation, qui doit être inculqué aujourd'hui c'est un c'est un combat mais c'est un combat qui se mène aussi mètre par mètre en demandant aujourd'hui aux acteurs de la Team France Export et particulièrement aux conseiller les chambres de commerce et d'industrie. En plus de ceux de Business France d'aller faire du porte-à-porte auprès de chaque PME que pour faire en sorte que l'on puisse les aider à se projeter à l'exportation sans coup de cas l'engagement que je prends devant vous, en tant que ministre déléguée en charge du commerce extérieur et de l'attractivité. C'est un combat que nous pouvons gagner et c'est un combat que nous gagnerons ensemble, je vous remercie. Merci. Je me permets de vous remercier, monsieur le ministre d'avoir vraiment fait le jeu de ce débat interactif en répondant à tous les orateurs. Merci, merci beaucoup. Alors pour conclure le débat. La parole est à monsieur Serge Babary, président de la délégation sénatoriale aux entreprises. Chris pour cinq minutes.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre. Madame, monsieur les rapporteurs. Mes chers collègues. Merci à chacun d'avoir participé. À ce débat, je pense toujours intéressant et utile pour un tel sujet. Les alertes du Sénat se sont multipliées depuis plusieurs années pour faire prendre conscience de notre dépendance aux importations. Notamment celles provenant d'Asie. Mon collègue Vincent Segouin évoquer les ruptures d'approvisionnement des médicaments si il avait répondu. Je rappelle que la commission des affaires économiques. En 2018 déjà, puis dans son rapport présentant 5 plan pour reconstruire la souveraineté économique souligner cette dépendance en effet l'approvisionnement de la France en ingrédients pharmaceutiques actifs provient à plus de 80% de Chine et d'Inde. évoqué dans un débat précédent aujourd'hui même le sujet des véhicules électriques et le même constat de dépendance aux importations asiatiques pourraient être dressée dans le cas des semi-conducteurs. Avait également répondu. Or les travaux de mes collègues de la délégation aux entreprises montrent clairement que les études sur les vulnérabilités les approvisionnements de la France minimise les risques encourus. Qu'il s'agisse des publications de la direction générale du Trésor ou du Conseil d'analyse économique. Elle s'appuie sur des données qui ne permettent pas de distinguer les différents un trend de la chaîne de valeur des biens importés. Ainsi par exemple un bien importés d'Allemagne n'est pas jugé risqué car il est identifié comme provenant de l'Union européenne même si il dépend de composants importés exclusivement de Chine. Il me semble, Monsieur le Ministre, ce que nous ne pouvons plus nous contenter d'une analyse qui minimisent autant les risques alors que les récentes crises ont montré aux Français les conséquences des délocalisations massives de nos sites de production, il faut mobiliser la Commission européenne pour que les données des États permettent d'appréhender collectivement la réelle dépendance de nos économies européennes. Comme souvent, il existe un décalage entre la perception de l'administration de l'État et la réalité économique vécue sur le terrain par les entreprises et les citoyens. Cette même des connexions et ressenties par les entreprises face à la complexité des normes qui leur sont applicables. Elles ne cessent de se multiplier au point de détourner les dirigeants de leur coeur de métier et plombé notre compétitivité. En matière de commerce extérieur, nous l'avons vu en Italie, en Allemagne les ETI sont un véritable atout. Pourtant, en France comme le Mouvement des entreprises de taille intermédiaire le rappeler récemment devant notre délégation 700 de nouvelles normes s'impose aux ETI. Chaque année, chaque année, en plus du stock de 400.000 normes existantes. Ce qui représente un coût total de 28 milliards d'euros pour nos ETI. La simplification des normes est un enjeu central pour le commerce extérieur et je ne doute pas que vous suivrait avec attention les conclusions de notre mission d'information actuellement en cours sur le sujet au sein de notre délégation on vous fera part de nos conclusions. Le redressement du commerce extérieur dépendra des efforts déployés par chaque ministère, chaque acteur, publics ou privés de l'écosystème. Les grandes entreprises devront apprendre à chasser en meute avec les PME. Les acheteurs publics devront prendre exemple sur nos voisins européens est dépassé, le critère du moindre coût pour ne plus défavorisés les TPE et PME françaises. Bref, nous avons tous un rôle à jouer. La désindustrialisation a produit un cercle vicieux car nous n'avons pas su ou pas voulu en mesurer les conséquences dans tous les domaines ayant un impact sur notre compétitivité, chômage endémique, affaiblissement de la compétence et l'innovation ça été rappelé. Il nous faut désormais nous doter d'une structure capable de piloter efficacement notre stratégie. Ce que nous proposons avec la rénovation du conseil stratégique de l'export. Le gouvernement doit enfin entendre l'appel du législateur qui réclame depuis longtemps de véritables études d'impact en amont des projets de loi prenant en compte tous les effets des politiques publiques qu'il s'agisse de formation de fiscalité ou de normes environnementales. Il est temps de permettre aux entreprises de développer leur talent à l'étranger mais aussi dans nos territoires en leur offrant enfin un écosystème favorable, je vous remercie. Alors, mes chers collègues, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 22h 05 hein pour le débat sur les conclusions du rapport compétitivité une urgence pour redresser la ferme France et la séance est suspendue.